la nuit de la séance de ce jour et inscrire la suite de l'examen de cette proposition de loi à l'ordre du jour du jeudi 16 mars à l'issue d'espace réservé au groupe RDSE et le soir. Y a-t-il des observations. Je n'en vois pas, il en a donc été ainsi décidé l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi organique visant à permettre à Saint-Barthélemy, de participer à l'exercice des compétences de l'État propositions présentées par Madame Micheline Jacques et c'est une demande du groupe Les Républicains et conformément à l'article L O 62 13 3 du code général des collectivités territoriales, le Sénat a consulté le conseiller territorial de Saint-Barthélemy sur cette proposition de loi organique dans la discussion générale. La parole est à l'autrice de la proposition de loi Madame Micheline Jacques.

Madame la présidente, madame la Ministre, chers collègues, cette proposition de loi organique vise à doter la collectivité de Saint-Barthélemy, de la faculté de participer à l'adaptation des règles destinées à favoriser la continuité des soins à Saint-Barthélemy. Il s'agit d'un sujet épineux qui préoccupe la population. Je tiens à remercier les rapporteurs nos collègues Valérie Boyer, Alain Milan pour leur implication et l'intérêt qu'ils ont montré pour ce texte qui n'était pas évident, il faut bien l'admettre. Le dispositif initial visait à permettre à la collectivité de Saint-Barthélemy, de participer à la compétence de l'État en matière de sécurité sociale. En effet, bien que cristalliser sous le terme de santé. Le véritable enjeu est celui du financement pour assurer la continuité des soins dans un contexte insulaire et de surcoûts engendrés par la petite taille de Lille et son économie. Le texte le présent texte s'inscrit dans le cadre de l'article 74 de la Constitution qui permet aux collectivités d'outre-mer doté de l'autonomie de participer aux compétences conservés par l'État. Cela permet de mieux prendre en compte les réalités locales dans des matières dont il doit rester le garant de la cohésion. Cette proposition de loi organique s'inscrit en outre dans la continuité du principe de maîtrise de sa destinée qu'a présidé à l'érection de Saint-Barthélemy en collectivité d'outre-mer. Elle a ainsi toujours été à l'initiative de mesures d'adaptation à sa réalité tout en ayant une relation très harmonieuse avec l'État. Mon prédécesseur Michel Magras ancien président de la délégation aux outre-mer avait lui-même porté en 2015 la demande d'une plus grande implication de la collectivité dans la définition de la politique de protection sociale en déposant 2 propositions de loi organique et ordinaire. La même année avait été créée, la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. La nouvelle majorité n'a du reste pas fait exception à ce principe en créant une commission ad-hoc diagnostic territorial de l'offre de soins sujet incarné depuis avec une implication et une énergie sans faille par la première vice- présidente certes aucune collectivité d'outre-mer n'a jusqu'à présent, participé à la compétence de l'État en matière de sécurité sociale et une fois de plus Saint-Barthélemy propose d'innover comme elle l'a fait déjà, avec plusieurs dispositifs. Ainsi, elle est la seule collectivité avoir renoncé au FCTVA de même que l'émission du SDIS et de la MDPH assurée par des services de la collectivité en lieu et place d'un établissement public et d'un GIP. Ce texte ne se vaut pas une révolution mais vise à utiliser les outils d'adaptation offert par le statut de collectivité d'outre-mer doté de l'autonomie. Il porte une demande. Qui n'est pas nouvelle. Depuis plusieurs années, les élus ont alerté le gouvernement sur la dégradation de l'offre de soins en particulier hospitalière qui a connu une accélération ces derniers mois. Le coût de la vie, en particulier les niveaux de loyer vertigineux combinées aux difficultés du quotidien, sur un territoire de 21 km2 contraignent la mise en oeuvre des politiques publiques. Fidéliser les médecins hospitaliers pour permettre un fonctionnement de l'hôpital continuent requiert de tenir compte de ce contexte. Lille est doté d'un établissement de proximité, l'hôpital De Bruyne et pour les cas les plus graves dépendante des évacuations sanitaires vers les centres hospitaliers de Saint-Martin 80 pour des évacuations de la Guadeloupe ou de la Martinique, avec une piste trop courte pour permettre à des aéronefs de plus de 20 places d'atterrir. Ces évacuations sont prises en charge sur le budget de l'hôpital ne pouvant pour cette raison être effectués sur des lignes régulières. Elle pèse sur les dépenses hospitalières. Ainsi en 2022 194. Évacuation été réalisés pour un coût de 600.000 euros pour l'hôpital pour une dotation de 420.000 euros. L'impossibilité d'atterrir de nuit et l'autre contrainte des évacuations sanitaires. Dès lors, lorsque l'hôpital fonctionne au sous-effectif au delà d'un certain nombre d'évacuations sanitaires il n'y a plus de Metz et urgentistes présents. Il s'agit donc de disposer sur place des ressources médicales. Chaque fois que cela est possible. Ce n'est pas la taille de la population mais les besoins et les risques qui doivent être des critères de définition de l'offre de soins. Je veux ici rassurer le Sénat et le gouvernement, l'attachement au principe de solidarité n'est pas remis en cause en effet la présente, proposition de loi organique ne vise en aucun cas allié capacité contributive et dépenses de santé mais à les ajuster aux besoins réels. La population de Saint Barthélémy est en droit d'attendre une offre de santé aussi large que possible. Sur un petit territoire insulaire surtout depuis 10 ans le projet politique s'est bâtie sur l'existence d'un excédent des comptes territoriaux que jamais personne n'a pris la peine d'infirmer sachant pourtant que les élus sont prévalait. le budget de l'hôpital affiche une dépense de 251.000 euros annuels pour loger des personnels en déficit d'attractivité ils recrutent difficilement des intérimaires peut impliquer la probable, adoption du texte dit Rist annonce par surcroît une contrainte supplémentaire pour ses recrutements durant plusieurs années, l'hôpital de bruit n'a fonctionné, disons-le, selon une organisation propre aux médecins de Lille. Mais le retour légitime aux règles de droit commun de fonctionnement de n'était établissements hospitaliers a conduit au départ de la quasi-totalité quasi-totalité des médecins hospitaliers basé à Saint-Barthélemy. La réalité de l'île est aussi celle du laboratoire de biologie médicale qui n'est plus aux normes d'accessibilité notamment qui a besoin de s'agrandir mais ne peut supporter à loyer multiplié par 3. La CPS, quant à elle est en réalité un démembrement de la MSA Poitou qui a permis d'amener un service de proximité jusque-là inexistant à Saint-Barthélemy doit pouvoir comme les autres collectivités d'outre-mer qui le souhaitent, disposer de sa caisse propre même sans qu'elle soit autonome. De plus, l'absence de personnalité morale de la CPS pose 2 questions majeures, d'abord celle de la fiscalité des pensions de retraite du régime général. D'autre part celle de l'efficacité du recouvrement 10 distant des cotisations comme en attestent les chiffres. Sur une île comme Saint-Barthélemy au regard de son niveau d'activité économique plus 97 millions d'payer de cotisations que nous découvrons, c'est inadmissible. Plusieurs pistes ont découlé du diagnostic lancée par la majorité actuelle. Le partage de la compétence santé par le biais d'une agence territoriale de la santé, la construction d'un pôle hospitalier qui regrouperait l'hôpital des logements le laboratoire. Une maison de santé accueillant des spécialistes ponctuellement la nomination de coordinateur de santé. Or la réglementation de la santé stricto sensu ne pose pas de difficulté à Saint-Barthélemy c'est l'organisation et le financement des soins. En particulier hospitaliers qui doivent être mieux adaptées, pour prendre en compte les réalités incompressible de Lille comme le coût de la vie et les contraintes de l'insularité. Le projet ambitieux à l'échelle de l'île de construction d'un hôpital est à l'étude. Or, je suis convaincu que la structure n'est pas le problème. Pas plus qu'elle ne le résoudra la restructuration de l'offre hospitalière doit être pensé en tenant compte de l'achèvement prochain d'un hôpital dernière génération en Guadeloupe. L'idée de développer le tourisme médical de luxe a également été évoquée au cours des travaux préparatoires, mais elle est inadaptée à la clientèle de Saint-Barthélemy. Je ne peux m'empêcher d'évoquer la querelle qui oppose la collectivité à la direction hospitalière s'agissant de la propriété du foncier. Le terrain sur lequel est construit l'hôpital De Bruyne a une dimension patrimoniale collective pour les habitants de Saint-Barthélemy, où l'État est arrivé tardivement. L'ancien président Bruno Magras avait proposé que les 4 millions 7 alloués par le Ségur de la santé soient plutôt affectés au fonctionnement véritable ne laissant à la collectivité le soin de financer les investissements dans son sillage les nouveaux élus sont prêts à réaliser les investissements afin de rénover le bâtiment mais estime que la collectivité ne peut investir tant que le foncier ne lui aura pas été transmis et c'est une demande que je relaie avec mon soutien. La collectivité c'est régulièrement impliqués dans l'amélioration des soins le scanner a certes été offert mais elle découle d'un choix stratégique du président, Bruno Magras orientant la générosité vers des équipements médicaux, Il en a été de même pour l'acquisition de mammographes ou encore la construction d'Nepad, mis à disposition de l'hôpital de même que la buanderie et la cuisine concourant ainsi à alléger les charges de fonctionnement de l'hôpital et de la sécurité sociale qui économise pour chaque examen le coût d'un aller retour à Saint-Martin. Aujourd'hui la collectivité bien que prête à faciliter le logement du personnel hospitalier et enseignants ne dispose pas d'un parc de logement suffisant et des constructions ne pourront être achevés avant. 2 voire 3 ans. Le Sénat a bien compris ma démarche en considérant que la voix par la voix du rapporteur Alain Milon. Que la présente PPL au propose une avancée. Par ce qui s'apparente à un droit de propositions de la collectivité avec une pertinence qui ne, qui ne surprendra personne. Les rapporteurs ont apporté des modifications au dispositif initial. Pour parvenir à un équilibre qui crée aussi les conditions de l'indispensable prise en compte de la volonté locale par l'État. L'expérimentation sur une durée de 5 ans laissera le temps d'évaluer l'intérêt de cette nouvelle faculté offerte à la collectivité. Cette majorité pourra s'en saisir ou la prochaine, le cas échéant, j'en terminerai avec cet extrait du rapport de Michel Magras sur la différenciation. L'État doit désormais accompagner les collectivités ultra-marines pour nourrir leurs capacités propres d'expertise et leur garantir une véritable autonomie qu'elles peuvent mettre au service de leur développement endogène. Cela vaut dans tous les domaines. Je vous remercie. Madame la présidente, madame la ministre. Monsieur le président de la commission des lois. Chers collègues, et en particulier cher Micheline Jacques autrice de cette proposition de loi. La proposition de l'organique que nous examinons aujourd'hui entend répondre à un problème qui mérite toute notre attention. Je veux parler des inacceptable difficultés rencontrées au quotidien par nos compatriotes ultramarins et ceux de Saint-Barthélemy dans l'accès à une offre de soins complète et adaptée aux particularités de leur insularité l'île de Saint-Barthélemy et situé à 25 kilomètres au Sud-Est de Saint-Martin au Nord-Ouest de la Guadeloupe continentale et 6500 kilomètres de Paris, elle est très dépendante des territoires voisins de Saint-Martin et de la Guadeloupe pour la prise en charge des cas graves, c'est complexe. Le problème est pourtant connue de longue date. Les élus locaux et particulièrement les sénateurs de Saint-Barthélemy notre ancien collègue Michel Magras. Ce qui a été cité par Micheline Jacques et aujourd'hui Micheline Jacques qui lui succède ont régulièrement alerté sur le manque d'adaptation des règles nationales aux réalités locales et sur la dégradation de l'offre de soins préjudiciable aux habitants de l'île. Lors des auditions menées avec Alain Milon, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Nous avons pu constater que les difficultés rencontrées par les habitants et les personnels soignants persistait aujourd'hui encore été de 4 ordres. Premièrement certaines prestations et actes pourtant indispensables au quotidien d'un hôpital ne sont aujourd'hui pas réalisé sur l'île, en particulier le dépôt de sang. Deuxièmement, les services de soins font face à des difficultés techniques et opérationnelles qui nuit à la prise en charge optimale des assurés de Saint-Barthélemy ainsi faute d'éclairage les pistes des aérodromes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les évacuations sanitaires ne peuvent avoir lieu la nuit. Troisièmement des obstacles réglementaires empêchent la pleine adaptation de l'offre de soins au territoire, et ce malgré les demandes répétées des élus comme des acteurs locaux de la santé. En effet, la pharmacie de l'hôpital. Irénée de bras ne peut aujourd'hui en application d'une disposition réglementaire national être gérées que par un pharmacien universitaire alors que cette pharmacie ne dispose que de 10 lits, faute d'adaptation de cette règle réalités locales. L'activité de la pharmacie hospitalière est aujourd'hui menacée. Quatrièmement, les services de soins peinent aujourd'hui à fidéliser les praticiens hospitaliers sur le territoire en raison d'une part des contraintes d'exercice sur ce territoire et d'autre part du coût exorbitant des logements pour ces derniers, cela a d'ailleurs été développée par notre collègue Micheline Jacques la présente, proposition de loi apporte donc une première solution pragmatique et équilibré à cet ensemble de difficultés en prévoyant de confier à la collectivité de Saint-Barthélemy un pouvoir de propositions, dans les domaines de l'assurance maladie et du financement des établissements et services de santé qui relèvent de la compétence de l'État. Reposant sur une approche ascendante que je sais, cher à notre assemblée cette proposition opère un point d'équilibre satisfaisant entre exigences d'adaptation des normes aux réalités locales trop longtemps attendu et et la nécessité de conserver un cadre garant des grands principes de la sécurité sociale sur l'ensemble du territoire national. Lors de l'examen en commission des lois, nous avons retravaillé cette proposition afin de recourir à l'expérimentation pour cette modification certes limitée mais novatrice du partage des compétences en matière de santé entre l'état et la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy. D'une durée de 5 ans une telle expérimentation permettra de mesurer les effets de ces dispositions et de les évaluer. Avant d'en envisager la pérennisation. Ces outils doivent être pleinement mobilisé tant ils permettent une réelle différenciation des normes et particulièrement pour les territoires comme les outre-mer qui doivent trouver dans notre cadre juridique des moyens concrets d'une adaptation des normes nationales à alors réalité si spécifique. Ainsi, il importe que la collectivité puisse disposer de nouvelles procédures organique pour renforcer la prise en compte par l'état des spécificités de l'île sans pour autant Bertrand brèche le principe d'une compétence étatique en la matière. C'est pourquoi nous avons à l'occasion du travail en commission souhaité renforcer les garanties applicables en la matière aux initiatives qui seraient ainsi prises par la collectivité. À ce stade de mon propos, je me dois néanmoins chers collègues d'être franche. Si cette proposition de loi marquent une première avancée salutaire, elle ne pourra à elle seule régler l'ensemble des difficultés rencontrées sur l'île en matière d'offre de soins. Et je dois malheureusement déplorer l'inertie de l'État sur ce sujet. À titre d'exemple, suite à l'expérimentation concluante visant à accorder aux directeurs généraux d'agences régionales de santé un pouvoir de dérogation pour adapter certaines normes aux réalités locales sur leur territoire expérimentation lancée dès dès 2017. Le gouvernement s'est engagé en novembre 2021. À la pérenniser en généralisant ces dispositions à l'ensemble du territoire national. Comment expliquer alors même que l'ensemble des élus et des acteurs locaux de la santé que j'ai auditionnés ont souligné l'importance de ce décret pour améliorer l'offre de soins Barthélémy et leur souhait de s'en saisir. Sans plus attendre que le gouvernement n'est toujours pas pris le décret pourtant annoncé. Madame la Ministre, l'État se doit de se montrer à la hauteur des enjeux et de jouer pleinement le rôle qui lui incombent en la matière. Vous pouvez compter sur notre vigilance et j'espère que nous aurons une date de parution du décret. Pour finir, si c'est un point sur lequel je souhaite insister tout particulièrement, nous avons dû mener ses travaux sans disposer des conclusions d'un rapport demandé par le Parlement il y a plus d'un an sur l'organisation du système de santé et la sécurité sociale à Saint-Barthélemy et ce sans disposer des chiffres de la consommation de soins pour les assurés de Saint-Barthélemy, que le gouvernement s'obstine à ne pas publier c'est non seulement incompréhensible mais c'est pas acceptable pour le législateur que nous sommes et élu le peu de considération portée par le gouvernement à notre endroit lorsque on demande ces chiffres, hé bien la moindre des choses c'est de les avoir comment exercer notre rôle dans ces conditions. Malgré ses remarques de méthode la présente, proposition de loi n'en reste pas moins nécessaire et je souhaite pour finir remercié Micheline Jacques auteur de cette proposition de loi et mon collègue Alain Milon, rapporteur pour avis que j'ai retrouvé à l'occasion de ces travaux effectués en commun. Comme il y a bien longtemps. Ce texte est équilibré négociée consensuelle, il me semble à même d'emporter sur un sujet d'une particulière importance une large adhésion aujourd'hui. Avant tout remercier. J'espère que le gouvernement accompagnera favorablement et soutiendra ce texte qui est écrit qui ait pensé qu'il a été auditionné qui a été imaginé par notre collègue Micheline Jacques en faveur des territoires ultramarins et de Saint-Barthélemy, en particulier, comme cela a été souligné, c'est un texte équilibré. Aussi j'espère et j'ai confiance dans le fait qu'ils recrutent qu'il recueillera votre assentiment. Je vous remercie. Merci la parole est maintenant à monsieur Alain Milon, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.

madame la présidente. Madame la Ministre, monsieur le président de la commission des lois. Madame la rapporteure chers Valérie Boyer. Mes chers collègues Saint Barthélémy n'est pas ce qu'on désigne parfois sous la désignation un peu malheureuse de désert médical mais des lacunes persistantes sont identifiés en matière de santé. Certaines spécialités médicales ne sont pas représentés sur l'île comme la cardiologie par exemple où sont d'un accès limité. L'offre hospitalière et fragile surtout puisque l'hôpital qui compte 10 lits de médecine de courte durée et le seul établissement de santé de médecine. De Lille et une peine à garantir l'effectivité des postes ouverts et à recruter notamment des urgentistes en nombre suffisant. C'est le cas un peu partout en ce moment. Malheureusement, c'est d'ailleurs là une des préoccupations de notre collègue, auteur du texte, qui alertent sur les ruptures dans la continuité des soins. L'actrice, l'attractivité médicale et comme ailleurs en France, une préoccupation majeure, alors que le coût des logements sur l'île est assurément incompatible. Avec les rémunérations proposées ou les moyens d'hôpital. Au delà de l'offre présente ainsi bien davantage l'offre manquante sur laquelle les élus ont régulièrement interpellé le gouvernement et continue de le faire aujourd'hui alors que le territoire est dépendant de Saint-Martin et de la Guadeloupe pour assurer la prise en charge des patients dans les cas les plus graves et particulièrement les urgences, les évacuations sanitaires les fameuses Hassan cristallise pour partie des revendications maintenant ancienne. Ces évacuations au nombre de 183 en 2022, doivent se faire par voie aérienne et sont parfois compromise. Les pistes des aéroports de Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont impossibles à utiliser la nuit alors que l'utilisation d'hélicoptères venant de Guadeloupe réduit les moyens de l'archipel pour plusieurs heures. Une étude est annoncé sur ce sujet. Mais le problème est identifié depuis 20 ans. Ces différents sujets comme d'autres problématiques d'inadaptation. De droit commun à la configuration de l'île de Saint-Barthélemy tarde à trouver des réponses. Je pense ici à la prise en charge de ces. Au regard des lignes régulières disponible mais aussi à la question du dépôt de sang Valérie Boyer en a parlé sur le territoire par exemple pour partie. Ces problèmes pourraient trouver une réponse de la part des services de l'État, un décret en Conseil d'État a été maintes fois évoqué, mais toujours pas publié. Je rappelle que la commission des affaires sociales avait à la suite de la mission à Mayotte en 2022. Appelée à donner aux directeurs généraux des agences nationales de santé outre-mer des pouvoirs de dérogations accrue pour adapter le droit aux réalités ultramarines. Faut-il encore que les textes réglementaires suivent et répondent aux domaines. Aux demandes des services sur place. Or on constate trop souvent une inertie. Je ne dirais pas du gouvernement mais des gouvernements inertie des gouvernements pour apporter des solutions concrètes aux problèmes posés par l'insularité ou l'éloignement de ces territoires à titre d'exemple, le rapport prévu par la loi 3DS. Sur l'organisation des soins outre-mer en particulier à Barthélémy qui n'a pas été produit à ce jour plus de 6 mois après l'échéance prévue. de notre collègue Micheline Jacques se présente donc aujourd'hui comme un moyen d'apporter des solutions à des problèmes structurels qui appelle des réponses urgentes et durable par cette participation à une compétence de l'État. Il est ainsi organisé ce que nous pourrions qualifier de droits de proposition formelle de la collectivité à l'adresse de l'État en laissant ce dernier à ce dernier la pleine compétence. J'insiste sur ce point, auquel la commission des affaires sociales et très attaché la santé comme la sécurité sociale demeure et doivent demeurer les compétences de l'État. Il n'y a ici ni transfert ni partage proposé. J'ai d'ailleurs en commission insisté sur le fait que de telles revendications ne saurait être recevable au motif que certains territoires serait hypothétiquement contributeurs nets pour la sécurité sociale et s'il est nécessaire que les territoires puissent intervenir et proposer des adaptations locales au droit commun. C'est à l'État d'assurer et d'assumer ses responsabilités. Pour une île comme Saint Barthélémy, ce principe est d'autant plus fondamentale que l'offre de soins ne peut se concevoir qu'en cohérence avec l'offre de soins disponible à Saint-Martin et ou en Guadeloupe, où un nouveau CHU je rappelle et d'ailleurs en construction, C'est en ayant à coeur d'accompagner l'amélioration nécessaire de le site du système de santé de Saint-Barthélemy en assurant la cohérence de l'offre de soins. À l'échelle régionale et la continuité de la prise en charge des patients que la commission des affaires sociales et à la commission des lois vous propose cette proposition de loi et vous propose de l'adopter, sous réserve d'une transformation du dispositif proposé sous la forme d'une expérimentation. Je vous remercie. Merci la parole est maintenant à Madame. Agnès Firmin Le Bodo, ministre. Délégué chargé d'organisation territoriale et des professions de santé Madame la Ministre, vous avez la parole. Madame la présidente madame la rapporteure. Monsieur le rapporteur pour air ravi. Monsieur le président de la commission des lois, mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs. Votre hémicycle examine cet après-midi une proposition de loi visant à permettre à la collectivité d'outre-mer Saint-Barthélemy, de participer à l'exercice de compétence de l'État. Votre chambre est bel et bien la représentante et le porte-voix si vous me permettez cette expression de tous les territoires dans leur diversité. Le débat qui nous occupe aujourd'hui, il y a donc toute sa pertinence. Il permettra, je l'espère, de lever les incompréhensions qui pourraient persister et apporter des réponses aux interrogations. C'est en tout cas la volonté qui est la mienne et celle du gouvernement. Cette initiative sénatoriale s'inscrit parmi les travaux du Sénat dans une histoire, celle d'une préoccupation légitime des parlementaires, que vous êtes face aux difficultés et inquiétude de nos compatriotes ultramarins. C'est toute l'action portée par Michel Malgras et qui se poursuit dans vos travaux d'aujourd'hui. Cette proposition de loi de la sénatrice Micheline Jacques en est l'illustration. Avant de revenir au texte même qui est en débat aujourd'hui. J'aimerais revenir sur plusieurs points évoqués lors de vos débats en commission. Vous avez regretté le manque d'adaptation des règles nationales aux réalités locales ainsi qu'une dégradation de l'offre de soins. Au delà votre commission a déploré un engagement financier en suffisamment de l'État et la persistance de difficultés rencontrées par les habitants et les personnels soignants. Je souhaiterais attirer l'attention de votre hémicycle sur quelques points. Le rapport de la commission souligne les difficultés des services de soins en matière d'évacuation sanitaire les Éva Sam faute d'éclairage des pistes, des aérodromes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ce qui entraînerait une perte de chance pour les patients. Sur ce point spécifique, je puis déjà vous dire que l'aéroport de Saint-Martin Grand-Case est tentant d'être équipés, sous l'égide du préfet pour permettre au courant 2023 des atterrissages de nuit. Par ailleurs, une étude est actuellement en cours, elle vise à examiner les possibilités de recours à un hélicoptère pour assurer les trajets entre les 2 îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et améliorer le marché et va à Nancy en vigueur. Des conclusions de cette étude seront connus en mai, ce qui permettra d'avancer avec l'ensemble des acteurs concernés et de résoudre cette difficulté réelle que vous évoquez. Il a également été souligné que les modalités de réalisation de certaines prestations et actes comme le dépôt de 100 rencontrent des difficultés alors qu'elles sont indispensables au travail quotidien des personnels soignants et à la qualité des soins. Face à ces problèmes du quotidien rencontrées par nos concitoyens. Il nous faut de trouver des solutions concrètes et apporter de la souplesse. La parution d'un décret en Conseil d'État permettra l'adaptation des modalités de fonctionnement de l'offre de soins aux spécificités locales grâce au futur pouvoir de dérogation du DG de l'ARS. C'est dans ce cadre également que certains obstacles réglementaires que vous évoquez, comme celui qui concerne la pharmacie à usage intérieur du CHU de Bruyne ou le fonctionnement des urgences. Sur l'île pourront être levées. Je souhaite par ailleurs m'inscrire en faux sur le peu de considération supposer que porterait le gouvernement à la situation de cette île. À ce titre, il faut rappeler que face à la tragédie qu'a constitué l'ouragan Irma en 2017 la collectivité de Saint-Barthélemy avec celle de Saint-Martin a bénéficié pleinement de la solidarité de l'État et de la sécurité sociale. L'enveloppe globale s'agissant du soutien face aux conséquences de Lourdes Regan Irma a présenté près de 500 millions d'euros pour Saint-Martin et Saint-Barth Emilie, soit 11.000 euros par habitant. En outre, l'État a également soutenu les entreprises en facilitant le déclenchement du dispositif d'activité partielle et en proposant un moratoire sur les charges sociales patronales. Lors de la crise du Covid, les, l'État a également pris toute sa part dans le soutien aux entreprises de ce territoire. Il a assez ainsi verser près de 1,4 millions d'euros d'aide au paiement des cotisations. Vous le voyez face aux difficultés rencontrées. L'État est au rendez-vous et compte poursuivre cet engagement, je peux vous l'assurer, madame la rapporteur. Je voudrais également revenir sur la situation globale de l'offre de soins à Saint-Barthélemy et évoqué les excédents supposé des comptes de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, comme le laisse entendre l'exposé des motifs de cette proposition de loi. Il faut d'abord rappeler que les flux de cotisations et de prestations versées sont centralisées au niveau des caisses nationales de Sécurité sociale et en particulier de la et de la Caisse centrale de la MSA puisque le principe de solidarité s'applique. Il n'existe donc pas d'autonomie financière des caisses locales dans le sens où elles ne peuvent pas décider librement de l'allocation de leurs recettes de cotisations. Concernant Saint-Barthélemy la caisse MSA du Poitou retrace dans un petit spécifique, les retraites et les dépenses relatives à sa gestion de la sécurité sociale dans l'île. Mais la CPS elles-mêmes ne retrace pas toutes les dépenses de santé, en particulier les dépenses des établissements sociaux et médico-sociaux ou certains types d'aide apportée aux professionnels de santé échappe à son Champ de compétences. Ainsi le coût de financement du centre hospitalier de bruine et des et Hassan qui s'élève à 8,5 millions d'euros et presque entièrement financier via des dotations de l'ARS. De même la CPS ne prend pas en charge toutes les recettes car elle ne gère pas tous les cotisants de Lille en raison de la complexité de certains dispositifs. En outre, les dépenses de gestion de la CPS et d'autres dépenses, comme celles liées aux échanges de données ne sont pas prises en compte. Quelques chiffres pour illustrer mon propos. Concernant la branche maladie, le montant des prestations versées s'élève en 2021 à 18,15 millions d'euros dans le même temps les cotisations maladie plus la CSG du avoisine les 19 millions d'euros. Ce dernier chiffre est à mettre en regard avec les dettes de cotisation restant impayés auprès de la Caisse Générale de Sécurité sociale de Guadeloupe qui s'élève à 66 millions d'euros. Cette situation budgétaire complexe trouve son explication dans la multiplicité des plans de soutien liées aux différentes crises climatiques et sanitaires auxquelles a été confronté sans Barthélémy. Loin de moi la volonté d'insister sur ces éléments chiffrés, mais il était nécessaire de rappeler que Saint Barthélémy a bénéficié et bénéficiera encore si le besoin s'en faisait sentir de la plénitude de la solidarité nationale. Vous évoquez légitimement la remise d'un rapport sur l'organisation du système de santé et de la sécurité sociale à Saint-Barthélemy. Je peux désormais déjà vous annoncer qu'il sera transmis au Parlement d'ici le mois d'avril. Il sera l'occasion de clarifier ses données chiffrées sur lesquels le dialogue a peut-être manqué de clarté ces dernières années. Le gouvernement ne partage donc pas le postulat qui est à l'origine de cette proposition de loi et la volonté d'autonomisation de la sécurité sociale qui en découle. Et ce même dans le cadre de l'expérimentation proposée par la Commission. Cette démarche se heurte à nos principes de solidarité et d'égalité entre les citoyens qui fondre notre système de sécurité sociale, elle appelle néanmoins des réponses concrètes et rapides aux besoins d'accès aux soins des habitants de Saint-Barthélemy. En effet, le gouvernement souhaite rappeler que différents outils offre déjà à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy, la possibilité d'intervenir pour améliorer l'offre de soins sans qu'il soit nécessaire de recourir à une faculté de compétences partagées. Je pense à sa participation au conseil de surveillance de l'ARS Guadeloupe dans laquelle est inclus Saint-Barthélemy et à l'élaboration du projet régional de santé d'ici la fin de l'année 2023. Je pense aussi à la faculté. Depuis la loi 3DS de participer volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé. En définitive, est d'abord à travers des évolutions institutionnelles que nous répondrons ensemble aux avancées très concrètes dont Barthélémy a besoin pour améliorer l'accès aux soins. Le gouvernement est déjà pleinement engagée dans ses travaux et ils sont nombreux en faveur de l'accès aux soins ça Barthélémy. Je n'en citerai que deux. Une étude a été lancée sur la mise en place à Saint-Barthélemy d'un centre de périnatalité de proximité afin de sécuriser la prise en charge avant transfert des parturientes à Saint-Martin. Un projet de restructuration du CHU du CH de Boeing pour améliorer le fonctionnement de ces services est également à l'étude avec 4 7 millions d'euros de crédits issus du Ségur de la santé. C'est une structure de proximité appréciée des habitants et dont il faut accompagner la modernisation et l'efficacité des soins qui sont prodigués. Est-il réellement nécessaire de construire un nouvel hôpital. Au-delà je souhaiterais conclure mon propos en soulignant que la santé constitue un axe majeur de la méthode de refondation voulu par le président de la République. Après une première phase territorial qui s'est achevé en décembre dernier la nouvelle étape du CNR en santé a bel et bien vocation à rentrer dans le coeur des solutions. François Braun et moi-même auront l'occasion de revenir sur sa déclinaison pour construire des solutions adaptées. Au coeur de la fiche de l'Office d'application du CNR. Le droit de dérogation aux normes réglementaires constitue ainsi un levier d'action puissant à même d'apporter des réponses aux besoins de santé spécifique de Saint-Barthélemy. Comme de l'ensemble des territoires. Le comité interministériel des outre-mer qui se tiendra le 19 mai est également un rendez-vous essentiel pour apporter des réponses concrètes et forte aux besoins de santé du territoire d'ores et déjà nous travaillerons avec le ministère de l'Outre-mer et l'auteur de cette initiative pour construire ensemble des solutions pérennes. Je vous remercie. Merci. Dans la suite de la discussion générale. La parole est à Monsieur Victorin Lurel pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, et pour 9 minutes. Madame la présidente. Madame le la ministre. Monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, chers collègues. J'avoue que je suis un peu gêné pour commencer ce discours après avoir entendu notre ministre. Puisque ça remet en cause tout ce que j'avais comme a priori favorable. Et puisque j'ai entendu égréner un ensemble de chiffres pour dire puisque. Il y a pas d'autonomie il y a pas de différenciation et en comptabilité et que on ne peut pas savoir exactement quels sont les résultats des différentes caisses mais j'ai quand même cru entendre que la Caisse assurance-maladie, caisse. Maladie serait légèrement excédentaire, 10, 12 millions de recettes 18 millions. De divorce mais qu'il y a une dette de 70 millions. Et que pour autant pour la première fois qu'une collectivité. Oh non, si j'ose dire. De principe presque sacré à savoir la solidarité. Nationale demande à participer à financer à la place de l'État et qui ne se défausse pas. Hé bien vous refusez. C'est assez étonnant. Alors que moi j'étais tout à fait satisfait et je ne suis pas le seul ici du travail fait par la commission des affaires sociales. J'ai entendu les avis c'est un excellent travail fait précisément pour trouver le bon périmètre. Et si j'ose dire la pertinence du dossier. Non, le gouvernement vient nous dire j'ai agi. J'ai toujours agi et je vais mettre un hélicoptère s'en fait moi j'ai été 10 ans, députée de.

Parce que il y a une proposition de loi déposée par notre collègue et qui a je crois l'air de ça, c'est de faire tout le monde sauf le gouvernement après l'excellent travail fait par la commission, je peux vous dire, pour être franc, parce que notre rapporteur a été franche je vais être franc et je l'ai dit à Amélie Signac. On sait les difficultés du texte telle que c'était écrit ça été réécrit et bien écrit et de dire soyons prudent dans dans l'affaire et que nous allons faire une expérimentation. J'avoue que j'ai quelques doutes sur l'expérimentation. Comment généralisé après. Est-ce que vous croyez que Saint-Martin, va demander à bénéficier de l'expérimentation. Surtout après l'expérience de la Polynésie française. Qui dans la gestion du code civil a dû se retourner. Vers l'État pour dire, je n'ai pas les moyens de mes compétences et et que je vous demande d'assurer la gestion de la crise. Vous croyez que. Les territoires bénéficiant de l'autonomie, une autonomie que je comprends et que nous admettons en différenciation qui est à géométrie variable. Vous croyez qu'un territoire va demander à généraliser cette expérimentation comment généraliser une expérience qui n'a vocation à rester cantonné à Saint-Barthélemy. Alors peut-être une généralisation dans le temps de dire c'est pour 5 ans après, on verra si on pérennise mais c'est déjà une déformation de l'esprit de l'expérimentation. Elles-mêmes. Oui, je suis un peu sceptique. Comment voulez-vous et c'est une prudence qui a été prise par la commission de dire compte tenu des incertitudes, on sait pas si aujourd'hui dans une économie mono-sectorielles. Si demain il y aura des excédents et si la collectivité qui demande à, à remplir une fonction qui n'est pas la sienne. À savoir participer dans. Un domaine, je dirais presque du régalien puisque les la santé et compétence exclusive de l'État. On vous demande de cofinancer quelque part avec vous, sans pour autant partager la responsabilité. Bref, le pouvoir de proposition et et de financement. Commun hein comment comment faire ça. Alors on a circonscrit. À au seul périmètre de l'assurance maladie. L'assurance maladie, c'est tout juste, équilibré, hier c'était déséquilibré. Alors ça veut dire que, alors que la proposition première, c'était de dire, c'est toute la caisse à CBS, qui est une CPS qui qui qui porte ce nom-là mais qui est une CPS croupion, disons-le très clairement puisque c'est un comité de suivi adossé à Poitou-Charentes et qui me tient même pas de comptabilité analytique. Si ce n'est une comptabilité séparée à Sèvres viennent c'est bien ça. Non, on a là un problème de compréhension de la loi organique. Nous croyons comme ici et ce qu'a dit en lettres de feu et avec quelques. Ardeurs le président Larché lorsqu'il est venu récemment en déplacement aux Antilles Guyane en Guadeloupe et en Martinique. De dire qu'il faut faire dans la différenciation vous refusez Madame la Ministre. Et pourtant, ça s'appelle l'organisation territoriale et et. Professions de santé. J'avoue, je ne vous cacherai pas que j'ai été étonné de ne pas voir le ministre des Outre-mer, ici, c'est vous qui représenter c'est votre compétence mais pour en train de dire cela, nous nous partageons ici je le coup après ce qui est unanimement que c'est un bon texte, c'est un texte prudent. Qui a été pesées et soupesées qui est équilibré et je n'ignore pas pour être encore plus franc que oui peut-être que les élus là-bas ont d'autres projets. Peut-être qu'. Ils veulent aller plus loin. En extension en j'ai acheté et que sais-je encore. Ici c'est un texte élaboré par la commission qui est de nature à faire un consensus et un consensus, j'allais dire solide. Solide et on on expérimentation. C'est bien pour voir si c'est solide, si c'est pertinent si c'est efficace là vous récusez tout et je ne vois pas qu'est ce que vous proposez-moi pour avoir appelé. Un peu partout. Je crois savoir que vous attendez le siom. En disant, il est urgent.

que nous avions tout se crée. À l'époque, en 2009 c'est normalement le président de la République, il doit présider cette affaire là. Si ce n'est le président. La première ministre, hé bien on attend. Le siom pour dire on peut voter ça ici, mais attendons le siom pour voir ce qu'est le consensus. Peut-on trouver le serbe n'apportera rien de plus que ce texte là. Je crois que c'est le tacle plus prudent le plus équilibré. Et et qui est de nature à rassurer l'État. Et par ailleurs ce texte là à vocation peut-être a essaimé à imprégner a a imprimer. Et et ça peut inspirer d'autres territoires et non pas dans le sens que que vous croyez vous voyagez oublier totalement mon discours parce que j'attendais, celui de l'État ici au nom et pour le compte du groupe. Socialiste, écologiste et républicaine nous voterons ce texte parce que nous estimons qu'il est fondé qu'il est pertinent qu'il est bien écrit qu'il est prudent et qu'il répond aux besoins urgents. De Saint-Barthélemy. Merci. La parole est à la présidente, Éliane Assassi. Pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste. Madame la Ministre, mes chers collègues. On nous nous retrouverons donc aujourd'hui pour débattre d'un sujet important qui est celui de l'accès aux soins et à la santé, les années qui viennent de s'écouler ont été marqués par une forte pandémie où les limites de notre politique de santé ont été démontré notamment en outre-mer. Nous pensons que cette proposition de loi organique de notre collègue Micheline Jacques doit permettre une égalité dans l'accès aux soins. Alors ce qu'on observe les rapports sur le sujet. Plusieurs éléments reviennent, celui d'une offre de soins qui ne correspond pas toujours aux demandes des habitants de la collectivité de Saint-Barthélemy. En effet, ces derniers ne sont pas responsables du manque d'infrastructures sur le ring les élus territoriaux ont souvent témoigné auprès des pouvoirs publics leur insatisfaction. Face à l'offre de soins qui ne prend pas en compte toutes toutes les réalités de la collectivité. Les communes et leurs élus ont besoin d'un accompagnement fort pour mettre en place des politiques publiques afin d'assurer leur mission première de service public plusieurs difficultés se font ressentir les évacuations sanitaires ne sont pas systématiques, puisqu'il n'y a pas de possibilité d'évacuer les patients la nuit car les atterrissages atterrissage sont interdits et il faut entendre ce que vient de dire notre collègue Lurel à ce sujet. Les prises en charge des évacuations sont limités puisque si l'on souhaite que l'assurance maladie financée déplacements. Il faut que les lignes d'évacuation soient régulières. Cela pousse donc à des choix. Ce qui veut dire que l'accès aux soins n'est pas garanti pour toutes et pour tous. Aujourd'hui le seul hôpital disposant de plusieurs spécialités est donc situé en Guadeloupe. Ce dernier, qui a vécu hein ah a vécu un terrible incendie en. 17 et retrouvera sa réhabilitation Finnair. Uniquement 2024. L'hôpital de Saint Barthélémy est aussi confronté à un manque de personnel. Cela s'explique par la cherté de la vie sur l'île. Les prix des loyers augmentent, ce qui n'est pas le cas du pouvoir d'achat et cela se se ressent plus fortement dans les collectivités d'outre-mer oui Madame la Ministre les salaires des personnels soignants ne sont pas compatibles avec le prix des loyers en France métropolitaine comme en outre-mer le manque de moyens pour l'hôpital est flagrant. De ce fait, l'accès aux soins n'est pas garanti pour toutes et tous. Le personnel soignant souffrent. Ils souffrent de la non revalorisation de son statut de la non-, augmentation des salaires alors que ces femmes et ces hommes de comptent pas leurs heures. La fermeture des lits est toujours d'actualité. Les services sont toujours en tension la passivité constante du gouvernement doit cesser. Lorsque le Parlement demande des rapports pour écrire éclaircir des situations pour nourrir des travaux. Vous ne répondez pas lors de la crise sanitaire et du confinement, les habitants ont vécu les limites de cette passivité c'était dur, c'était très dur pour eux de ne pas pouvoir être évacués alors que leur santé en dépendait cette PPL eau est un 1er pas pour permettre une meilleure offre de soins et surtout une offre de soins qui puisse réponde aux réalités de l'île de Saint Barthélémy. L'État doit donner des moyens nécessaires pour l'accès aux soins et à la santé, la santé est une prérogative de l'État et ce dernier doit pouvoir prendre en compte les dysfonctionnements et les défaillances vécu au niveau des collectivités. Le présent texte est aussi un moyen de mettre en musique des méthodes horizontales de travail et d'échanges qui sont en demandée par les acteurs locaux plutôt que des approches toujours imposé par le haut sans concertation préalable, le caractère expérimental de ce texte en. Adopté en commission est effectivement prudent il permettra d'adapter les actions par rapport aux résultats de ce fait l'évaluation qui s'est qui se fera par l'état et la collectivité sera un moment, un moment fort et important et pour Saint-Barthélemy et pour l'État. Nous espérons surtout que les habitants de Saint-Barthélemy pourront bénéficier d'une offre de soins adaptés et que l'hôpital trouvera l'attractivité nécessaire pour assurer sa mission de service public, alors nous serons attentifs à la mi-et attentive à la mise en place de cette proposition. Nous resterons les fervents défenseurs de l'égalité et cela est aussi va là pour l'accès aux soins pour toutes ces raisons, le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste votera pour cette proposition de loi organique. Merci. La parole est à monsieur Philippe Folliot. Pour le groupe Union centriste. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission. Madame, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Chers collègues Micheline hein. Jacques. C'est Christophe Colomb qui découvrit. L'île de Saint-Barthélemy et et du reste le nom est lié au frère de Christophe Colomb Bartolomeo. Et 3 dates ont marqué l'histoire de cette vie tout d'abord c'est 1784 quand Louis XVI décide. De la donner à à la Suède. Et près d'un siècle. Un peu plus de siècles plus tard. 1878. Elle redevient française suite à. à. Terrible cyclone qui avait déjà à l'époque hein dévasté l'île une 3ème date importante dans l'histoire de Saint-Barthélemy ces 2007 2007 quand. Ce qui était une commune, du département de la Guadeloupe devient une collectivité et et à partir de là, peut commencer à prendre mieux en main son destin avec des éléments qui caractérisent. Saint-Barthélemy c'est tout d'abord. J'allais dire la la la la mono-. Activité pour ainsi dire, qu'est le tourisme et qui ne manque pas d'avoir des conséquences y compris par rapport au sujet dont nous parlons aujourd'hui puisque la population qui est de 9000 habitants. Va jusqu'à 15.000 habitants avec les saisonniers l'été plus les les touristes et donc avec la nécessité d'avoir des éléments de sanitaires et qui puissent être adaptées par rapport à cette situation. Spécifique. Bien entendu ce texte. Que vous portez chers collègues dans le droit fil de votre prédécesseur, Michel Madrasse que je que je salue et est un texte qui est un texte tout à fait à propos et ce à plusieurs titres. Tout d'abord par rapport. Au caractère expérimental de celui-ci et la volonté qui le. Donc de la collectivité d'assumer. Aux côtés de l'État un certains nombres de conséquences et des conséquences qui sont particulièrement importantes pour la population puisque ça a trait à la santé et on peut dire ce que l'on veut mais sans le socle j'allais dire d'un service de santé efficace et adaptée toute perspective de développement, j'allais dire économique et sociales d'un territoire est complètement annihilé et donc en ce sens cette un élément important que la collectivité accepte et souhaite et veuille prendre ses responsabilités, aux côtés de l'État en la matière. Le 2ème point qui me paraît paraît essentiel c'est c'est de dire que ce texte est un texte qui est éminemment bien construit, cela a été dit. Madame, monsieur, le le le rapporteur longs l'souligné. Avec une durée limitée dans le temps et des rapports d'étape et des capacités qui vont faire que ceci permettra de répondre de la meilleure façon qui soit aux besoins exprimés par la collectivité donc et et ses habitants. Pour autant. L'offre de santé. Ne peut pas reposer que sur Saint-Barthélemy. À proprement parler et que bien entendu. Les Liens. T'obliger à ce stade de parler de géographie puisque distante de 25 kilomètres donc de Saint Martin de 240 à quelques kilomètres de la Guadeloupe si vous me permettez l'expression de cette tyrannie des distances fait que on ne doit tenir compte de ce cadre et de 7 éléments de spécificité. Par rapport à l'offre qui. De soins va être apportée.

donc de la Guadeloupe hein. Les malades qui en ont le besoin. Je voudrais revenir sur un point, un élément qui me paraît important c'est cette notion d'évacuation sanitaire à plusieurs collègues ah non parler et et donc dans ce cadre-là,

Que. Les questions relatives à une approche spécifique pour nos départements et nos collectivités d'outre- mer dans ce cadre-là, revêt sa plus particulières singularités. Je m'explique.

Mais l'approche qui serait peut être judicieux, c'est d'avoir ce n'est pas d'avoir une une approche si vous voulez uniquement basé sur un seul aspect des choses. Ce qui ne pourrait être intéressant d'expérimenter en liaison avec l'État, les différentes administrations, la collectivité de Saint-Barthélemy, mais aussi la collectivité de Saint-Martin, c'est d'avoir un hélicoptère qui soit basé sur place mais qui soit totalement polyvalent, c'est-à-dire qu'ils puissent se servir pour les évacuations sanitaires qui puisse servir pour la douane Douane qui puisse servir pour la gendarmerie qui puisse servir pour la protection civile, c'est-à-dire donc un outil qui pourrait être totalement polyvalent et adapté et qui pourrait amener ce service localement parce qu'on le sait très bien que. Dépossédé. Donc que la Guadeloupe de son hélicoptère d'évacuation sanitaire pour aller à Saint Barthélémy ça ne manque pas de poser des difficultés parce qu'ensuite la Guadeloupe se trouvent dépourvus de de moyens et donc je crois que. Cette singularité et cette nécessité de d'essayer de faire de telle sorte que toutes les administrations puissent travailler ensemble pour apporter un liaison avec les collectivités. Une solution qui soit une solution originale et spécifique me semblerait très modestement être une piste tout à fait intéressante qui pourrait permettre de répondre à ce besoin mais à d'autres besoins aussi la lutte contre le narcotrafic. Les les éléments relatifs donc. À la sécurité à la sécurité publique. Et, et en cas d'urgence aussi. Bien sûr, les évacuations sanitaires. en conclusion je je je voudrais dire au au nom du groupe Union centriste que bien entendu nous allons voter ce texte parce que, comme nous l'avons dit et comme cela a été répété par les uns et par les autres, il est bien construit, bien équilibré et puis ensuite il va répondre à un besoin qui est le besoin des populations de Saint-Barthélémy mais qui est aussi exemplaire par rapport à cette capacité que vous nous mais permettez de mettre en oeuvre. Ma chère collègue d'expérimentation et nous sommes très attachés au sein de notre groupe à cet aspect des choses parce que. Il est clair que dans ce domaine comme dans bien des domaines une approche uniforme national est totalement inadaptée et plus encore, donc par rapport à nos outre-mer et donc c'est pour cela qu'avec. Ambition et volonté mais aussi surtout conviction nous voterons favorablement pour ce texte. Je vous remercie. Madame la présidente, madame la ministre. Madame messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, ma conviction est que les statuts uniformes ont vécu. Et que chaque collectivité d'outre-mer doit pouvoir désormais si elle le souhaite évoluer vers un statut différencié en quelque sorte un statut sur mesure. Ces quelques mots du discours du président Jacques Chirac prononcé le 11 mars 2000 à Madiana en Martinique font encore écho aujourd'hui. Et j'ai mon arrêté là finalement parce que j'avais comme Victorin Lurel préparer une allocution. et je dois bien le dire, que le gouvernement m'a beaucoup aidé, puisque le gouvernement Madame le Ministre vous venez nous donner raison finalement quand on entend la position du gouvernement, c'est pas une position personnelle bien évidemment sur le texte vous donner raison aux travaux du Sénat menée actuellement par le président Larché sur plus de décentralisation, plus de déconcentration et on voit à quel point également, on a affaire à une espèce de rigidité de l'État central sur le sujet. Je vais quand même revenir sur sur le texte. C'est vrai que initialement pour avoir participé à à une audition et la dernière, en l'occurrence, une des plus révélatrice peut être avec nos deux rapporteurs. On se rend compte quand même que l'espèce de démembrement d'une compétence entre l'État, une collectivité est compliqué. Et on peut le concevoir intellectuellement et ça a été assez révélateur entre la direction de la sécurité sociale à la direction générale de l'organisation des soins. Et on peut effectivement identifié déjà les points de blocage et les points de difficultés qui peuvent être soulevés à cet égard. Mais je sais j'aimerais saluer le le travail de deux rapporteurs qui ont pu aller jusqu'au bout de cette démarche et trouver un équilibre et Victorin Lurel a rappelé avec l'auteur de de la proposition, dans le cadre des auditions et cet équilibre, finalement c'est l'expérimentation. Alors ce qui est quand même étonnant, c'est que ce qui est possible dans certains territoires ne l'est pas dans d'autres à Saint-Pierre-et-Miquelon et Miquelon par exemple nous n'avons pas la compétence transport maritime en fret et nous venons avec le gouvernement de signer une expérimentation. Pour justement permettre à la collectivité. Sur un ton donnée par convention de tester la compétence son fret et je ne comprends pas justement c'est pour ça que je dis que le gouvernement nous rend bien service aujourd'hui sur ce texte en particulier. Pourquoi ce qui est valable dans une collectivité de l'article 74 ne l'est pas dans une autre collectivité de l'article 74. Avec quelque part finalement quelque chose de bon sens une proposition des rapporteurs et de l'auteur visant à dire que finalement sur ce secteur de la santé, la sécurité sociale et on peut comprendre les difficultés que ça peut poser, on partage de compétences, une expérimentation a le mérite effectivement avec les réserves évoquées par Victorin Lurel sur la démultiplication ou du moins l'élargissement par la suite de l'expérimentation mais à tout le moins, j'aimerais quand même rendre hommage à à Micheline Jacques qui a le mérite de vouloir faire bouger les choses et je pense que cette proposition effectivement a le mérite de faire bouger les lignes. À charge évidemment aux législateurs et aux acteurs locaux de prendre leurs responsabilités dans les années qui viennent pour voir de quelle manière, cette expérimentation et je souhaite malgré tout. Mes chers collègues, que le Sénat puisse rallier à cette proposition de loi organique mais également la position de la commission il ne rapporteur de voter ce texte qui de mon point de vue est strictement l'expression de ce que vous demandez tout c'est ce que nous demandons tous dans le territoire une approche de l'État différencier dont chacun de nos territoires qui tiennent compte de nos réalités qu'elle soit en outre-mer ou dans l'Hexagone dans les zones de montagne ou dans des zones de ruralité, de manière générale, cette expression finalement et cette proposition de Micheline Jacques elles ouvrent la voie finalement aux travaux que nous menons au Sénat et qui aboutiront comme ils ont abouti en 2020 à des propositions concrètes. Le président du Sénat la rappeler et Victorin Lurel a dit lors de son déplacement en Guadeloupe et en Martinique, avec plus de différenciation plus de décentralisation, mais un État plus fort sur les territoires et là on se rend compte malgré tout que cette position du gouvernement, elle vient fragiliser malgré tout cette ambition qui est une ambition je trouve plutôt saine et une une ambition légitime, je pense que comptez collectivités ont sont poussés à ce niveau de, de monde c'est qu'on constate finalement que les choses ne fonctionnent pas et comme je le disais à Victorin Lurel cet hélicoptère effectivement dans une quinzaine d'années, on en parlera sans doute encore parce que ce n'est pas si simple. Ça n'est pas si simple que ça a réglé ça se saurait. Et si c'était le cas Madame le Ministre je pense que les élus ne se serait pas posé la question et je pense que Micheline n'aurait pas initié ce projet de loi organique. Tout simplement parce que si la réponse exister. Je pense qu'on n'est pas là pour légiférer à tort et à travers ni se faire plaisir, on se tapant sur la poitrine, c'est qu'on est là pour régler des problèmes de nos concitoyens et qui a une vraie difficulté sur ce territoire, en particulier une demande qui est récurrente et qui est ancienne et franchement le groupe RDSE dans son ensemble se tiendra bien évidemment, ce projet de loi organique modifier modifier avec l'assentiment des rapporteurs qui ont trouvé, me semble-t-il un point d'équilibre et j'aimerais évidemment contre la la position que le Sénat adoptera et la navette qui va avoir lieu on, espérons que le texte soit repris à l'Assemblée nous puissions également trouver un équilibre. Même si l'avis du gouvernement doit évoluer. Moi j'aurais aimé également connaître l'avis du ministre délégué aux Outre-mer qui est de mon point de vue est fragilisée par cette position parce qu'il porte. Évidemment, l'ambition du président de la République qui, le 7 septembre a dit qu'il était pour une approche différenciée en outre-mer, or aujourd'hui on voit qu'on est sur une approche jacobine et je vous invite évidemment à voter ce projet de loi. La parole est à Mathieu Darnaud pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente. Madame la ministre sur le président, madame le rapporteur Monsieur le le rapporteur. Il est toujours savoureux avec ce gouvernement. De goûter. Aux ascenseur émotionnel qu'il nous permet de vivre. J'utilise le mot à dessein. Toutes les expressions qui se sont succédé comme les travaux préparatoires et nous avons eu l'occasion d'en parler avec l'auteur de ce texte Micheline Jacques que je tiens à saluer. Nous laissait à penser que l'équilibre revendiqué de de ce texte que son fondé amènerait le gouvernement a donné un avis favorable face à à cet élan d'espérance. Cet elle en a trouvé malheureusement. Que d'égal la déception qui est trop souvent à l'arrivée, alors même que tous nous laisser à penser que, comme je viens de le dire ce texte pouvait recueillir l'assentiment du gouvernement. Je le dis parce que. Et celles et ceux qui, à cette tribune viennent de s'exprimer ont démontré à la fois le caractère équilibré. L'Intelligence du recours à l'expérimentation et comme l'a souligné le le rapporteur Alain Milon. La nécessité. De donner. Des gages et surtout de permettre une continuité des soins, de permettre. À l'évidence de répondre à la problématique des évacuations sanitaires et de bien d'autres problématiques. Au fond, Madame la Ministre j'ai parfois le sentiment de revivre ce que nous avons vécu à l'occasion de l'examen du texte 3DS. Certains y ont fait référence avec un gouvernement avec un État qui est toujours très allant à demander aux collectivités de participer aux investissements. C'est ce que nous avons fait confiant dans la parole de l'État et de l'autre côté, un État qui peine à vouloir partager les compétences lorsqu'il s'est agi de faire des présidents de région des coprésidents d'ARS. En réalité c'est faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais et c'est assez triste finalement parce que au delà de ce texte vous renvoyer comme beaucoup de collègues Blondy un bien mauvais signal. Je vais revenir. Revenant à ce texte. C'est un texte qui je pense avait le mérite et je veux à mon tour rendre hommage, comme je l'ai fait à l'instant à l'auteur Micheline Jacques précédemment à notre collègue. Michel Magras qui a été un des aspirateurs de ce texte qui a inspiré aussi beaucoup de réflexions, s'agissant de l'outre-mer et puis. À la collectivité. Je pense notamment la première vice-présidente Hélène dernier qui a participé à ces travaux parce que au final et la seule raison qui vaille dans ce texte, c'est bien de répondre, comme je l'ai dit aux aspirations très concrète des habitantes et des habitants. De Saint-Barthélemy et de permettre à la collectivité, de participer et quand j'entends votre propos Madame la Ministre j'ai l'impression que vous parlez d'une automatisation. On a le sentiment finalement que. Saint-Barthélemy. Va larguer les amarres et veut gérer à elle seule cette compétence de tout cela il n'en est rien. Nous avons simplement face à nous une collectivité qui dit vouloir partager l'effort et être au rendez vous des attentes et surtout surtout s'inscrire et je vais faire bien les propos qui ont été tenus par notre collègue. Victorin ou par notre collègue Stéphane Artano qui s'inscrivent dans un principe de différenciation. Je reviens sur le texte 3DS. C'est bien beau, que l'État veuille invité à plus de différenciation mais quand tu l'occasion vous est donnée. Madame la Ministre vous tournez le dos à cette différenciation encore une fois, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que l'État fait et tout et c'est là bien quelque chose de bien regrettable. Au fond. Et on le sait. La tentation c'est de renvoyer ça a été dit aux travaux. Du. Mais qu'attendre finalement de ces travaux si alors que l'occasion vous est donné finalement de prendre la balle au bond et de saisir l'esprit d'initiative portée par le texte de notre collègue Micheline Jacques et par la collectivité. Qu'attendre, si ce n'est finalement désespoir qui seront encore une fois 20 et je crois qu'il y a là un vrai sujet en tout cas notre groupe. S'interroge sur la volonté réelle, nous l'avons déjà soulevée à l'occasion des textes précédents. Nous avons d'ailleurs je le dis pour en avoir été le rapporteur avec Françoise Gatel travailler sur l'expérimentation pour ouvrir le Champ des possibles et pour faire en sorte que des initiatives comme celle-ci puisse être possible Malheureusement notre espoir va encore être aujourd'hui déçu. Alors bien évidemment, nous voterons. Avec conviction ce texte considérant. Finalement, il permet de d'ouvrir et de tracer un sillon. Nous espérons que demain le gouvernement et je regrette aussi. Que le ministre des Outre-mer n'est pas de livrer son son avis sur sur ce sujet-là. Je regrette malheureusement. Que le rapport encore une fois votée dans le cadre du texte 3DS n'ait pas été rendue. Alors même si j'ai entendu que tardivement. Nous aurons les réponses à nos interrogations. Mais je crois qu'il y a madame la Ministre urgence aujourd'hui à agir urgence à répondre aux aspirations des territoires et à l'aspiration du territoire de Saint-Barthélemy qui depuis longtemps fait preuve de cet esprit d'initiative qui ne doit pas rester sans réponse de votre part. Comme je l'ai dit nous voterons avec conviction ce texte un texte équilibré, un texte qui permet de répondre de façon pragmatique aux interrogations des habitants qui permet aussi d'ouvrir la réflexion de façon là aussi très pragmatique sur la question de la différenciation encore une fois à rendre hommage à Michel Magras ancien président de la délégation aux outre-mer qui a ouvert la voie sur ce sujet avec encore une fois des. Des propositions inspirantes espérons que notre assemblée qui a été souvent précurseur sur ces sujets le soit encore. J'ai noté dans la tonalité des intervenants qui se sont succédé une volonté de soutenir ce texte, espérons. Madame la Ministre. Que ces positions vous invite à à faire évoluer dans le temps et le plus rapidement possible votre avis en tout cas vous l'aurez compris, nous serons bien évidemment en soutien et en approbation du texte de notre collègue Micheline Jacques je vous remercie. Merci la parole est. Non à Denis va te blé pour le groupe les indépendants.

Madame la présidente, madame la Ministre. Monsieur le Président. La commission des lois. Madame la rapporteure. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Les problèmes la digue judiciaire sont médical et d'accès aux soins ne concerne pas uniquement le rue territoire métropolitain. En effet en matière d'offre de soins. Nos compatriotes de Saint-Barthélemy sont confrontées à d'importantes difficultés. Aux formes très variées en raison de l'isolement. Et de la scolarité de leur territoire. De nombreux exemples-ils cette situation. Ainsi, lorsque la prise en charge de cas graves nécessitent des des évacuations sanitaires vers Saint-Martin ou la Guadeloupe. Celle-ci ne peut s'effectuer qu'en journée en raison de l'absence d'éclairage des pistes. Et on déplore en outre la présence d'un seul hélicoptère. Pour la zone et l'de procéder à des rapatriements par bateau, compte tenu des distances. Concernant le personnel hospitalier, il est fait appel à des contractuels. Les services de soins ne parvenant pas à fidéliser les praticiens du fait du prix élevé des logements des contraintes d'exercice. Or, il est indispensable que nos compatriotes Saint-Barthélemy puissent accéder à une offre de soins de qualité et adaptés aux particuliers du territoire. C'est pourquoi je me réjouis de l'initiative de notre collègue Micheline Jacques qui par cette pression de loi tente de remédier à ces difficultés. L'article 1, confie ainsi au conseil territorial un pouvoir de propositions, dans les domaines de la sécurité sociale et du financement des espérances de santé relevant de la compétence de l'État. L'article de des la procédure de participation de la collecter à des compétences. L'article 3 prévoit la définition d'un budget annuel de dépenses de fonctionnement et de financement des surcoûts d'épuisement médicaux et Mikko sociaux ainsi que les évacuations sanitaires. Je tiens à saluer l'esprit consensuel qui a prévalu lors de l'examen en commission. Les modifications qui ont été apportées vont dans le bon sens. D'une part je partage la position de la Commission lorsqu'elle a considéré qu'il serait pertinent que ce dispositif soit expérimenté pendant 5 ans avant de l'envisager en pérennisation. D'autre part la prochaine de loi prévoyait d'imposer au conseil territorial, la définition d'un objectif annuel de dépenses

qui faisait poser une contrainte nouvelle sur une collectivité qui ne possède ni les moyens ni les compétences pour procéder à une telle évaluation. Avant de conclure, je souhaite saluer le travail accompli par la rapporteure Madame Boyer et son implication sur le sujet d'importance pour la côté de Saint-Martin et le compatriote ultra moins Madame la Ministre, chers collègues, cette proposition de loi présentent un intérêt indéniable, même si elle ne peut résoudre. À elle seule tous les problèmes d'accès aux soins. Elle constitue un 1er pas salutaire vers une meilleure prise en considération par l'état. Des spécificités et des nécessaires adaptations de l'offre de soins à ça marque Barthélémy. Ainsi le groupe les indépendants votera à l'unité ce texte qui répond au besoin urgent. D'une véritable différenciation territoriale.

Madame la présidente. Madame la ministre. Madame l'auteur la rapporteure mes collègues. Le nouveau séjour de pencher sur un problème qui est récurrent d'organisation territoriale à laquelle le Sénat est toujours particulièrement attentifs. La problématique qui a été mise en avant. Par l'auteur et qui a été étayée par les excellents travaux des rapporteurs et celle du manque de moyens pour les collectivités territoriales pour agir sur des compétences étatiques en l'occurrence de confier à la collectivité de Saint-Barthélemy, à pouvoir de propositions dans le domaine de la sécurité sociale, du financement des établissements de santé, qui relèvent de la compétence de l'État. L'offre de soins local de Saint-Barthélemy et très restreinte s'appuie fortement sur la Guadeloupe et c'est Martin la situation certes n'est pas nouvelle mais la pandémie a permis de mettre en avant le rôle et la réactivité qui ont pu développer les collectivités locales partout dans le domaine de la santé. À Saint Barthélémy la situation locale ne permet pas la prise en charge de cas graves et complexes et conduit à de nombreuses évacuations sanitaires vers Martin en particulier nos conditions a rappelé l'aspect indispensable de ces évacuations sanitaires mais aussi les difficultés qu'elle présente. Matériel, bien sûr avec les conditions on en a parlé, mes collègues, on en parlait de l'aéroport de Saint-Martin. Les contraintes aussi de l'utilisation de l'hélicoptère basé en Guadeloupe mais aussi financière puisque ces évacuations sont réalisées souvent par des sociétés privées. À défaut de pouvoir être faite via des lignes régulières. Et pour permettre un financement par l'assurance maladie coup eau quand même 600.000 euros par an pour à peu près de 100 rotations. 2 autres sujets ont été mis en avant par l'auteur et par la rapporteure, à savoir l'absence à ce jour de reconstruction de l'hôpital. Cinq ans après le passage de l'ouragan. Ce qui ne permet pas d'améliorer d'ailleurs l'attractivité des conditions d'exercice des soignants qui déjà entravé. Ma collègue. Rappeler aussi par le coût de la vie sur l'île mais aussi les problématiques à huit par la gouvernance de l'ARS qui l'ce peu de place à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy. Ces difficultés ne sont pas nouvelles on nous avions déjà eu par le passé des propositions de modifications pour un régime prend ah Barthélémy. La version initiale de cette proposition écartée la possible ouverture de la participation à l'exercice de la compétence de l'État en matière de santé car requérant des compétences techniques dans Saint Barthélémy et dépourvu et qui représente un coût exorbitant. L'auteur que je salue. Avait souligné le besoin impérieux que la santé reste un domaine qui doit être mis à l'abri des aléas politiques Le besoin d'une plus grande participation de la collectivité avait donné lieu à la rédaction de trois amendements permettant une plus grande autonomisation du système Assia Barthélémy. Toutefois, après les discussions dans le dos d'nos 2 commissions, plusieurs points ont été soulevées. Les constats de la direction de la sécurité sociale en met en avant une mauvaise appréciation de la situation financière dès lors que la situation de la caisse ne reflète pas celle de régime de Sécurité sociale autonome et mais une part substantielle des financements dont bénéficie le système de santé de Lille. Établissement que la solidarité nationale s'exerce bien aussi au profit de l'île. Les deux rapporteurs ont pu assister à juste titre sur ce principe de solidarité au coeur de notre système de sécurité sociale. Principe fondamental qui qui inscrit dans le texte de la commission aussi au lieu d'une réforme statutaire initialement proposé la commission s'est dirigé vers une expérimentation. De l'exercice de ce pouvoir de proposition par la collectivité. La durée de cette expérimentation de cinq ans. Laisse le temps d'une mise en oeuvre et d'ajustements nécessaires afin d'évaluation et un rapport devrait être rendu dans les 6 mois suivant la fin de l'expérimentation. Au passage, monsieur Mes collègues à Alain et Valérie Boyer, vous le rappeler. Parmi les rares rapport que demande l'autre assemblée au gouvernement ne demande pas énormément. On pense que le gouvernement pour pourri Ido des suites. Ce qui nous permettrait des fois d'éclairer nos débats alors j'ai bien compris qu'on l'aura au mois de juin après la loi, bon pourquoi pas, en tout cas on l'aura peut-être un jour l'inertie de la prise de décrets d'ailleurs s'y ajoutent hein parce que là aussi ça ne va pas très, très vite. Et donc ça ne contribue pas dans plus améliorer les choses. Au au sujet d'ailleurs d'une nécessaire réflexion d'une organisation territoriale plus décentralisée. Et des travaux de notre assemblée sur ce sujet des décrets plus rapides et des rapports plus rapide permettrait à d'autres travaux des fois de prendre plus de sens. L'encadrement de ce nouveau pouvoir permet de rester dans une réflexion au coeur du donc de soi à Saint-Martin en Guadeloupe. C'est pour ça que sera soumis à l'ARS compétente tout projet d'acc de conseil territorial afin d'assurer la compatibilité du tête propositions avec l'organisation existante et régionalisé. les travaux en restera le Champ des compétences susceptibles de faire l'objet de propositions du conseil territorial à la salle assurance maladie au financement des établissements et des services de santé en vue de garantir la continuité des soins et l'adaptation aux particularités besoins spécifiques de l'Ordre de soins liés à l'insularité aller loin de éloignement cette l'océan quand il était des soins et la question fondamentale sur laquelle nos concitoyens et nos élus locaux nous interroge toujours et à juste titre, notre groupe attaché à l'engagement local à l'expertise des élus en ce sens à l'expérimentation votera donc pour cette proposition de loi, tout en rappelant que sans un engagement fort et rapide de l'État. Toute démarche locale sera vaine. Merci la parole est maintenant à Nadège avait pour le groupe RDPI. Madame la présidente, madame la ministre madame la rapporteure. Monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues. Perte mettez-moi tout d'abord de remercier notre collègue Micheline Jacques et son groupe d'avoir demandé l'inscription de cette proposition de loi organique à l'ordre du jour de notre assemblée. L'examen de ce texte permet de mettre en lumière certains des défis auxquels fait face la collectivité de Saint-Barthélemy. Des défis qui sont accentués par son isolement géographique et sa faible population comme dans les autres territoires ultramarins. Les questions de santé sont au coeur des préoccupations des habitants et des élus. Les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune ont tous rappeler les difficultés sont nombreuses. Pénurie de soignants lié à un manque d'attractivité de Lille, difficultés d'accès aux médecins spécialistes, obligation de procéder à de nombreuses évacuations sanitaires parfois dans des conditions difficiles. Impossible de constituer un stock de 100 impossible pour l'hôpital de recruter un pharmacien d'officine infrastructures hospitalières partiellement détruite par l'ouragan Irma. Elles sont donc nombreuses les difficultés. Afin de remédier à ces difficultés, notre collègue de Saint Barthélémy propose de recourir à l'article 74 de la Constitution aux termes duquel la loi organique peut déterminer les conditions dans lesquelles une collectivité d'outre-mer doté de l'autonomie peut participer sous le contrôle de l'État à l'exercice des compétences qu'il conserve. Et cela dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques. Ce dispositif permet d'ores et déjà Saint-Barthélemy, de participer, sous le contrôle de l'État à l'exercice des compétences qui relève de l'État en matière pénale, il est proposé d'étendre cette possibilité en matière de sécurité sociale et de financement des établissements de santé. Il y a un peu plus de 7 ans, une initiative similaire avait été prise par le Parlement. En effet, l'article 6 de la loi organique du 17 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy prévoyait la possibilité pour l'État d'habilité par décret en Conseil d'État et pour une durée maximale de trois ans, le conseil territorial de Saint-Barthélemy a adopté d'exact dans le domaine de la sécurité sociale. Cet article avait été censurée par le Conseil constitutionnel en raison d'une incompétence négative. Contrairement au dispositif adopté en 2015 celui prévu par la présente, proposition de loi apparaît conforme à la Constitution. Dans la mesure où la fixation des règles entourant la participation de la collectivité aux compétences de l'État n'est pas renvoyé au pourvoir réglementaire. La solidité juridique du dispositif proposé est d'autant plus forte que la commission des lois restreint le Champ des compétences pouvant faire l'objet des propositions du conseil territorial à la seule assurance maladie. Les améliorations apportées au dispositif initial sont d'autant plus opportune, que le gouvernement a fait de la santé sur l'île une priorité. Grâce à une aide importante de l'État, les évacuations sanitaires ont pu être maintenus lors d'un récent déplacement à Saint-Barthélemy. Le ministre des Outre-mer Jean-François Carenco, Carenco, a demandé au préfet délégué de s'investir fortement sur le sujet afin d'aboutir rapidement à une solution. La collectivité et la préfecture ont ainsi engagé des travaux communs. Parmi les pistes explorées figurent l'investissement dans un avion ou un hélicoptère. Pour ce qui concerne l'hôpital Saint Barthélémy à une enveloppe a obtenu une enveloppe pardon de 14, 7 millions d'euros dans le cadre du Ségur de la santé. Cette enveloppe va permettre la réalisation d'aménagements dont l'agrandissement du service des urgences. La récente arrivée de nouveaux médecins sur l'île est également bienvenue. Par ailleurs, il semble que des obstacles réglementaires pourraient être levées par un décret en Conseil d'État ce Beda ce débat nous donne l'occasion d'inviter le gouvernement a publié ce décret dans dans les meilleurs délais. De même que le rapport prévu par la loi dite 3DS sur la situation sanitaire de Saint Barthélémy. Enfin, nous devrons veiller à écarter tout risque de remise en cause du principe de solidarité nationale sur lequel repose la sécurité sociale. Un transfert de compétences sous le contrôle de l'État et sous la forme d'une expérimentation.

Oui merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs. Tout d'abord pour rappeler qu'il s'agit bien ici de la position du gouvernement et donc aussi du ministre des Outre-mer, madame Assassi a dit que c'était un sujet important, je suis d'accord, c'est un sujet important et nous donnions aucune difficulté aucune difficulté et le constat, nous le partageons la différence entre ce que vous proposez est l'analyse que fait le gouvernement c'est que nous ne souhaitons pas nous ne souhaitons pas faire prendre le risque hein. À à Saint Barthélémy à travers cette modification concernant la CPS de ce que fait notre pacte républicain, sur la solidarité que représente la sécurité sociale, c'est le risque. Dont nous pensons qu'il peut être pris par cette modification à travers cette loi organique. Nous pensons que c'est pas à travers cette réponse institutionnelle qu'on peut apporter des réponses structurelles. D'abord la loi 3DS permet aux collectivités d'intervenir, notamment dans le cadre du logement par exemple. Et que le président de la République nous a demandé de travailler sur le pacte territorial que nous proposons à toutes les collectivités et donc aussi. À la collectivité de Saint-Barthélemy ce pacte territorial il repose bien sur la volonté et c'est la ministre en charge de l'organisation territoriale qui vous le dit de travailler avec les territoires à partir des territoires et ce pacte territorial ne sera proposé à toutes les collectivités d'ici la fin de l'année. Enfin pour redire que le décret dont tout le monde parle et à parler. Il. Paraîtra fin mars le décret qui donne les dérogations aux ARS que je le redis, monsieur le sénateur. Il est parti je crois. Que le rapport paraîtra bien en avril et et qu'enfin. Tout ce qui. À faire au problème d'atterrissage. À travers l'éclairage de la piste de la nuit et de l'hélicoptère a été comme ça a été dit. Le préfet, le préfet a été mandaté par le ministre-Carenco pour que ces problématiques soient prises rapidement et très au sérieux car nous savons bien que c'est un, un des enjeux majeurs donc. Vous redire que tout ce que vous avez évoquées, nous partageons nous ne nions pas les difficultés. Simplement nous n'avons pas du tout la même lecture. De la modification que vous souhaitez apporter dans le cadre ça qui est la déclinaison de la sécurité sociale, nous souhaitons conserver ce que la sécurité sociale apporte de beau à nos concitoyens, c'est-à-dire la solidarité. C'est sur l'article 1, une demande de parole de Alain marque.

Qui s'abstient il est adopté l'article 2 était supprimé l'article 3, été supprime supprimer et je vais maintenant mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi et à toutes les demandes d'explications de vote. Madame Conconne. Madame la présidente madame la mini-, chers collègues. Bien sûr que mon soutien total ira à ma collègue Micheline Jacques pour son initiative que je salue vraiment de tout mon coeur. Il y a un Martiniquais célèbres chez nous qui a déclaré que les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises sont les Martiniquais. J'ai envie d'appliquer cette Maxime à Saint-Barth et ma collègue en fait la démonstration. On peut être français mais on peut être également extrêmement imprégné des réalités de son pays et souhaité le mieux pour ses compatriotes, elle en fait la démonstration. Il faut savoir Madame la Ministre qu'il n'y a aucune incompatibilité entre égalité des doigts et doit à l'initiative et ça le gouvernement l'univers tout entier doit s'habituer à cette révolution culturelle qui consiste à dire que les peuples. En particulier les pubs de la dite outre-mer ont le droit d'avoir en regard le plus précis, le plus pertinent le plus légitime possible sur leur réalité tout en demeurant dans l'espace français et européen. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup gêné dans ce que j'ai pu entendre venant du gouvernement. Cette énumération presque impertinente de ce qui a pu être réalisé dans nos territoires pendant la crise Covid. C'était impertinent. Déplacé et au sujet. Oui madame. Il y a eu une crise Covid et nos territoires comme tous les territoires français ont bénéficié de la solidarité nationale sinon. À quoi bon avoir le pavillon français qui battrait sur nos territoires. Madame, est-ce qu'on va reprocher un auvergnat breton un normand ou à marseillais d'avoir reçu ce qu'on a regroupé sous le chapiteau du quoi qu'il en coûte. Non ah nous il faut toujours le rappeler, il faut toujours le dire comme si régulièrement il faudrait ici presque. Excusez-. Habillée, en robe de bure d'avoir bénéficié d'une solidarité pertinente et légitime. Évitons désormais ce genre de travers ça fait de nous. De nous, collectivement, je parle une forme de résurgence de ce que ces rappelait le vieil homme

d'un pays comme la France qui serait un pays progressiste ouvert à la différence, ouvert aux particularités ouvert à la spécificité et qui ne. Kroichvili pas sur lui même, dans une forme de nombrilisme qui peut être mortelle.

Au terme de l'examen de ce de ce texte. Je veux redire ma gratitude au rapporteur Valérie Boyer à la Milan mes remerciements vont également à tous les orateurs, des groupes qui ont apporté leur soutien. Ma proposition de loi organique et de l'intérêt qu'ils ont montré pour Saint-Barthélemy Madame la Ministre je regrette en revanche que nous n'ayons pas pu réfléchir ensemble. Pour preuve, la transmission la semaine dernière comme je l'ai souligné en discussion générale des chiffres de la sécurité sociale. Cela fait plus de 10 ans pourtant que nous nous en prévalant et que le ministère de la Santé parfaitement. Informé. Comment ne pas avoir le sentiment d'une défiance Saint-Barthélemy a toujours entretenu une relation harmonieuse avec l'État. Cette proposition de loi n'est pas contre l'État, j'attends la publication du rapport prévu par la loi 3DS je remercie en outre votre cabinet qui m'a reçu ce matin pour sa grande disponibilité, là encore, je ne peux que regretter que c'est cet échange particulièrement poussé et riche n'ait pas eu lieu plus tôt. Depuis le 14 octobre. Je veux rappeler ici qu'il n'y a pas de volonté d'autonomisation exprimé à à travers ce texte seulement une organisation en écho au statut. J'aimerais aussi souligner que les 4 millions sept du Ségur qui devait permettre la reconstruction de l'hôpital détruit en partie par l'ouragan Irma n'a toujours pas été reconstruit après 6 ans. Au-delà des aspects de compétences. Il reste que la médecine coûte plus cher à Saint-Barthélemy et que pour garantir un accès continu à universel son financement doit être adapté en ma qualité de co-, rapporteur de l'allégation outre-mer sur la différenciation je relève que ce débat prouve, s'il en était besoin au département d'outre-mer l'attachement de l'État, la solidarité nationale, par le biais de la sécurité sociale. Je souhaite que le Sénat adopte ce texte car il pose également la question de la, de de la manière dont l'État conçoit la mise en oeuvre des politiques publiques outre-mer en lien avec les collectivités. Je vous remercie. merci madame la présidente, madame la ministre. Chers collègues, j'ai une pensée toute particulière. À l'ancien président sénateur. De Saint-Barthélemy, monsieur Michel Magras qui avait initié aussi ce que nous allons adopter. Aujourd'hui. Merci à notre collègue de savoir d'avoir remis

et je crois que je parle au nom de tous mes collègues. Des Outre-mer c'est simplement le droit à la différenciation. Soir l'état nous fait confiance, soit l'État nous fait plus. Confiance après le le sujet de la réforme de la de ou. Nous regrettons aucune disposition relative. Aux outre-mer a été mis. Dans le texte. Je ne peux que me réjouir aujourd'hui enfin. Que Saint-Barthélemy obtiennent. Ce que ce que nous votons aujourd'hui mais. Je voudrais aussi profiter de l'occasion. Pour partager un peu avec. Mes collègues de Saint-Barthélemy. Venait aussi de garder comment fonctionne. En Polynésie. Il y a la Caisse de prévoyance sociale, et puis il y a tous les fonctionnaires d'État affiliés à la Sécurité sociale. Je peux vous garantir que c'est plus facile d'être. Affiliée à Larqué de prévoyance sociale que à la sécurité sociale surtout en matière. D'Évra ça ne en métropole ou de prise en charge en matière de santé, je vous le merci. Merci madame la présidente. Je félicite notre collègue Micheline Jacques pour son initiative. Et je tiens à dire que les 8 et 9 mars dernier. Donc il y a seulement quelques jours ont eu lieu en Guadeloupe, les 16ème journée de conférences de coopération régionale ainsi Guyenne. Des interventions de l'ARS de Guadeloupe, à Saint-Martin, c'est Barthélemy et de l'ARS de Martinique en permis de bien comprendre que nous étions tous. Complémentaires interdépendants. Surtout dans des situations critiques. Et c'est pour cela que je dirais. Que c'est important que nous puissions être solidaire, que nous continuons à être solidaires. Parce que en temps de crise. Nous sommes repliés sur nous-mêmes. Donc il est important aujourd'hui que je vous dise que nous devons continuer cette solidarité parce que le CHU de Guadeloupe. Malgré ces difficultés, malgré les difficultés budgétaires restera. Le lieu où les évacuations sanitaires continuera à se faire. Donc nous sommes toujours solidaire et en tant que sénatrice. Mais en tant que professionnel de santé, je ne peux que pouvoir continuer à vous dire que vous pouvez compter sur nous et compter sur la Guadeloupe merci. Merci madame la présidente, monsieur. Madame la ministre et j'ai un collègue. J'avoue n'avoir toujours pas compris. Le. Le fond de la différence, ce qui nous sépare. Je n'ai pas compris la vision différente exposés par la ministre. Et quel est le véritablement le motif je je n'ai pas très bien compris. Je l'avoue. Ensuite moi je félicite Micheline Jacques qui. Va plus loin et imprudence comme Michel, Michel a fait un texte, on le connaît tous sont là soutenus, bon il y a eu ici ou là quelques. Censures là elle va plus loin et en responsabilité sans pour autant dessaisir l'état d'une compétence sans vouloir aller dans l'autonomisation comme elle le dit le le texte prudent, d'autant plus que ça implique, si j'ose dire. La caisse. De la collectivité. J'avoue que j'ai, j'ai du mal à comprendre la la la différence ensuite puisque la ministre a évoqué. Un décret qui sera un prix très bientôt. Je lui dis puisque ça fait là aussi quelques longues années qu'on nous dit qu'un décret portant parité de rémunération des. Praticiens hospitaliers. Et des contractuels et c'est valable pour Saint Barthélemy bien c'est 20% c'est pas 40% de sur rémunération c'est 20% chaque fois qu'on demande au directeur de l'ARS. Quand est-ce que ce décret sera publié. On nous dit très bientôt, c'est à la signature. Ça fait 3 ans que c'est à la signature. Alors on aimerait bien que ce décret pour l'attractivité parce qu'on a des problèmes de recrutement et c'est le cas de Saint-Barthélemy. Eh bien que ce décret la soit également mon Dieu publié. Voilà donc on votera j'allais presque dire avec enthousiasme ce texte là donc. L'État fait l'unanimité contre lui. Merci monsieur le sénateur, je vais donc mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi organique visant à permettre à Saint-Barthélemy, de participer à l'exercice des compétences de l'État en application de l'article 59 du règlement le scrutin public et de droit. Et il va être procédé au scrutin public et le scrutin est ouvert.

On ne demande à voter le scrutin est clos. Votants 343. 343. Pour, 343 contre 0, le Sénat a donc adopté à l'unanimité. Bien je vais suspendre la séance quelques instants afin de permettre à chacun de s'installer pour le prochain point de l'ordre du jour, la séance est suspendue.

La séance est reprise. Et l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de zéro artificialisation nette au coeur des territoires présenté par Monsieur Jean Baptiste blanc Madame Valérie Létard et plusieurs de leurs collègues la procédure accélérée a été engagée sur ce texte. Dans la discussion générale. La parole est à madame Valérie Létard, autrice de la proposition de loi. Madame la présidente. Monsieur le rapporteur. Chers Jean-Baptiste Leblanc. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre. À l'heure où nous débutons cette discussion générale je souhaiterais vous lire quelques phrases. En matière d'artificialisation des sols. Le gouvernement propose des objectifs ambitieux mais se trompe sur la méthode. Il propose un dispositif extrêmement centralisée peu en prise avec la réalité du territoire français qui se caractérise par des dynamiques d'artificialisation très différentes. Il est à craindre que la compétence régionale ne donne davantage de poids aux revendications des métropoles et des zones urbanisées au détriment des territoires ruraux en outre la notion d'artificialisation nette n'est aujourd'hui ni défini ni mesuré par les collectivités ou par l'État. Enfin, la loi fixe des délais absolument irréaliste. Ces mots ne m'appartiennent pas, ce sont ceux de la commission des affaires économiques, il y a déjà de cela. Presque 2 ans. Au moment où notre assemblée avait examiné le projet de loi climat résilience. Il est frappant de constater. Qu'avant même l'adoption de cette loi fleuve en l'absence d'étude d'impact fournis par le gouvernement. Nous avions déjà pointé du doigt les problématiques qui nous réunissent aujourd'hui. Ce n'est un secret pour personne que la mise en oeuvre Dusan est aujourd'hui extrêmement compliqué à la fois par des problèmes d'ordre presque technique. Comme en ce qui concerne la nomenclature des sols artificialisés et d'autres éminemment politique, comme le degré de contrainte du document régionales ou les équilibres entre territoires. Je pense que ces problèmes proviennent au moins en partie d'une concertation insuffisante avec les élus, au moment de la loi climat résilience puis d'un certain défaut des coups de la part du gouvernement. Le Sénat avait déjà proposé certaines évolutions dès l'examen de la loi en 2021 comme une territorialisation plus poussée ou un décalage du calendrier de révisions des documents d'urbanisme. Elles avaient pourtant été rejetées dans la suite de la navette. Il nous a donc fallu remettre la loi climat résilience sur le métier d'abord dans le cadre de la loi 3DS pour prévoir les délais supplémentaires devant l'impossibilité des conférences des Scott à tenir le calendrier fixé par la loi. Puis il a fallu que les décrets d'application soient attaqués devant le Conseil d'État pour que le gouvernement admette l'inapplicabilité de la nomenclature des sols artificialisés et les carences du décret relatif aux sera Le chemin qui nous amène ici dans l'hémicycle pour examiner ce texte a donc été long. Il y a désormais consensus sur le fait qu'il faut modifier la loi et je pense que nous sénateurs et sénatrices. Avons fait un travail important pour mettre ce sujet en haut de l'agenda comme nous il enjoignait les élus locaux. Je veux à ce titre saluer le travail important de notre rapporteur Jean-Baptiste Leblanc au sein des murs du Palais comme en dehors, sur le terrain pour expliquer éclaircir améliorer la loi sur Lausanne. Je remercie aussi évidemment l'ensemble de nos collègues issus de tous les bancs qui ont participé à la mission conjointe de contrôle créée par le Sénat en septembre dernier qui a abouti au dépôt de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Dès l'examen de la loi climat résilience nous avions adopté une approche collective avec le rapport de monsieur Blanc Monsieur Redon Arazi et Madame Loisier. L'objectif than à l'épreuve des territoires. Nous nous sommes tous retrouvés en septembre dernier, autour de cette mission format inhabituel qui témoigne de la manière dont Lausanne envahi aujourd'hui toutes les politiques publiques tous nos débats de commission tous nos territoires. Le texte qui a émergé des travaux de la mission vise à répondre de manière très concrète aux difficultés d'application Dusan il s'est nourri de nos dizaines d'auditions et d'un travail approfondi sur les données je regrette à ce titre que nous n'ayons pas disposer de ces données précises dès l'examen de la loi car elles auraient pu nous éclairer plus précisément sur les choix que nous au Pérignon cet enjeu de transparence et d'étude de l'impact des textes et fondamental. Je tiens à le dire ici devant nous. Monsieur le Ministre, cette transparence sera aussi essentiel pour la suite de l'application Dusan et je pense notamment au traitement des grands projets ou encore à la collecte des données d'artificialisation je le disais, le chemin qui a mené cette proposition de loi a été long, malgré certaines annonces au cours des derniers mois, c'est le Sénat qui a dû prendre l'initiative de déposer un texte pour faire bouger les lignes. Législatives. Nous avons perdu un temps précieux, même s'il a finalement contribué à faire mûrir les réflexions de de part et d'autre. Je salue néanmoins le ministre Christophe Béchu ainsi que la ministre fort qui ont accepté le dialogue initié par le Sénat, autour de ce sujet complexe qu'ils ont hérité du gouvernement précédent et je remercie aussi le gouvernement d'avoir demandé le recours à la procédure accélérée sur ce texte, ce qui nous permettra en cas d'accord d'apporter plus rapidement les réponses qu'attendent les élus locaux qui se retrouvent en ce moment dans une situation intermédiaire qui est difficilement vivable. Je voudrais dire un mot plus général de la philosophie du texte présenté par la mission conjointe de contrôle que nous examinerons aujourd'hui d'abord c'est un texte qui vise à apporter davantage de pragmatisme et d'efficacité. Les imprécisions et le formalisme de la loi climat résilience complique énormément la tâche des élus locaux qui finalement sont les seuls à porter la responsabilité, pratique de l'atteinte des objectifs sans pour autant en avoir les outils. Il faut donc nous assurer que ce que la loi mette en place est effectivement applicable, que l'on ne crée pas un monstre administratif ni des situations absurdes. C'est aussi la raison pour laquelle nous plaidons pour davantage de temps car toutes les personnes auditionnées nous ont dit clairement que la qualité de la réflexion en amont permettra d'aller plus vite et plus efficacement. Ensuite cela justifie enfin d'offrir de nouveaux outils juridiques pour que les élus est efficacement effectivement la maîtrise concrète de l'artificialisation comme le sursis à statuer ou le droit de préemption spécifique Ozanne. Enfin c'est un texte qui vise à éviter la création de nouvelles inégalités. Le dispositif de territorialisation si absolument nécessaire peut présenter certains risques notamment celui que les grandes métropoles comme les communes urbaines quatre une grande partie des enveloppes futur d'artificialisation c'est un enjeu fondamental. Il faut permettre à chaque territoire urbain comme rural de réaliser son potentiel si Lausanne est perçue comme une nouvelle inégalité comme une mise sous cloche des territoires ruraux au profit de la consommation des zones urbaines comme organisant le sous-développement des de certains territoires. Alors il échouera. Il faut aussi prendre en compte les conséquences sociales Dusan que l'on pressant mais qui ne sont pas encore tangible. tangible. Car il entraînera une redistribution de la richesse des patrimoines attention ne pas créer des gilets jaunes Dusan les collectivités seront en prenant les ligne pour gérer les conséquences concrètes. C'est la raison pour laquelle nous proposons des mécanismes de pas réservé de surface minimale de développement communal conçu comme de vraies garanties au profit des territoires notamment ruraux. Il faut aussi que le système que nous mettons en place pour les 30 prochaines années, soit assez souple pour évoluer, pour prendre en compte l'imprévu et le nécessaire logique décennale ne veut pas dire immobilisme. Il faut pouvoir accueillir les grands projets de demain s'adapter aux évolutions démographiques ou économiques adapter les approches l'architecture du zen est aujourd'hui rigide, il nous faut y apporter de la souplesse, c'est l'objectif des dispositifs comme la part réservée prévues par le texte et l'intention derrière notre proposition d'une gouvernance plus large qui puisse suivre et adapter les trajectoires. Le chemin a été long et il n'est pas terminé, vous le savez Monsieur le Ministre, que le gouvernement a du pain sur la planche pour aller au bout du sujet, Dusan sans hypocrisie et sans idée préconçue. Mais je suis sûr qu'ensemble nous y arriverons. Il faudra c'est indéniable rebattre les cartes de la fiscalité, de l'Aménagement et du logement. Il faudra dégager de nouvelles ressources pour que les collectivités territoriales et les moyens de concret de piloter leur artificialisation de renaturer, de traiter les friches un fonds Vert n'y suffira pas. Ce sont des ressources durables d'ingénierie de fiscalité locale qu'il faut mobiliser je n'évoquerai pas les constats très franc de la Cour des comptes concernant les moyens de l'État déconcentrer. Nous savons tous ici, que malgré les bonnes volontés locales les collectivités sont bien souvent très seuls face à leurs obligations. Nous souhaitons que l'État prenne ses responsabilités pour que la décentralisation n'en est pas que le nom. Le chemin est encore long mais j'espère, nous espérons que nos discussions aujourd'hui permettront de faire aboutir bientôt ce texte qui sera un grand pas vers une application plus efficace et plus apaisé Dusan au coeur de nos territoires. Je remercie encore une fois l'ensemble de nos collègues sur tous les bancs qui. Dans la commission spéciale elles nous ont accordé leur confiance leur construction, leur esprit constructif, ainsi que notre rapporteur Jean-Baptiste Leblanc pour son écouter sa compétence. nous entamons le chemin à cette à ce moment à cet instant, il faut que nous aboutissions dans l'intérêt des territoires et je suis sûr que nous y arriverons. Une fois de plus. Monsieur Monsieur le rapporteur de la commission spéciale Jean-Baptiste Leblanc, vous avez la parole. Madame la présidente. Monsieur le Ministre. Mes chers collègues. Une nouvelle expression s'est donc imposé dans le débat public. Le zéro artificialisation nette sous une apparence assez technique, voire technocratique, ce terme recouvre une réalité qui s'impose d'ores et déjà au territoire et affectera peu à peu les modes de vie de nos concitoyens. Nous avons approuvé cet objectif, il y a 2 ans dans la loi climat et résilience nous ne le remettons pas en cause pardon aujourd'hui car l'enjeu du changement climatique et plus que jamais actuel. Toutefois, nous sommes à l'écoute des habitants et des élus et depuis des mois, nous alertons sur les difficultés pratiques auxquelles ils font face dans la mise en oeuvre des dispositions de la loi climat et résilience. C'est pour cela que la commission spéciale vous présente aujourd'hui un texte qui est issu de 18 mois de réflexion collective depuis l'entrée l'entrée en vigueur de la loi climat résilience. Il a été rédigé par une mission qui réunissait 4 commissions permanentes et qui à travailler au-delà des clivages politiques traditionnels. a poursuivi le travail dans des délais contraints est parvenu au texte que nous examinons aujourd'hui en rendant ces dispositions plus opérationnel, sans en modifier l'esprit général. C'est donc un travail de fond qui a été menée bien dans la tradition d'écoute qui est la marque de fabrique de du Sénat. je veux à mon tour à remercier une nouvelle fois l'ensemble des membres de la commission spéciale sur tous les bancs de cet hémicycle, à commencer par notre présidente Valérie Létard dont le travail a été essentiel et le compétences une fois de plus reconnu ce qui a favorisé l'atteinte. C'est un très large consensus. Merci Valérie. Pourtant ce le texte que nous vous présentons a été parfois présenté de manière un peu caricaturale. Non il ne remet pas en cause les dates cible de 2031 et 2050 fixé par la loi climat et résilience, il a juste seulement les dates intermédiaires d'ici à 2031 afin de rendre plus opérationnel le calendrier de modification des documents d'urbanisme. Non, la définition des grands projets retenus par la proposition de loi ne conduit pas un abandon des ambitions de réduction de l'artificialisation au contraire il responsabilise les acteurs non seulement les régions mais aussi l'État lui-même la proposition de mutualisation. À l'inverse dilue la responsabilité en la faisant peser sur des régions qui ne sont pas à l'origine de ces projets et qui ne bénéficient pas de la retombée, le texte présenté par la Commission spéciale n'est pas seulement une mesure de justice pour les régions en créant une incitation à réduire l'artificialisation des grands projets. Je crois qu'il renforce les chances les chances d'atteindre réellement les objectifs de sobriété foncière non la garantie du droit à l'hectare n'ajoute pas 35.000 hectares à l'artificialisation des sols en France c'est sans doute le chiffre le plus contestable qui a été avancé d'abord ce droit reste comptabilisés dans l'enveloppe régionale. Donc il ne portent pas du tout atteinte aux objectifs de 2031 2050. C'est seulement une répartition différente des droits à construire en outre la garantie rural comme toute garantie n'est activé qu'en cas de nécessité. C'est seulement eu pour une minorité de communes les plus rurales en général qu'elle aura un effet des communes qui n'ont pas forcément eu beaucoup de projets depuis 2011 mais qui est précisément pour cette raison pourrait en avoir quelques-uns dans les années à venir. Au total ces 9200 hectares environ qu'il faudra répartir différemment entre les communes, soit 7,5% du total. Je suis prêt à parier que cette garantie rural aura en réalité un effet positif sur l'atteinte des objectifs than car elle ne sera pas consommée par toutes les communes. Ces mesures ont un point commun, faciliter la mise en oeuvre des objectifs than c'est bien ce qui est inscrit dans l'intitulé de la proposition de loi qui précise, d'autre part au coeur des territoires. Car il n'y a rien de plus territoriale que la mise en oeuvre des objectifs de sobriété foncière. Rien ne sera fait sans les élus. Rien non plus ne devraient être faits contre car il représente tout simplement les habitants ils sont les mieux à même d'apprécier l'ensemble des besoins d'un territoire. C'est pourquoi le texte et cherche à leur apporter des outils Je pense à la conférence régionale. De gouvernance Dusan car de nombreuses communes avaient ressenti que leur parole n'avaient pas pu être entendu dans le fonctionnement actuel des conférences des Scott. La commission spéciale a en effet améliorer le fonctionnement afin de répondre à certaines des objections qui avait été faites et l'examen en séance permettra sans doute d'améliorer encore ce dispositif. Je pense aussi et surtout aux outils juridiques a apporté par la proposition de loi le sursis à statuer, le droit de préemption et le motif de refus d'autorisation d'urbanisme spécifique aux enjeux de lutte contre l'artificialisation des sols. La création ou le renforcement de ces outils ont été largement saluées lors des auditions que nous avons l'accès aux données est également un enjeu essentiel. Les élus constate dans bien des territoires que celles fournies par l'État sont insuffisantes et il est important qu'ils puissent utiliser celles qui proviennent des observatoires locaux je pense enfin à la prise en compte des spécificités de certains territoires par exemple ceux soumis au recul du trait de côte, ainsi qu'à la prise en compte et les efforts passés de sobriété foncière les débats restent réelles sur certains sujets Jean distinguerait de Monsieur le Ministre. S'agissant de la nomenclature des espaces artificialisés. Nous avons approuvé la souplesse apportée par le texte qui permet aux communes et EPCI de délimiter dans leurs documents d'urbanisme des périmètres au sein desquels l'artificialisation des surfaces herbacées n'est pas décompté car les appréciations varient selon les lieux. Dernier point et non des moindres, l'articulation entre les sera dettes et les documents d'urbanisme le. N'est pas un document d'urbanisme. Nous pensons nécessaire d'indiquer explicitement qui s'applique dans un rapport de prise en compte et non de compatibilité l'acceptabilité des des objectifs dans les territoires passe encore une fois, par la responsabilisation de l'ensemble des acteurs en particulier ceux à qui la loi attribue la compétence en urbanisme et non par la verticalité. Bien que la politique de sobriété foncière sont imposés pilotée au niveau national et régional, les élus locaux sont en première ligne. Ils n'ont pas bénéficié d'un soutien suffisant malgré la nouveauté et la complexité des enjeux. C'est à nous de leur donner les moyens et les outils pour mettre en oeuvre cette politique. La mise en oeuvre de la loi climat et résilience doit respecter les compétences et l'Intelligence collective de nos collectivités. Elle ne peut nous imposer d'organiser leur sous-développement. L'objectif est bien de concilier la sobriété frontière avec le développement harmonieux. Le gouvernement nous a d'ores et déjà écouté sur plusieurs points. Il a reconnu que l'artificialisation induite par les grands projets ne pouvait pas être comptabilisés intégralement sur les droits à construire de la région dans laquelle ils sont implantés. Il a admis une évolution du calendrier et la nécessité de préserver des possibilités de construire minimal dans les communes rurales. Il faut reconnaître et saluer ces avancées mais disons-le Monsieur le Ministre, ce n'est pas encore assez. Je sais que vous avez identifié les enjeux posés par Lausanne dans les territoires mais nous essaierons de vous convaincre que les réponses que vous proposez sont encore insuffisantes. Cette proposition de loi à vocation à poursuivre sa navette jusqu'au bout avec ce texte, le Sénat donne l'occasion d'ajuster les conditions de mise en oeuvre de la loi et le gouvernement là d'compris en déclarant la procédure accélérée, nous vous encourageons à favoriser à présent l'inscription la plus rapide possible lors du jour à l'Assemblée nationale. En effet, il faut aller vite. Ce texte s'inscrit dans un double calendrier celui de la révision du Sraddet qui doit s'achever, pour le mois d'avril 2024 et celui de la mise en oeuvre du moins 50%, il est essentiel de rang de la loi lisible opérationnel adapté aux réalités de nos collectivités, voilà bien l'objet du texte présenté aujourd'hui par la commission spéciale, je vous remercie. La parole est maintenant monsieur Christophe Béchu Ministre de la Transition écologique et de la cohésion du territoire. Madame la présidente. Mesdames et messieurs. Et sénatrices et sénateurs je salue. Les deux rapporteurs Valérie Létard et Jean-Baptiste Leblanc et et je vous indique d'emblée. Que l'état d'esprit qui est le mien en montant à cette tribune et plus largement, discutant avec vous des 210 amendements qui ont été déposés. Hé bien de trouver un chemin d'entente à une solution. Vous l'avez dit. Ce dispositif, il a été à il a été adopté. Dans le cadre de la loi climat et résilience un texte de 305 articles. Il a soulevé à la fois une forme d'enthousiasme. Par le fait que la France puisse prendre ce sujet de la lutte contre l'étalement urbain à bras le corps et parfois des difficultés de mise en oeuvre ou des incompréhensions dans la manière dont les choses allaient se passer. Dès mon arrivée au mois de juillet, j'ai eu des occasions d'échanger avec vous et très tôt, dès le mois de septembre. La question que ce soit un véhicule législatif. Qui viennent du Sénat. Et d'une proposition de loi qui soit déposé par la Haute Assemblée. Ah non seulement recueilli mon assentiment mais m'a souhaité la façon d'avancer. On est aujourd'hui. Au moment où les discussions comment et je veux devant vous. À partir du moment où j'ai entendu que l'objectif n'était pas de voter un texte pour envoyer un message mais bien de voter un texte qui ensuite permettent de modifier la loi. Pour préciser ce qui me semble être les sujets sur lesquels il sera facile d'avancer et ceux sur lesquels je pressens qu'il pourrait y avoir des difficultés, le moment venu, à l'occasion d'une commission mixte paritaire qui devrait ensuite nous permettent d'aboutir à un accord. D'abord je salue les propos à la fois écrits et oraux qui rappelle que. La question de la lutte contre l'artificialisation personne de la discute. Dans un contexte où je n'ai pas besoin de revenir devant vous sur le dérèglement climatique sur la nécessité d'atténuer notre empreinte environnementale. En insistant peut être. Sur le fait que un seul artificialiser ne stocke plus de CO2. Qu'il ait un espace stérile pour la biodiversité. Et qu'ils participent massivement au dérèglement du cycle de l'eau en empêchant la recharge des nappes phréatiques et en faisant ensuite en sorte d'accélérer les écoulements. Vous rappelez que la croissance que nous avons vécu deux l'artificialisation. A été marquée par le fait qu'elle s'est débridé au cours du dernier demi-siècle et qu'elle s'est totalement décorrélées de la progression de population. On a une artificialisation qui en termes d'efficacité d'accueil. A été 3 fois plus vite dans le dernier siècle que au cours. Des périodes précédentes du dernier demi-siècle Dans ces conditions. La perspective de diminuer. Par 2 la consommation d'espaces naturels sur la décennie en cours revient. D'abord à prolonger une baisse déjà observé de la consommation d'espaces naturels après le pic qu'on a atteint dans les années 80, vers des modèles où. Nous arrivions de 60.000 hectares par an à une situation au début de la décennie précédente, nous étions à 30.000 et où l'objectif quand on prend la moyenne de ces 10 dernières années, avec une consommation de l'ordre de 25.000 hectares par an en moyenne nous amène. Aux 12.500 qu'il faudrait attendre jusqu'en 2031. La marge d'après le zéro artificialisation nette. Il nous reste un peu de temps et je signale en passant. Qu'on passe parfois plus de temps à discuter de ce qui se passera après 2050 qu'entre 2031 et 2050 avec des enjeux qui pourtant me semble autrement plus importants à court ou moyen terme. Vous rappelez aussi au moment où nous commençons ces débats que il y a à l'échelle européenne. Une demi-douzaine de pays qui sont en engagés dans des procédures de ce type. C'est le cas de l'Allemagne de la Suisse de l'Espagne, de l'Italie, du Royaume-Uni, des Pays-Bas avec globalement la même philosophie diminuer puis tendre vers un zéro artificialisation nette dans un. Contexte où la question de la souveraineté alimentaire de l'Europe, où la question de sa réindustrialisation impose. De limiter l'artificialisation mais de faire en sorte malgré tout de continuer à accueillir des projets qui sont nécessaires, y compris dans une perspective de transition écologique. L'esprit de responsabilité et le souci du dialogue, qui sont constants. Au Sénat, ce texte en porte la marque à bien des égards, me conduit à remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à son élaboration. Et qui souhaite la convergence. De nos objectifs. Certaines dispositions que nous allons évoquer reçoivent. L'assentiment du gouvernement de manière totale. C'est le cas pour la prise en compte de la renaturation Avedon dont 1031. C'est le cas pour la mise en place de nouveaux outils pour les communes pour mieux maîtriser les projets avant 2031, je pensais l'extension du droit de préemption et la mise en place de périmètres de sursis à statuer. C'est le cas pour la communication aux communes des données dont elles ont besoin pour mesurer l'artificialisation c'est encore le cas pour la possibilité offerte aux communes littorales d'anticiper le recul du trait de côte dans la recomposition urbaine qu'il induit. Ces ajustements de bon sens. Ces modifications, nous semble indispensable préserve l'esprit et garantissent la possibilité de tenir les objectifs. Comme vous le savez les principales attentes exprimées par les collectivités, porte sur 2 sujets particuliers les grands projets nationaux et la création d'un mécanisme de garanties de développement pour les communes rurales. Je vous le dis comme je le pense, nous partageons l'objectif, il faut qu'on arrive à trouver le chemin, à la fois sur les grands projets et sur la garantie rural à ce stade. Non seulement nous sommes convaincus qu'il y a matière à compter, à part des grands projets d'état et nous parlons d'infrastructures. Mais la ligne qui pourrait nous séparer, c'est le fait de savoir si ces projets doivent être considérés comme n'étant même pas deux l'artificialisation qui doit faire l'objet d'un comté à part avec un décompte national. Il va de soi. Que si nous sortons des projets d'une trajectoire d'artificialisation et qu'en plus nous ouvrons la porte sur la catégorie des grands projets là, ça devient compliqué d'expliquer. Qu'on vise l'objectif est qu'on veut le tenir alors que nous n'avons pas de limite et pas d'étude d'impact sur ce que serait. L'ouverture de la porte sur ses grands projets d'envergure nationale. Ensuite sur la prise en compte spécifique des territoires ruraux. Je rejoins. Pleinement la nécessité de cette garantie rural évoquée par la Première ministre lors du congrès de. L'association des maires. Qui nous permettra de favoriser la revitalisation des territoires ruraux. Il faut qu'on s'entende sur les critères vous savez ma préférence sur le fait de raisonner en surface plutôt qu'on attribue un hectare pour tout le monde mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Là où nous avons un sujet sans doute plus complexe. C'est celui. Du décret dit sera sera être n'a pas de caractère prescriptif la quasi-totalité de l'échange que nous allons avoir. Va s'arrêter à une discussion sur le. La visée courtoise des objectifs mais sans mécanisme juridique qui nous permettra de tenir cette trajectoire et de l'tante. Je ne m'étendrai pas sur le décret nomenclature le travail avec les associations, de collectivités pour le réécrire est quasiment terminée, selon le calendrier qui avait été indiqué. Remise d'un rapport par la Fédération nationale des agents urbanisme avec plusieurs communes. Pour la fin du mois de novembre et réécriture du décret pour le printemps. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Le texte qui est soumis à votre examen comprend de très nombreuses dispositions bénéfique qui doivent nous permettre une meilleure mise en oeuvre de la trajectoire than et une meilleure appropriation. Par tous les acteurs cependant. Certaines de ces dispositions. Tout comme une partie des amendements qui ont été déposés qui viendront nourrir le débat. Me semble. Présenté le risque de vider de sa substance désengagement dont nous disons pourtant tout ce que nous y sommes attachés. En définitive, ce qui est en jeu c'est à la fois ce qu'est une trajectoire de sobriété foncière et aussi ce qu'elle n'est pas. Mettre en oeuvre, Lausanne. C'est bon pour lutter contre le dérèglement climatique et préserver la biodiversité. Je vous rappelle qu'un hectare c'est entre 190 et 290 tonnes. De CO2 non émis. Si nous ne les artificielle, ils ont pas et avec nous permettant de stocker. Je vous rappelle que mettre en neuf Lausanne. Ça n'est pas choisir l'environnement contre le développement. On ne va pas arrêter de construire. Nous avons 170.000 hectares de friches dans ce pays, dont près de 50.000 qui sont en zone tendue. Nous avons 1.100.000 logements qui sont vacants. Dans lequel il y a personne et qui pourtant ont fait l'objet de construction et de réalisation. La priorité. Elle est d'organiser une sobriété foncière. Qui est le prolongement de ce que les élus locaux ont d'ores et déjà commencé au travers des chiffres d'artificialisation. De l'articuler avec les besoins que nous avons au titre de la transition écologique. D'accueillir des infrastructures qui nous permettent d'accompagner notre décarbonation et de réindustrialiser notre pays et dans le même temps. De faire en sorte que nous puissions et continuer à accueillir nos concitoyens. Au moment où une partie de ceux pour lesquels nous construisons ce texte se montrent réticents à l'idée de signer des permis de construire, comme en atteste une partie du recul des mises en chantier sur le plan national, c'est dire. Si les discussions que nous allons avoir, elles sont nécessaires à la fois parce qu'elles sont attendus sur le terrain par des élus qui veulent des précisions. Et si dans le même temps, le maintien de l'objectif doit se conjuguer avec le souci permanent d'un point d'équilibre qui ne permettent pas seulement de rappeler des principes mais d'arriver à un texte qui puisse être adopté rapidement pour permettent d'enclencher cette trajectoire. C'est l'état d'esprit qui me guidera dans nos échanges. Dès cet instant. La parole est à madame Cécile Cukierman. Pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à travers cette intervention générale. Je réserverai bien évidemment intervention spécifique au moment du débat sur les amendements je veux peut être en préalable rappeler une chose, si nous sommes là aujourd'hui c'est parce que finalement. À l'image d'Aristote, l'homme est un animal politique et parce que nous faisons société parce qu'il y a maintenant des millénaires, l'homme a décidé. Et s'est sédentarisé. De prendre en compte son destin et d'aménager son territoire sans subir le territoire qui s'impose à lui. Si je dis cela, c'est parce que il ne faut pas je pense que nous ne trompe ions de débats. Oui il y a des enjeux aujourd'hui environnementaux. Il y a des enjeux à préserver le climat, pour pouvoir continuer de vivre sur la planète mais ne laissons pas penser en parallèle qu'il y aurait des, des qui n'aurait aucune responsabilité de l'environnement de leur commune et de la préservation de leurs espaces communal. Bien au contraire, je crois qu'il y a aujourd'hui des milliers et des milliers d'élus locaux qui ont au quotidien la volonté de préserver l'espace de leur territoire communal parfois soumis à de nombreuses contradictions. Contradictions environnementale contradictions sociales contradiction, contradiction agricole contradiction industrielle et qui au mieux cherche en tout cas toujours à projeter leur territoire vers demain et cela se traduit notamment par. Alors c'est vrai, dans mon département et c'est vrai dans beaucoup d'autres. Dans un certain nombre de villages. Si l'on ne fait rien. Ce que j'appelle le syndrome du village de La Belle au bois dormant menace beaucoup de villages des paysages qui se referme. Des paysages ou au nom de ne rien faire,

parce que je parlais de contradiction effectivement des élus locaux qui, sans vouloir se refaire ce refermement des paysages ont aussi le souci est bien de préserver des espaces naturels ici une réserve naturelle ici à travers un parc naturel ici à travers une zone humide ici à travers un certain nombre en tout cas d'. Qui permettront de pouvoir concilier les 2 et je crois que c'est fondamental parce que finalement en miroir des objectifs affichés par la loi climat et résilience de réduction de l'artificialisation des sols. Il demeure des impératifs tout aussi fondamentaux. À l'espèce humaine qui sont ceux des impératifs socio-économiques et donc nous devons également tenir compte, il y a tout d'abord l'enjeu d'autonomie alimentaire. Oui, nous devons continuer de soutenir l'installation agricole, de pouvoir développer dans notre dans notre pays une agriculture au service de toutes et de tous une agriculture qui n'accroît pas le marqueur de différenciation sociale entre les Françaises et les Français et qui permet à toutes et tous d'être nourri correctement. Il y a pour cela un acteur qui, monsieur le ministre doit demeurer engagée particulièrement aux côtés des des collectivités. C'est bien évidemment l'état et il nous faut revenir sur des politiques qui ont laissé, finalement, année après année défriche s'installer dans nos territoires des et des des logements qui demeurent vacants des entreprises qui, pour X ou Y raison je n'ouvrira pas le débat ici ont mis la clé sous la porte, laissant des hectares entiers aujourd'hui à la charge des collectivités sans que nous ne puissions y faire grand chose. Faute d'ailleurs souvent de moyens ton ingénierie comme moyens financiers. Il y a besoin dans cette France des sous-, préfectures, celles dont on a beaucoup parlé d'ailleurs ces derniers jours. De continuer d'accueillir des commerces des entreprises mais aussi des habitants de pérenniser des services publics pour pouvoir aménager le village et la ville de demain. Construire, ça ne veut donc pas dire forcément artificialiser je l'entends il y aura donc besoin en parallèle, y compris de cette proposition de loi d'une véritable action forte pour pouvoir requalifier réemployer les espaces fonciers existants parce qu'il est trop facile de dire qu'il faut reconstruire la ville sur la ville. Encore faut-il en donner les moyens aux élus locaux. 67% des intercommunalités déclare avoir refusé des projets d'implantation économique ou subi les déménagements d'entreprises par manque de foncier. C'est le CEREMA qu'il le dit. Alors bien évidemment, ce ne sera pas n'importe comment, ce sera pas n'importe quel prix. Mais je crois qu'à travers cette proposition de loi, nous avons la possibilité de redonner un peu de souplesse, un peu de visibilité et de capacité à aménager dans la va-t-elle notre territoire pour ces raisons, nous voterons pour cette proposition de loi. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission chère Valérie Létard. Monsieur le rapporteur. Chers Jean-Baptiste Leblanc, chers collègues, disons-le clairement, nul ne conteste la nécessité de sobriété foncière à la fois pour préserver notre agriculture mais aussi notre environnement. La preuve, Monsieur le Ministre, vous l'avez, vous l'avez vous-même rappelé la diminution significative de l'artificialisation passer de 60.000 hectares environ 20.000 hectares depuis les années 2000 qui atteste de la conscience et du sens de la responsabilité des élus locaux mais les dispositions actuelles de mise en oeuvre Dusan illustre parfaitement comment une bonne intention peut se transformer en absurdité, voire en impasse d'abord à cause de la pensée en silos que nous adorons qui cultive à chaque fois une bonne intention, mais qui se contredit. Réindustrialisation oui logement oui mais Anne non à cause de la dérive réglementaire qui contrevient à l'esprit du législateur, y a-t-il un meilleur exemple que les décrets d'application Dusan à cause de la vacuité d'une étude d'impact, mise en évidence par le CNE. À cause de l'impensé de l'équilibre territorial et du droit à l'espérance et à l'avenir de tous les territoires je vous sais gré, Monsieur le Ministre de partager notre envie de sortir de cette impasse et de reconnaître la démarche très constructive de la mission sénatoriale conduite par nos collègues Valérie l'État et Jean-Baptiste Leblanc donc je tiens à saluer la qualité du travail concrètement sur cette proposition de loi, je parlerai de deux amendements évoquerait un souhait le premier amendement porte sur la nécessaire prise en compte de la diversité de nos territoires et de la libre administration des collectivités en donnant droit à un accord local sur la gouvernance Dusan le second amendement porte sur l'exigence de réactivité mais aussi de réalisme et rappellent le danger de figer les choses à un instant T, en permettant qu'un projet d'intérêt général conforme aux enjeux environnementaux ou de souveraineté et qui apparaîtrait après la répartition des droits initial à l'artificialisation puisse voir le jour, par le recours au pouvoir réglementaire locale du préfet auquel le Sénat tient particulièrement après consultation de l'instance de gouvernance, régionale, usage et comme promis. Je conclurai par un souhait puissions nous tirer les leçons du passé par une fabrique de la loi moins hasardeuse et plus vertueuse et qui met en son coeur l'étude d'impact et l'évaluation. C'est ce qui fera l'objet des états généraux de la simplification ce jeudi au Sénat auquel nous aurons le grand plaisir de vous accueillir Monsieur le Ministre, comme chacun peut le supputer ici le groupe centriste votera ce texte qui servira tout à la fois la vertu et le bon sens et puisque Portalis veillent sur nous. Je voudrais nous rappeler collectivement que la loi est faite pour les hommes, les femmes aussi naturellement mais en tout cas les hommes et les femmes doivent être entendus et eux ne sont pas fait forcément pour des lois qui sont un peu mal faite je vous remercie. La parole est à monsieur Éric Gold pour cinq minutes pour le groupe RDSE. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission spéciale. Monsieur le rapporteur, chers collègues. Moins de 2 ans après la promulgation de la loi climat et résilience, qui a été qui a créé les objectifs du zéro artificialisation nette des sols. Nous voici déjà quasi contraints d'en modifier les paramètres. La complexité et l'opacité du dispositif ont entraîné tant d'incompréhension de frustration qu'il était indispensable d'opérer certains ajustements sous peine de voir ces mesures essentielles raté leur cible. Mais la frustration est bien plus ancienne. Depuis notamment que certains EPCI ont atteint une taille si grande que certains maires de communes rurales se sentent exclus de la politique d'aménagement du territoire. Aussi c'est de simplicité et de souplesse. Nous, nous avons besoin pour que chaque élu local soit en capacité de s'approprier ces outils qui permettront de développer chaque territoire dans le respect des objectifs de transition écologique que le pays s'est fixé. L'artificialisation est aujourd'hui la première cause de l'érosion de la biodiversité en France en 40 ans, elle a progressé de 70 pour son quand la population n'a augmenté que de 19 pour 130.000 hectares d'espaces naturels sont consommés chaque année majoritairement au profit du logement. Or ces conséquences néfastes sont bien connus altération durable des fonctions écologiques du sol. Augmentation des risques naturels par le ruissellement atteinte au potentiel de production agricole et du stockage de carbone et dans le cas de l'étalement urbain, augmentation des émissions de gaz à effet de serre à la dépendance à la voiture individuelle. L'alerte rouge. Climatique a été lancé et la France, il a répondu en se fixant des objectifs ambitieux mais que faire des objectifs s'ils ne s'accompagne pas de mesures applicables. L'ambition est de réduire par 2 d'ici 2031, le rythme de consommation d'espaces naturels et d'atteindre d'ici 2050 le zéro artificialisation nette des sols. C'est-à-dire que pour chaque parcelle. Nous devons rendre une parcelle équivalente à la nature. Les sénateurs ont souscrit à cet objectif en 2021 tout en posant de principes fondamentaux. Un lien souple entre documents d'urbanisme régionaux et locaux et une différenciation locale plutôt qu'une application uniforme et purement mathématique. Force est de constater que les décrets d'application ne répondent pas à ses exigences et que persiste un manque de visibilité d'accompagnement alors même que les documents de planifications régionaux doivent être modifiée d'ici 2024. Représentants des élus locaux. Nous ne pouvions rester inactifs devant les difficultés et les inquiétudes soulevées. Cette proposition de loi tente d'y répondre. Nous souscrivons au report d'un an pour la déclinaison des objectifs au sein des documents de planification et d'urbanisme. Le calendrier n'était pas tenable. En l'état, notamment parce qu'il manque encore de nombreux outils d'information à la main des collectivités, à commencer par l'essentiel, l'accès aux données relatives à la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers. Nous partageons la volonté des auteurs de la proposition de loi d'assouplir. Il y a la hiérarchie des normes entre les documents d'urbanisme et de planification. Dans le cadre des Scott des épais lui écarte communale. Les élus devront désormais prendre en compte les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols fixé par les documents régionaux au lieu d'un rapport de compatibilité. S'agit danse de la surface minimale d'un hectare. Bleu par commune jusqu'en 2031. Nous soutenons cette mesure qui garantit aux communes rurales la capacité de se développer et de répondre à leurs besoins locaux, notamment en service public. Concernant l'article IV. Relatif à la compatibilité compta qu'on stabilisation pardon des grands projets de construction au sein d'une enveloppe nationale il était urgent de répondre à cette problématique, sans quoi nous risquons de priver fortement les régions des droits à construire, du simple fait d'accueillir un projet d'envergure nationale européenne. Cependant. Nous maintenons notre proposition d'intégrer tous les bâtiments et services publics à cette enveloppe nationale pour favoriser la solidarité entre les territoires. En effet, la définition des projets devant se situer sur l'enveloppe nationale régionale et supra-communal pourrait virer au casse-tête. Enfin. Si nous comprenons l'intérêt d'améliorer le dialogue territorial. Il est illusoire de croire que les nouvelles conférence régionale composée de plus de 56 membres qui n'ont aucun droit de propositions, des projets régleront le problème de la prise en compte des besoins des territoires ruraux. En ce sens, l'article 3 ne nous paraît pas nécessaire. Le groupe RDSE votera ce texte mais souhaite avant tout passer un message de lisibilité de simplification pour les élus locaux. Il n'est pas normal que, même pour nous qui sommes habitués à voter des lois parfois ardu ce sujet des ânes demeure aussi complexe. nous appelons à trouver des sources de financement plus dynamique pour les communes sans quoi leur développement continuera à se jouer sur l'arrivée de nouveaux habitants et donc la construction de nouveaux logements. Je vous remercie. La parole est maintenant à monsieur Philippe Bas pour le groupe Les Républicains monsieur le 1er questeur, vous avez la parole. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, présidente de la Commission spéciale rapporteur, mes chers collègues. Je voudrais vous dire qu'il me paraît essentiel aujourd'hui d'intégrer l'objectif du zéro artificialisation nette à une politique. De développement durable. Qu'est-ce qu'une politique de développement durable. C'est une politique qui ne se contente pas de la protection de l'environnement mais qui. Comme le dit l'article 6 de la charte de l'environnement concilie. Protection de l'environnement. Développement économique et progrès social. Nous en sommes encore loin. Si, comme le montrent les premières interventions à cette tribune. Il y a un accord général. Sur la nécessité de la sobriété en matière de consommation foncière pour protéger la biodiversité pour défendre l'agriculture. Pour maintenir nos paysages pour éviter. La saturation des grandes métropoles les des territoires. Qui en sont l'arrière-pays. l'être également indispensable de donner la priorité à la réaffectation des logements vacants et au redéploiement des friches. Il y a aussi la nécessité de tenir compte. Des exigences du développement de nos territoires. Ruraux dans la mise en oeuvre de cet objectif. Or jusqu'à. Maintenant. Le processus qui a été engagé par son caractère exagérément étatique menace de. Déséquilibre profond. La mise en oeuvre de cette. Planification. Il faut que aujourd'hui nous réussissions par ce texte qui fait l'objet d'un très large consensus de la gauche à la droite en passant par le Centre à trouver les voies et moyens d'une approche plus consensuel de cette difficulté qui. S'impose. Au regard de tous les élus de notre pays. La planification. Ne doit plus être une planification descendante mais reposé sur l'initiative des élus locaux. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas que le schéma régional s'impose comme un document d'urbanisme supérieur à tous les à tous les autres mais plutôt. Existe en tant que recommandations les pouvoirs des maires en matière d'urbanisme. C'est l'essentiel de la grande décentralisation de 1982 que l'État ne récupère pas les pouvoirs qu'il a laissée aux communes mais surtout il était essentiel que nous réussissions à lever les obstacles mis au rééquilibrage du territoire national et que nous fassions en sorte qu'une nouvelle politique de l'aménagement du territoire et du développement des territoires puissent être mises en oeuvre sans être entravés par l'objectif du zéro artificialisation nette. Or justement depuis la crise sanitaire nous constatons dans tous nos territoires une forte demande de migration venant des territoires métropolitains. L'expérience du confinement, mais aussi le développement de nouvelles formes de travail avec le télétravail fonte espérer de nouveaux modes de vie par beaucoup. De concitoyens du monde urbain ou péri-urbain. Allons-nous laisser passer cette chance de mettre en oeuvre une nouvelle politique d'aménagement du territoire qui correspond au souhait profond des Français. Allons-nous interdire à nos bourgs ruraux de se développer, alors que la demande existe et que leur développement ne contredit en rien les exigences de la protection de la biodiversité et de l'environnement cette chance. Il nous faut absolument la saisir et c'est la raison pour laquelle vraiment je veux rendre hommage au travail de notre commission spéciale de sa présidente de notre rapporteur qui ont réussi à rapprocher les points de vue pour. Rédiger un texte qui me paraît particulièrement équilibré car il ne laisse de côté. Aucune des exigences qui doivent s'appliquer au traitement de cet objectif du zéro artificialisation nette. Je le disais tout à l'heure. sera être ne doit pas s'imposer aux documents d'urbanisme. Le calendrier de son élaboration doit permettre la. La concertation, le décompte des projets nationaux et. Régionaux, on doit pouvoir se faire dans de bonnes conditions les droits minimum à construire dans les bourgs ruraux, le fameux droit à l'hectare doit être respecté. La prise en compte des espaces submergé par le recul du trait de côte doit se faire dans le respect des droits à construire dans les communes littorales et enfin il est important de continuer à assouplir l'objectif du zéro artificialisation nette pour les bâtiments agricoles, des amendements particulièrement pertinent ont été présentés pour obtenir ce résultat. Voilà, mes chers collègues. Ce que je voulais vous dire, en espérant que nous saurons manifesté une volonté sénatoriale puissante que l'Assemblée nationale, comme le gouvernement devront prendre en compte. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission spéciale. Monsieur le rapporteur. Cela L'artificialisation des sols doit faire l'objet d'une attention particulière dans notre pays, ce n'est plus un sujet de controverse. Nous nous sommes fixés collectivement des règles de réduction dans ce domaine. Cela fait maintenant. L'unanimité nous le disons tous ici depuis tout à l'heure. Ce que nous nous apprêtons à faire aujourd'hui, c'est rendre ces règles plus applicable et en prise avec la réalité des territoires. Là encore, c'est tout simplement du bon sens et cela répond aux inquiétudes du terrain qui nous remonte. Je me réjouis que ça se passe ici dans cette enceinte qui connaît si bien le rythme de nos territoires. Leur particularité, leur histoire et tout ce dont ils sont capables dans cette enceinte. Monsieur le Ministre, que vous connaissez particulièrement bien. Nos transition. Quelle qu'elle soit viendront du dynamisme du terrain des femmes et des hommes qui crée et des élus qui les accompagnent et nous sommes ici les représentants de ses élus et de ses territoires. Je salue ici. Votre travail. Monsieur le Ministre, votre engagement. Vous avez su être à l'écoute. Dès que vous avez hérité du dossier. Et ce n'était pas un dossier facile. Suspension des décrets proposition de réécriture débats et éclaircissements lors des échanges notamment avec la mission d'information, puis avec la Commission spéciale et enfin ça a été rappelé par madame la présidente, choix de la procédure accélérée pour cette PPL sénatoriale. Cela en fait. Officiellement le véhicule législatif privilégié pour faire évoluer notre réglementation. C'est un sujet. On l'a compris, éminemment complexe. Nous sommes sur une véritable ligne de crête. D'une part les objectifs de sobriété doivent être respectées. D'autre part, nous devons les adapter aux réalités. C'est l'objectif que nous avions au sein de la commission spéciale avec notre collègue Joël Guerriau avec moi même nous avons représenter le groupe les indépendants. Je me félicite. Des discussions concrètes que nous avons eu et du travail exigeant du rapporteur Jean-Baptiste Leblanc. Des membres de la commission spéciale et de sa présidente, Valérie Létard. Lausanne c'est laisser s'exprimer des visions souvent différente. Parfois contradictoires. Mais dont l'esprit convergent toujours vers la protection et la réussite de nos territoires. Nos efforts se sont tournés vers le respect de leurs caractéristiques et de leur évolution prochaine. Nous avons souhaité prendre en compte les efforts déjà fournis par beaucoup d'entre eux. Notamment les plus ruraux. La protection de l'environnement ne peut évidemment pas. Être se faire au détriment des territoires ruraux. Parmi tant d'autres. Je voudrais citer 3 sujets. Tout d'abord. Ça a été évoqué la comptabilisation des projets d'ampleur et d'intérêt au sein des objectifs Dusan. Notre réindustrialisation passera par ces projets. 2ème sujet. La surface minimale de développement communal. Entre le droit à l'hectare et le 1% rurale qui vont manifestement animé nos débats. Un terrain d'entente pourrait se situer dans l'amendement j'ai déposé avec le sénateur Alain Marc et qui propose un hectare pour les communes dont l'artificialisation est inférieur à 3% c'est-à-dire inférieur aux 7 9 % d'artifice. D'artificialisation qui est la moyenne nationale. Une voie médiane de ce type qui propose une juste balance pourrait être retrouvés. Je ne doute pas que nous allons parvenir à un consensus sur cette base ou toute autre. 3ème sujet. Enfin la renaturalisation et là des artificialisation des zones exposées au recul du trait de côte de Guérande à Saint-Jean-de-Luz. Avec le changement climatique. C'est un sujet auquel nous allons être confrontés de manière récurrente. Nous devons prévoir les aménagements nécessaires et poser un cadre précis. Voilà, mes chers collègues je ne doute pas que nous garderons collectivement chevillée au corps, l'intérêt des Français. Et que nous ajusteront nos objectifs pour rendre notre transition à la fois possible et équilibré. C'est en tout cas l'état d'esprit du groupe les indépendants. Je vous remercie. Parole est

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission spéciale. Monsieur le rapporteur. Cela a déjà été souligné le rythme d'artificialisation de nos espaces naturels agricoles et forestiers les Hénaff est absolument insupportable. Il remet en cause notre autonomie alimentaire la biodiversité de nos territoires. Nos capacités de stockage du carbone. C'est fort de ce constat que la Convention citoyenne pour le climat avait fait de l'objectif du zéro artificialisation nette une de ses propositions les plus fortes. Nous le savons, l'engagement du président de la République de reprendre sans filtre les propositions de la convention n'a pas été tenues et vraiment pas tenu engendrant une immense déception de la part des 150 citoyens tirés au sort. Néanmoins, une mesure forte et passer à travers les mailles d'un tamis politique et technocratique, pourtant particulièrement serré et cette mesure, c'est l'objectif du zéro artificialisation nette en 2050, inscrit dans la loi climat et résilience de Barbara Pompili. Cet objectif est ambitieux car aideront avait bien des logiques de développement il rompt avec la course à l'installation de surface commerciale et de nouveaux habitants dont les conséquences sont particulièrement visible dans nos territoires entre lotissement ses talents dans les périphéries des bourgs et zones commerciales de nos entrées de villes. Il est aussi juste de dire qu'avant même la loi than une prise de conscience était déjà à l'oeuvre sur le caractère intenable de ce modèle de développement sur la nécessité de réduire la consommation des Hénaff déjà dans bien des territoires, la taille des jardins des lotissements par exemple s'étaient fortement réduites. La loi climat et résilience, a le mérite d'accélérer le rythme pour atteindre les objectifs que nous nous sommes collectivement fixés et nous soutenons donc clairement l'objectif Dusan il a c'est vrai inquiétait les élus locaux et le Sénat s'en fait l'écho de fait des difficultés réelles n'étaient pas résolus par le caractère un peu mécanique de l'application des objectifs initiaux le moins 50% entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie passée appliquée à tous les territoires, quels que soient les efforts déjà effectuées par les territoires les plus responsable. Il fallait aussi un nécessaire éclaircissement dans la prise en compte des grands projets nationaux qui ne pouvait être intégrés dans le décompte locale. La création d'une commission spéciale au Sénat pour répondre à ces questions et aboutir à une proposition de loi était donc tout à fait légitime et je souligne l'importance du travail mené par la présidente et le rapporteur. Le groupe écologiste ce ainsi plusieurs propositions de cette PPL mais. Car il y a vraiment un très gros mais ne peut pour autant soutenir plusieurs propositions importantes. 3 mesures, nous sommes particulièrement problématique et me semble rejoint les préoccupations de Monsieur le Ministre, tout d'abord si nous soutenons la création d'un compte spécial pour les projets d'envergure nationale. Il n'est pas possible de les passer purement et simplement par pertes et profits sans les réaffecter aux enveloppes régionales suivant une règle a précisé sinon on remet simplement en cause l'idée même Dusan. À ce stade, vous le savez, ce point n'est pas éclaircie et il reviendra aussi à l'État de préciser comment il s'applique à lui-même cet objectif de réduction de la consommation des Terres naturelles agricoles et forestières. Ensuite, si nous soutenons les processus de renforcement en amont de la concertation avec une conférence inter-Scott Uzan renforcée. Nous ne pouvons remettre en cause le rapport de compatibilité, dans le fascicule. Entre le Fradette le Scott et le plus sauf à prendre le risque que les élus de certains territoires ne ne rejoue le match en aval ce qui conduirait à une multiplication des contentieux et rate nantissement évident de la mise en oeuvre d'usage. L'ajout des terrains herbacées des particuliers dans la nomenclature après 2031 est une véritable aberration qui pourraient permettre des lotissements avec de plus grandes parcelles de jardin dans la période 2031 2050 que dans la précédente décennie la comptabilisation se fait sur la base de la consommation des Hénaff. C'est aberrant. Ce point est pour nous un grand sujet de préoccupation. Il découle aussi il faut le souligner d'un changement de méthode dont nous aurions probablement pu nous passer en restant sur la logique de préservation des Hénaff jusqu'en 2005 nous déposerons ainsi un amendement en ce sens qu'il propose aussi de préciser ce qui est vraiment une grande faiblesse de cette loi les consommations maximale de foncier entre 2031 et 2041 et 2041 et 2050 avec une nécessaire décélération progressive qui nous amène au zéro artificialisation en 2005 ans ces 3 points s'il devait rester dans la PPL ne nous permettront pas de la voter, même si elle ne remet pas en cause. Je souligne l'objectif Dusan en 2050 un enjeu environnemental majeur Jérôme. Merci Merci la parole est maintenant Monsieur Bernard buis pour le groupe RDPI. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission spéciale. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. En 50 ans, nous avons plus artificialisés dans notre pays, quand 500. Concrètement. En France, entre 20.000 et 30.000 hectares sont. Artificialisés chaque année. Une artificialisation qui augmentent quasiment quatre fois plus vite que la population et cela a des répercussions directes sur la qualité de vie de nos concitoyens mais aussi sur l'environnement. Cette artificialisation est préjudiciable à la biodiversité et au climat. Parmi les vices de l'artificialisation des sols en rappellera par exemple que sols artificialisés. N'absorbe plus le CO2 ou encore l'eau de pluie. Et le danger est réel en cas de fortes intempéries. Les phénomènes de ruissellement et d'inondations sont amplifiés. Les nappes phréatiques se renouvelle plus difficilement du fait de cette imperméabilisation des sols et les fortes pluies emportent tout sur leur passage. Il nous faut également veiller au développement durable de notre agriculture et à notre souveraineté alimentaire nous défendons tous le développement d'une agriculture nationale garante de notre indépendance alimentaire et pour cela il faut agir. Voter dans le cadre du projet de loi climat et résilience et traduisent heures la feuille de route européenne. L'objectif de parvenir à zéro artificialisation nette est ambitieux et à la mesure de l'urgence. Pour ce faire, la réduction de moitié du rythme de la consommation d'espace dans les 10 prochaines années, nous paraît être une mesure de bon sens, mais doit se faire dans la concertation avec pragmatisme, souplesse et en lien Direct avec les élus de nos territoires. C'est l'objet de cette proposition de loi sénatoriale, fruit de consultations et de travaux expertisée par notre assemblée depuis la promulgation de la loi climat et résilience une pro position de loi qui permet de prendre en compte un certains nombres d'évolution et les préoccupations des élus locaux car en cela je vous rejoins quand il s'agit de légiférer, il faut trouver la juste mesure afin de ne pas imposer à quiconque. Un effort qui ne serait pas en mesure d'atteindre. Mais je tiens tout de même à rappeler que la loi climat résilience avait fait l'objet d'un accord important en CMP et je n'oublie pas que ceux qui appellent aujourd'hui à revenir sur le compromis trouvé dans la loi climat et résilience ce jury réjouissait hier d'avoir abouti à une rédaction équilibrée. Un seul à Lausanne. Toute la complexité du défi de la transition écologique. Tout le monde s'accorde sur le constat et la nécessité d'agir mais personne ou presque ne s'accordent sur les moyens d'y parvenir. La clé est alors dans la juste mesure des objectifs que nous nous fixons et dans une gouvernance suffisamment souple et proche du terrain pour accompagner le changement et ajuster les efforts en moyenne chacun sans pour autant perdre le cap. Je le dis ici avec force. Il nous faut modifier la loi sur la ZAD. Nous avons entendu les inquiétudes des élus locaux dans les auditions que nous avons menées au sein de la mission de contrôle lors de son audition, monsieur le ministre a également rejoint notre volonté d'agir. Faisant d'ailleurs la part belle à notre travail sénatorial mon groupe partage un grand nombre des préconisations de ce texte. Nous avons toutefois quelques interrogations sur l'article 7 relatif à la garantie rural. Favorable au principe d'une garantie rural. Nous restons toutefois dubitatif à ce que l'on attribue de manière arbitraire hectare à toutes les communes sans prendre en compte des réalités locales. C'est une bien curieuse manière de répartir l'effort au plus près des territoires. Je le vois très bien chez moi dans la Drôme, que ça soit pour la commune de rouge proche fourche à avec un seul habitant celle de La Bâtie défend avec 2 habitants ou bien ma commune de lait. J'habite à la chambre dit, ouah, commune de 50 habitants à quoi rimerait donc une telle proposition. En l'état, nous sommes donc globalement favorable à une grande partie des mesures visant à répondre aux interrogations des maires je pense par exemple à la prise en compte des projets d'envergure nationale a décompté des autres projets. N'oublions pas d'ailleurs que les délais fixés d'un climat et résilience ont déjà commencé à courir depuis 2 ans. Mais je rappelle également que nous considérons comme aux ciel de disposer d'un document d'urbanisme contraignant. Il doit donc subsister un lien de compatibilité entre l'Austra dette et le Scott c'est essentiel si nous voulons respecter nos objectifs de réduction de l'artificialisation chers collègues. Attention à ne pas perdre de vue notre cap et à ne pas abandonner aujourd'hui nos préoccupations d'hier. Je partage l'esprit et l'ambition de cette PPL mais je m'étonne des propositions de certaines nos collègues qui reviendrait à balayer purement et simplement nos engagements car je me souviens ce que l'un de vous déclarer à ce sujet lors de l'examen du projet de loi climat et résilience, oui il y a des impacts. Oui il y a des résistances, oui il y a des enjeux économiques et sociaux. Oui il y a des adaptations complexes mais c'est un mal nécessaire une dette que nous détenons envers les générations futures. Que diriez-vous aujourd'hui. Une autre de nos collègues nous reprocher au contraire des renoncements nous accusant de briser les promesses et de ne pas nous donner les moyens de répondre à la feuille de route initiale, un autre en fait nous infirmer l'examen sénatoriales de climat résilience devait avoir une seule finalité, le rehaussement de son ambition. Attention donc à ne pas balayer d'un revers de main, ces belles déclarations et à procéder aux ajustements nécessaires sans toutefois perdre de vue l'ambition initiale. Pour toutes ces raisons, nous soutiendrons les mesures d'adaptation des objectifs Dusan aux réalités territoriales les assouplissements bienvenus au service des élus locaux. Mais nous resterons vigilants quant au respect des grands objectifs que je viens de rappeler notre groupe ajustera donc son vote en fonction du sort des amendements discutés en séance et des évolutions du texte. Je vous remercie. La parole est maintenant à monsieur Christian renonce Arazi pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la présidente. Monsieur le ministre. Madame la présidente de la commission spéciale. Monsieur le rapporteur. La question de la déclinaison de l'objectif de zéro artificialisation nette dans les territoires et sans doute le sujet qui depuis la promulgation de la loi climat et résilience constitue la principale préoccupation de nos élus, quelle que soit leur département et leur sensibilité politique. Leur inquiétude attrait aux 4 points suivants. Donc quels sont les outils pour freiner les développements très consommateurs d'espace et respecter le calendrier imposé comment répartir l'effort de réduction de l'artificialisation d'un territoire à l'autre comment associer les collectivités du bloc communal aux décisions structurantes qui seront prises à l'échelle régionale et quelle place pour les grands projets d'avenir dans le modèle Dusan. En résumé, comment réussir à articuler les objectifs légitimes de sobriété foncière avec le développement des territoires, les zones les plus rurales craignent en effet de devenir la voilà à la valeur d'ajustement des zones plus attractive et d'être empêchée dans leur projet de de développement société et développement peuvent apparaître comme une injonction paradoxale et à cet égard, je tiens à souligner que le groupe socialiste n'a jamais remis en cause l'objectif Dusan comme d'ailleurs la plupart des maires et des élus. En témoignent les résultats de l'enquête qui avait été conduite par la commission des Affaires étrangères pour autant il faut entendre les craintes des élus et nous estimons que la différenciation locale demeure en l'espèce un sujet essentiel pour répondent nous demandons simplement au gouvernement de la lisibilité une concertation ascendante une égalité de traitement entre les territoires une implication de l'État pour les grands projets d'intérêt général et des moyens d'accompagnement. En réalité, nous suivons attentivement cette question depuis les travaux préparatoires du projet de loi climat résilience. Il y a 2 ans maintenant. En mai 2021, un groupe de travail spécifiquement avait été créée à l'initiative de la commission des affaires économiques de la trentaine d'auditions menées auprès d'acteurs de l'aménagement du territoire, notre rapport avait proposé

À la levée de boucliers des élus locaux contre l'objectif. Le Sénat il y a répondu en proposant dans un 1er temps une consultation en ligne des élus locaux. Le constat qui en fut tiré fut simple le cap Dusan est perfectible et doit être précisée et complétée. Pour ce faire, la mission de conjointe le contrôle créé en septembre 2022 à l'initiative des 4 commissions permanentes du Sénat réalisé ainsi que d'auditions qui ont débouché sur la présente, proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Elle contient 13 articles articulée autour de 4 axes, le dialogue territorial et la gouvernance, l'accompagnement des projets structurants structurant de demain. La prise en compte des spécificités des territoires et la préparation de la transition vers Les sénateurs socialistes ont proposé plusieurs enrichissement essentiels qui ont été retenus par la commission. Tout d'abord le maintien de l'objectif de sobriété foncière telle qu'adoptée dans la loi climat. L'article 4 prévoit désormais que l'artificialisation des sols résultant des projets d'intérêt national fasse l'objet d'une comptabilisation séparés et d'une trajectoire spécifiques d'atteinte des objectifs Dusan placé sous la responsabilité de l'État un rapport du gouvernement présentera tous les 3 ans, l'état d'avancement des projets et surtout les actions du rythme de réduction du rythme de cette artificialisation que l'État entend mettre en oeuvre pour respecter ses propres engagements. L'utilisation des friches l'appartement lui appartenant. Le financement où là où les actions de renaturation. Nous avons aussi obtenu une comptabilisation de l'artificialisation. Des projets d'envergure régionale au sein des seconde avancer l'arrêt la réappropriation des fiches qui défrichent qui sont autant de terrain disponible pour être réinvestis ou renaturer. Compte tenu de l'importance des enjeux de territorialisation et de mutualisation des territoires pourront désormais bénéficier en toute transparence de l'État exhaustif et documenté du stock disponible. Des détails sur la localisation des terrains par département sur leur nature leur statut juridique ainsi qu'une estimation des coûts des opérations de renaturation lors de l'examen de du texte en séance publique nous souhaitons formuler des propositions sur la réhabilitation du bâti existant car elle correspond à la fois aux objectifs Dusan et au besoin en logements de nouvelles activités dans les territoires ruraux. Un amendement un amendement proposera des dispositions spécifiques pour les bâtiments agricoles. De même, nous proposerons un article additionnel. dira l'artificialisation issus de projets de construction ou d'aménagement pour des opérations destinées à la réalisation de programmes comportant majoritairement des logements sociaux. Monsieur le Ministre, quelques points vont devoir être réglée devant nous. Durant nos débats les modalités de mise en oeuvre de la garantie rural le choix du rapport de compatibilité. Et ou

Il nous faudra ensuite aborder la nécessaire suite qui s'imposera après le vote de cette loi, à savoir l'aspect fiscalité et financement qui est comme toujours le sujet qui fâche le plus en tout cas je salue Monsieur le Ministre votre volonté de laisser au Sénat la primauté des améliorations à apporter pour une application raisonnée Dusan cette question concerne évidemment en 1er lieu le territoire et leurs élus. J'espère donc que nos débats et la CMP qui suivra seront rapidement conclusif et nous aurons obtenu l'essentiel que nos mères disposent enfin des clés d'application pour tenir cet objectif. Merci la parole est maintenant Madame, Sonia de la Provoté pour le groupe Union centriste.

Madame la présidente, monsieur le ministre de madame la présidente de la commission spéciale. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues je tiens avant toute chose, a salué le travail de madame la présidente, monsieur le rapporteur, et les membres de la commission spéciale sur cette proposition de loi qui a surtout cherché à rendre le zéro artificialisation nette le fameux Anne acceptables par tous les territoires. Cette PPL porte l'équité au-delà des dogmatismes avec réalisme et pragmatisme. Si la sobriété foncière est un objectif nécessaire pour affronter le défi de l'urgence climatique. Sa mise en oeuvre nécessite un travail sur le terrain où chaque voix de chaque territoire doit être entendu, chaque discussion rendu possible et être le résultat de la prise en compte des solidarités territoriales. Cette PPL favorise donc le dialogue territorial renforçant la gouvernance décentralisée, elle accompagne les projets structurants de demain prend mieux en compte les des spécificités des territoires et prévoit les outils techniques et réglementaires facilitateurs l'équité par la solidarité territoriale consenti et discuter entre tous, c'est la clé de la réussite de l'objectif de la sobriété foncière. Dans l'article de la loi. Climat et résilience portant sur le zone reviennent souvent les termes décliné déclinaison. La logique hé bien central et descendante. Pour les élus de terrain que nous sommes ou avons été ou pour ceux aux noms desquels nous nous exprimons, nous savons que ce ce que ce que la loi décline l'état l'impose. Les quelques décrets déjà trop vite, paru en sont la parfaite illustration. Or l'application Dusan à l'ensemble du territoire et des politiques publiques conduit les élus locaux à subir des injonctions contradictoires permanentes c'est Lausanne plus garantir l'accès aux services publics et para-publics essentiels plus assurer notre survie de souveraineté industrielle alimentaire et sanitaire plus obéir aux obligations en matière de logement social plus permettent le maintien des espaces publics et le développement indispensable à la qualité de vie ou encore par exemple favoriser la biodiversité au travers des trames vertes. Chacun de ces objectifs traîne son cortège de normes de contraintes toutes prioritaire, il devient impossible d'y répondent systématiquement. Face à la technicité de ses injonctions contradictoires à la multiplicité des acteurs, les élus locaux ne peuvent qu'être désemparés. Il est donc urgent de leur donner les voies et moyens qui aide à l'arbitrage au choix et simplifier leur tâche ainsi l'objectif de nos travaux et des amendements que portera le groupe Union centriste sont de permettre que la mise en oeuvre Dusan se fasse par un consensus territorial garant d'équité et d'équilibre rural urbain. Pour cela, la proposition de loi favorise, d'abord le dialogue territorial autour du zen et renforce l'association des collectivités qui décident ensemble et échange avec l'État sur les objectifs pour cela aussi la proposition de loi répartis les consommations foncière en fonction des responsabilités, responsabilités et de la réalité des besoins. Pour cela, encore, la proposition de loi prend mieux en compte les spécificités territoriales notamment les territoires ruraux ruraux se frappés par l'érosion côtière ou montagne car Lausanne ici est aussi et surtout une affaire de différenciation pour cela également la proposition de loi vise à prévoir les outils locaux à la main des collectivités pour faciliter la transition vers Lausanne, notre groupe proposera ainsi de consolider la chaîne maillé de l'de l'ingénierie territoriale sur la sobriété foncière renforçant les outils locaux d'observation de mesures de planification opérationnelle et de gestion foncière pour cela. Enfin cette PPL. Appuie sur les besoins en matière de maîtrise et de requalification des friches véritable décennies gratuite d'artificialisation dans le than mais terriblement coûteuse et complexe à utiliser. Vous l'avez compris, Monsieur le Ministre, cette proposition de loi, c'est la mise en oeuvre plus démocratique et concertée partout et par tous d'un objectif certes louable, mais qui s'impose et qui d'état de la loi oppose et divise car Lausanne ne peut, ne doit pas aggraver les fractures territoriales déjà si présent dans d'autres pays, terreau des refuser des colères. Le groupe Union centriste votre ainsi en faveur de cette proposition de loi en attendant bien sûr un second volet qui portera sur les outils fiscaux et financiers Dusan je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Marc Boyer pour le groupe Les Républicains. Seule ministre Madame et messieurs les sénateurs, chers collègues. Je tiens en 1er lieu a salué le travail remarquable de la présidente Valérie Lothar et du rapporteur Jean-Baptiste Blanc ainsi que l'écoute attentive de Monsieur le Ministre. Il me paraît important de mettre en exergue quelques chiffres, 80% des communes rurales sont à croissance démographique. 22 millions de Français, soit un habitant sur 3 vivent dans les communes rurales. De millions de néo-ruraux se sont installées dans des communes de moins de 1000 habitants. Ces 20 dernières années, les zones rurales accueille ainsi plus de 100.000 habitants par an, c'est dire l'importance que nos communes rurales de disposer de surface disponible pour accueillir ses habitants sans remettre en cause la légitimité de la loi climat et résilience son application sur le terrain, vous le savez, est très contesté notamment pour Lausanne. Ce n'est pas dans un étude chez les élus ruraux. Chers collègues ne lâchons pas le légitime combat pour nos communes. Battons-nous pour une ruralité vivante. La mise en oeuvre Dusan implique le calendrier qui doit laisser du temps à la concertation, il y a la discussion entre les différentes collectivités locales. J'ai eu le plaisir de participer aux nombreuses auditions menées par la mission than depuis septembre 2022. Qui révèle que la que la réflexion doit s'organiser dans une démarche ascendante de la commune vers le National et non l'inverse. Ce sont les besoins et la volonté des élus du terrain, des maires de la plus petite commune à la plus grande qui doivent primer et être pris en considération. Il est donc primordial d'avoir une gouvernance décentralisée pour piloter C'est la condition essentielle pour une acceptabilité Dusan à l'échelle locale pour une ruralité vivante qui tient compte des spécificités des territoires ruraux et de montagne dans la territorialisation des objectifs Dusan et qui s'assure qu'aucune commune ne sera sera sacrifiée par Lausanne surtout les communes rurales et ayant consommé peu de foncier par le passé. Chers collègues battons nous aussi pour un droit au projet au développement sortir les grands projets nationaux de l'enveloppe than est une impérieuse nécessité. Le développement des entreprises renouvelable d'aussi être comptabilisés Ozanne, nous ne pouvons pas favorisé et imposé dans la loi le développement des entreprises photovoltaïque, la géothermie, l'éolien et par ailleurs pénalisé des collectivités que leurs droits à urbaniser. Ce serait la double peine. Que l'État s'applique à lui-même ce qu'il veut imposer à nos communes. Il en est de même pour les projets d'envergure régionale et départementale. Les petites communes rurales et de montagne non pas à subir les projets de développement très consommateurs de foncier au détriment de leurs projets communaux. Il est impératif de trouver un équilibre entre la volonté de développement des territoires et la préservation des impératifs environnementaux. Les communes rurales ont aussi le droit au projet et à leur développement. Pour assurer le renouvellement de leur population. Le maintien des services publics. Si demain le maire d'une commune de 300, de 500 ou voire 2000 habitants on ne peut plus attribué de permis de construire. Alors c'est la fin de la vie de nos territoires et la fin de leur développement. Nous savons tous dans nos territoires des refus d'autorisations d'urbanisme ou de permis de construire pour discontinuité de l'habitat bâti séparation d'une parcelle par une voie communale incompatibilité avec une activité agricole et j'en passe, tous ces arguments et ces normes s'oppose aux porteurs de projets et aussi au maire, chers collègues. Battons-nous pour la liberté d'agir des maires afin de la préserver. Je défends la proposition d'assurer qu'une surface minimale de développement ne peut être inférieure à un hectare cette garantie rural est essentiel afin de donner une marge d'action aux maires quand on sait qu'une commune sur deux à moins de 500 habitants. Après la marche forcée de la loi notre les maires ruraux se sentent déshabillé de leur mission et de leur capacité d'action Lausanne ne doit pas amplifier ce découragement mais au contraire renforcer le rôle des petites communes et valoriser l'action du maire en ce sens. Le maire doit rester le seul décideur des permis de construire sur sa commune, cela paraît évident, mais cela va mieux en disant. Monsieur le Ministre, nous savons compter sur notre écoute des territoires et en conclusion Lausanne réussira et sera acceptable, si ces 3 volonté sont affichés pour une ruralité vivante pour un droit au projet pour la liberté d'agir du maire. La parole est maintenant madame Frédérique Espagnac pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente et monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Équité efficacité et apaisement. C'est par ce truc type que que l'on peut résumer l'esprit qui a guidé nos travaux jusqu'à aboutir au texte que nous y a examineront aujourd'hui. Fruit d'un travail sénatorial transpartisan que je tiens ici à saluer. Équité car la lutte contre l'artificialisation des sols. Concert le pays tout entier dans le salle la diversité de nos départements et parce que la conciliation entre la sobriété foncière et le développement territorial est un enjeu collectif. Il convient donc que l'effort à mener soit également également répartis sur l'ensemble du du territoire sans discrimination dit avantages cela signifie par exemple reconnaître les réductions déjà engagés par les collectivités lors des pré-ces enjeux objectifs ce que ce texte propose efficacité car la demande principale des élus et des collectivités dont nous sommes ici les porte-voix c'est d'être bien informé pour bien avancer les élus comprendront d'autant plus l'objectif Dusan s'ils sont réellement associés et si du temps leur est donnée pour s'approprier sa mise en place en leur permettant d'avoir des délais suffisants pour modifier les documents d'urbanisme, notamment car en l'espèce, les chiffres sont clairs, trois quarts des élus interrogé en juillet de 2022, admettait être insuffisamment informés sur Lausanne laisser un an de plus au dialogue territorial c'est l'assurance du. D'une plus juste compréhension d'une plus juste appropriation et donc d'une meilleure puis qui implication du dispositif. Et pour cela il faut des aux outils précis et maniable je citerai pêle-mêle la conférence régionale de gouvernance, le droit de, de propositions de propositions des communes et EPCI pour la mutualisation de projet. Le droit de préemption ou encore l'obtention de données fiables sur l'artificialisation je pense aussi à l'inclusion dans la liste des projets d'ampleur nationale ou européenne et d'intérêt général majeur des projets relevant d'une concession de service public de l'État notamment apaisement enfin pour que l'acceptabilité de la lutte contre l'artificialisation par exemple des acteurs locaux, soit la plus grande possible en cela la logique décentralisatrice qui traverse le texte est un marqueur important de même que la considération des spécificités des territoires. À ce titre je voudrais brièvement insister sur 3 enjeux la grande garantie rural les spécificités des zones de montagne et littoral et la situation des exploitations agricoles. Les discussions engagées depuis plusieurs mois, ont permis d'aboutir à la création d'une garantie rural offrant ainsi aux petites communes des perspectives de développement, assurer à chaque commune une surface minimale de développement communal d'un hectare est une réponse concrète aux besoins des élus d'y voir plus clair dans l'effort de réduction et de l'artificialisation cette garantie est particulière mais nécessaire pour les communes rurales qui s'appuie sur le règlement national d'urbanisme ou leur carte communale. Elle est d'une condition essentielle pour leur avenir pour y maintenir nos jeunes ou les attirer pour préserver notamment nos écoles. Ainsi privée de la garantie rural les communes or est revenu comme vous le proposez, Monsieur le Ministre reviendrait notamment à exclure 821 communes de montagne de ce dispositif c'est intenable et ce serait une répartition territoriale inéquitable

faire encore plus pour les communes de montagne en tenant compte leur Space singularité pour assurer leur développement. Outre la surface minimale de développement communal. Je pense au cas des pistes de ski notamment d'on ne les compte comme espaces artificialisés semble inadéquate. Je terminerai en évoquant la situation des exploitations agricoles nous souhaitons, d'une part que le changement de destination des bâtiments agricoles sans création de surfaces nouvelles ce ne soit pas pardon, Nous souhaitons, d'une part que le changement de destination des bâtiments agricoles sans création de surfaces nouvelles ne soit pas considéré comme une nouvelle artificialisation. L'objectif est bien de favoriser la réhabilitation du bâti existant pour répondre à des besoins de logement ou pour des nouvelles activités, dans les territoires ruraux. D'autre part, il est essentiel qu'une surface occupée par les constructions installations et aménagements nécessaires à une exploitation agricole ne soit pas comptabilisées dans la surface artificialiser. Les enjeux du changement climatique du bien-être animal de l'attractivité de la profession implique que d'une nouvelle structure puisse voir le jour sans que cette mesure ne pénalisent nos agriculteurs équité efficacité apaisement. Je souhaite que nous poursuivons nos débats dans ce sens avec cet élan au service de nos communes et de leurs élus qui attendent de nous un esprit de responsabilité. Je vous remercie. La parole est maintenant à Bruno Sido pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission spéciale. Monsieur le rapporteur. Nous partageons tous, l'objectif de sobriété foncière et de protection des sols, notamment agricoles face à l'urbanisation galopante, la perte d'espaces naturels dans lesquels s'exprime la biodiversité. C'est pourquoi le gouvernement a souhaité instaurer l'objectif du zéro artificialisation nette dans la loi climat et résilience de 2021 et pourtant voté il y a à peine plus d'un an. Nous devons déjà revenir dessus. En effet, si l'intention du gouvernement sembler louables. Il faut avoir la, la réalité en face. Aujourd'hui, cette loi est un une véritable catastrophe pour tous les départements ruraux et les communes rurales. Il est aujourd'hui nécessaire de la rendre plus équitable pour tous les territoires villes urbaines comme pour les villages. Comble cette loi climat et résilience. Les collectivités sont aujourd'hui soumises à un calendrier à des règles du jeu intenable qu'il nous faut modifier très vite depuis plusieurs mois Monsieur le Ministre, vous avez multiplié les annonces relatifs aux Anne et même admis que son cadre devait évoluer madame, la Première ministre a même demandé au préfet de lever le crayon. Vous avez dit vouloir prendre en contre nos échos du terrain et traduire avec justesse la vision du Sénat. C'est ce qu'a fait d'une façon tout à fait remarquable, la commission spéciale. Oui, monsieur le Ministre. Il y a une très forte inquiétude de la part des élus locaux et surtout une très forte attente notamment des élus ruraux envers le Sénat afin de modifier cette loi. J'espère que cette PPL pourra y répondre. Je vais m'attarder plus longuement sur le 3ème axe de cette proposition de loi sénatoriale qui vise à mieux prendre en compte les spécificités de chaque territoire. À cause de cette loi qu'il faut modifier les maires se sentent à juste titre complètement dépossédé d'un des seuls outils qui reste à leur disposition l'aménagement de leur commune. En effet il y a un véritable sentiment d'injustice à ce que cette politique Dusan s'applique à tous les territoires urbains comme ruraux de manière uniforme les élus ruraux sont tout simplement ont tout simplement peur d'être sacrifiés dans la répartition Dusan d'être encore une fois, les grands perdants en leur enlevant leur droit de construire enfin. Avec l'application stricte de cette loi, quelles seront encore les grandes les grandes perdantes, ce sont bien entendu les communes rurales. Après la fermeture des commerces du dernier service public vous enlevez aux territoires ruraux leur droit de construire et donc de voir arriver de nouvelles familles de voir s'implanter une entreprise de plus 50 pour de 0 pour beaucoup de communes, cela fait toujours 0. C'est mathématique. Cette situation va poser d'inévitables problèmes d'aménagement du territoire. Que va faire le maire d'une commune rurale devra-t-il choisir entre la construction d'une habitation ou d'une exploitation agricole. D'un côté il y a la volonté gouvernementale de favoriser les petites villes de demain et de l'autre au contraire vous freiner avec Cézanne. Le Sénat a formulé une proposition simple à l'article 7 que toutes les communes puissent disposer d'une enveloppe minimale souhaité souhaité fixer ce minimum à un hectare dans la PPL en effet sous la soirée une garantie pour les petites communes rurales. Pour ma part, je serais favorable à ce qu'on aille encore un petit peu plus loin que le rapporteur en proposant que Lausanne ne soit pas appliquée dans les territoires hyper-ruraux. Nous avons des cantons qui ont moins d'habitants que le Sahara en Haute-Marne. La liste des séries Touaregs serait fixé par décret. En effet, je serais pour davantage de différenciation cela a été dit concernant l'aménagement entre les territoires. Mais surtout, cette loi ne doit pas pénaliser nos communes rurales et hyper rural. Pourtant, avec cette question de la sobriété de l'aménagement foncier cela pouvait être l'occasion d'avoir une véritable politique, cela a été dit de d'aménagement du territoire. Et de développement durable. Il n'en est rien et je le regrette aujourd'hui. Il est urgent d'en avoir une ambitieuse pour les territoires ruraux. Je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre, vous souhaitez dire. Quelques mots. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les les sénateurs si la discussion s'arrêter là nous pourrions croire que nous sommes d'accord puisque, pour l'essentiel dans les prises de parole successives, nous sommes attachés. Convenir que nous étions d'accord sur les principes. Il va néanmoins falloir et ça va être tout l'enjeu de ce qui commence désormais qu'on vérifie dans le détail de chacune de ces mesures. Jusqu'où nous allons. Je vais pas reprendre la totalité de ce qui a été dit, mais de quelques mots bien sûr la question du social évoqué par Cécile Cukierman est crucial. Et je vais directement à Sonia de la Provoté. Dans les injonctions contradictoires, elles ne sont pas nouvelles. Quand on est maire, je l'ai été. Même quand il n'y a pas de nouveau texte vous êtes dans des injonctions contradictoires, y compris compte tenu parfois de la réaction des riverains, selon la proximité d'un équipement ou d'un service public. Et la destination ou la distance qui les sépare de leurs propres maisons de leur propre habitation et même un container enterré pour aller jeter du verre alors que nous sommes tous d'accord sur le recyclage peut faire l'objet de discussions âpres parce que tout le monde est d'accord mais pas à côté de chez soi. Et donc de ce point de vue sur la ruralité nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut apporter une garantie rural. Je souhaite quand même. Dire qu'il y a plusieurs ruralité dans ce pays. Et que nous avons un quart des communes dont la population a baissé dont l'artificialisation augmenter et à l'autre bout du spectre, on a effectivement 800 communes qui n'ont pas construit un mètre carré, en plus de 10 ans. Et plus encore si on élargit. Un territoire rural qui n'est pas celui qui a le plus contribué à consommer, pas plus que le territoire urbain. On en fait une consommation qui s'est concentrée sur le péri-urbain. Quand on regarde en terme de dynamique de population et qu'on observe les chiffres. D'où l'importance de la manière dont dont va écrire et décrire un certain nombre de choses. Je n'ai pas précisé, tous les sujets qui étaient pour nous des irritants. L'article 9 avec effectivement les pelouses qui pourrait cesser d'être artificialiser et devenir des réservoirs d'artificialisation est évidemment. Une ligne. Rouge total qui ne pourrait pas trouver un chemin d'accord avec l'Assemblée nationale, compte tenu de la manière dont ça transforme y compris le calcul de l'artificialisation partout. D'autres sujets, je pense au bâtiment agricole qui sont en zone. Ah. Les attentes de la sénatrice. Espagnac sont en quelque sorte déjà obtenu par l'actuel calcul du mode d'artificialisation et donc nous aurons sur certains de ces sujets des positions qui nous permettront d'entrer dans le détail, je vous redis que le souhait qui est le mien, c'est bien entendu qu'on puisse faire oeuvre utile une oeuvre utile, qui consiste, pas seulement avoir un document qui sortent de la chambre haute on étant le plus parlant possible pour les territoires mais en étant le plus opérationnel pour ensuite dans le cadre d'une navette changer la loi, parce que toutes les critiques qu'on a, les uns et les autres pu exprimer. Elle concerne pas un projet du gouvernement. Elle concerne un texte qui a été votée, qui à force de loi. Sur lequel vous travaillez depuis un certain nombre de mois et sur lequel il y a moins d'un an. En qualité de maire d'une ville. Je regardais comment l'appliquer sur mon territoire et en partager la contrainte dans mon intercommunalité. On aura donc des occasions de faire en sorte de prolonger ses visions dès maintenant.

Oui madame la présidente. Qui légifère mal s'expose à légiférer deux fois. On l'a entendu dans la discussion générale mais je crois. Le terrain considère que cette législation sur Lausanne et plus qu'un et plus qu'un, un irritant les procédures enchevêtrés. Les acronymes improbable la très grosse différence entre les communes les plus rurales et les autres dans un département rural comme le mien. La construction d'un d'un contournement d'une ville moyenne, va nous interdire de construire le moindre clapier pour 10 ans. Tout ça n'est pas très raisonnables. totalement irrité complètement dépourvu et aussi très mobilisés. Comment voulez-vous Monsieur le Ministre, qu'on puisse assurer le maintien d'une population en milieu rural et, et en même temps ne pas avoir de droit à construire l'hectare sur 10 ans peut être, mais en attendant il faut survivre. Donc, ce texte est est une rustine. Moi je considère que il faut faire mieux. Personne ne nie la nécessité de cette de cette maîtrise du du sol et et de la construction, c'est une évidence. Mais il y a mieux à faire avec des décrets d'application qui vont au-delà. Dalwa de la loi avec une étude d'impact qui a été complètement carencé. Je suis assez favorable à l'idée d'Alain Lambert de pouvoir attaquer les études d'impact quand elle confine au Dole parce que finalement cette étude d'impact ne ne disait rien sur le résultat exact de ce qui allait se passer sur nos territoires et notamment les plus ruraux, une disparité entre les communes plus importantes et les bourgs ruraux une impossibilité pour les communes de construire et puis surtout un texte complètement illisible, Monsieur le Ministre. Donc moi je reconnais tout à fait l'importance de ce qu'ont fait nos collègues dans la rustine que nous, nous vous proposons aujourd'hui je vous propose plus simplement d'abroger les dispositifs Dusan dans la loi climat résilience que par ailleurs, par prudence et Flers. Je n'avais pas voté.

Qu'est-ce que ça cache plus 1% en Île-de-France, moins 0,2% en Haute-Saône, dans mon département et il faudrait diviser tout ça par 2 d'ici à 2030. Depuis Paris, d'une manière totalement unilatérale. Mais je voudrais replacer ça monsieur le ministre, dans le contexte général que nous vivons. Fusion des régions fusion des intercommunalités disparition d'intercommunalité sera être prescriptif Lescott les tout puissants ABF les transferts de compétences dans tous les sens, à tous les niveaux. Nous passons notre temps à appliquer de nouveau texte qui change alors même qu'ils ne sont pas encore en application réelle. Tout ça a un coût absolument exorbitant pour nos collectivités. Alors nous prenons à chaque élection, l'engagement de simplifier la vie des Français de nos élus et à chaque mandature on en rajoute et on continue à complexifier le résultat nos élus locaux n'en peuvent plus. Nos concitoyens ne comprennent pas les refus de permis de construire ou d'autorisation suite à des demandes diverses et variées. Nos entreprises du monde rural déjà très peu nombreuses risque de nous quitter. Donc je dis pour une fois, pour une fois. Osons, mes chers collègues, osons la simplification. Je rejoins ce que vient de dire. Madame Goulet supprimons pour une fois un texte dont nous n'avons pas pas besoin et nous donnons de la liberté à nos élus locaux dans la grande responsabilité qui est la leur. Tout le monde est attaché à la qualité de notre campagne, tout le monde est attaché au monde rural. Tout le monde est attaché à l'école à l'écologie. On aime nos campagnes Monsieur le Ministre on a simplement envie de pouvoir continuer à y vivre, continuer à avoir des enfants continuer à avoir des entreprises, des emplois, laissez-nous la vie dans un peu de liberté et faites-nous confiance pour la responsabilité qui a toujours été la nôtre. D'où cet amendement de suppression. Merci Madame Goulet pour le 39. de suspendre les dispositifs de la loi climat résilience jusqu'à ce que la présente loi que nous n'allons pas manquer de de voter rentre en application et je retire le 38 mal la président. Merci qui. De David. La commission sur ces amendements. Madame la présidente, chers collègues. Alors en fait c'est le c'est cri de colère qu'on entend, pour commencer cette séance, on les a tous entendu hein c'est c'est ce qu'on a exprimé les uns et les autres, et ceux qui se sont exprimés l'ont dit à leur tour, les élus sont très en colère depuis le début. Néanmoins nulle part et prononcer le mot abrogation dans les assemblées de mer nulle part. Ce qui est demandé, c'est du temps de la liberté. Les aménagements des garde-fous de la souplesse et des moyens. Voilà, voilà ce qui est ce qui est dit partout. C'est dans ce cadre que la commission spéciale d'abord une mission conjointe de contrôle ensuite une commission spéciale intergroupe inter-commissions s'est réuni pour faire des propositions pour aller dans la trajectoire mais en changeant de méthode, voilà une méthode plus ascendante avec plus. Plus de droits pour nos élus un droit de proposition. Ça a commencé par ça et maintenant d'autres outils que nous voulons mettre à disposition des élus. Alors voilà. En fait on souhaite rester dans ce cadre là de de la Commission spéciale après vous l'avez dit vous-même hein c'est-à-dire que il y a vous croyez vous-même à la sobriété foncière. Voilà donc c'est un des objectifs qui est qui est qui est le nôtre. Ainsi qu'à Alain Joyandet, la liberté, c'est bien là qu'elle va se défendre. Effectivement, il sera question dans quelques instants de d'un schéma prescripteurs qu'elle sera dette dit diront que nous voulons d'une prise en compte. C'est au niveau on peut y avoir là de la liberté pour les élus. Donc ces quelques outils comme ça et quelques principes comme ça que nous allons défendre et c'est, c'est dans ce cadre que je ne peux que demander. Que solliciter un avis. Qu'avoir un avis défavorable, merci Monsieur le Ministre, quel est votre avis sur ces amendements. qui consiste à nous appeler à continuer à pouvoir avoir des enfants. Accueillir des entreprises, de développer nos territoires. Je veux juste remettre les choses quelques instants à leur place. Cinq terrains de football par heure. C'est ce que nous consommons dans ce pays. Et ma conviction la plus absolue, c'est que la défense de notre qualité de vie, elle passe aussi par la défense de nos paysages et de nos espaces agricoles. Il s'agit pas d'aller demander des efforts aveugle et le texte de loi actuelle ne dit pas ça. Vous avez décidé. De pas dire qu'on divisé par 2, ce qui était les trajectoires de chaque collectivité. Mais de faire confiance aux conseils régionaux. Ça c'est le texte tel qu'il est sorti de la loi climat et résilience pour justement faire en sorte qu'il y ait des élus. Dans le processus. Et pas des fonctionnaires qui à un moment. Regarde comment répartir ses territoires. Ça a été le sens de vos débats et du fait de ne pas reprendre telles quelles les propositions de la Convention citoyenne. Donc il y a plein de choses que je peux entendre ce texte est améliorable mais si on abroge ces dispositions aussi on le suspend. Ça veut dire qu'on n'écoute pas. La réalité d'une érosion de la biodiversité qui à terme. Menace aussi la qualité de vie, des espaces qu'on prétend défendre. Et donc, je veux croire que parce que vous pensez sincèrement qu'il faut permettre à nos territoires de continuer à se développer vous porter davantage ces amendements pour faire en sorte d'animer le débat au début de cette discussion que pour véritablement obtenir l'abrogation des dispositions. Et donc avis évidemment défavorable. Si je vais donc mettre aux voix d'abord les 2 amendements identiques six et 230 qui est pour. Même pardon. Oui j'ai j'avais demandé une explication de vote président juste une seconde. Monsieur le rapporteur. Je pense que si on avait interrogé les mères. Sur une possibilité d'abrogation pour réécrire une loi dans des meilleures conditions. Je suis pas certaine qu'il est, il n'est pas demandé et qu'il y ai pas pensé. On leur a pas proposé d'abroger ces dispositions qui sont totalement et puis Monsieur le Ministre, le fait que le le sera soit au niveau régional fait que vous comprenez bien que que l'Orne est défavorisé par rapport à Cherbourg au Havre quand il s'agit d'avoir des superficie constructible dont moi je maintiens. Cet amendement et et je considère que. Il vaut mieux légiférer sur un texte nouveau qui prend mieux en qui prend mieux en considération les les problèmes des territoires les plus ruraux qui garantissent l'équilibre plutôt que rustines La présidente. Madame la présidente de la commission. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre. Je crois que c'est quand même important en début de, d'examen de ce texte de relayer quand même ce que nous entendons sur le territoire parce que sans quoi on pourrait croire que tout va au mieux dans le meilleur des mondes possible ce qui n'est pas le cas il y a effectivement ça l'a déjà été dit, mais je crois que ça mérite d'être répété, beaucoup de doutes et d'inquiétudes. Sur cette vraie révolution des esprits que constitue Lausanne et nous sommes tous interrogé par les élus locaux. Beaucoup m'interroge en Saone-et-Loire. Comment la même semaine, peut-on au Sénat effectivement tenir un, un colloque sur la simplification administrative et ne pas l'appliquer toute de suite aux en en supprimant ces dispositifs cette usine à gaz qui apparaît déjà lorsque nous préparons sur le terrain, un certain nombre de pays lui. Par exemple, d'autres élus m'interpelle monsieur le ministre, en me disant, mais pourquoi ne pas faire le pari de la liberté locale et de l'esprit de responsabilité des élus territoriaux en de sobriété foncière et d'artifice il a égalisation limitée dans les textes mais sans passer par ce corset rigide susceptibles d'être impliqué avec brutalité par un certain centralisme régional qui pourrait être sous l'influence des territoires les plus riches, les plus dynamiques, les plus peuplées au détriment de ceux qui sont en déclin ou des territoires ruraux et d'ailleurs nous en parlions avec ma collègue Anne-Catherine Loisier dans notre région et bien les premières discussions. Au sein. De de la région font apparaître que les pourcentages qui sont distribués, ici ou là. naturellement on donne beaucoup plus à la métropole dijonnaise qu'aux élus. Qu'aux territoires ruraux. Ce sont donc des vraies préoccupations. Alors naturellement la grandeur du Sénat c'est toujours de pouvoir qu'on peut compromis et au-delà des messages que nous pouvons faire passer, il faut bien sûr apporter des solutions, c'est ce que. Jean-Baptiste Leblanc et la Commission recherché mais je crois qu'il était important de pouvoir grâce à ces amendements relayer ces ces inquiétudes qui sont bien réels. Monsieur bas. Merci madame la présidente, je ne voterai pas ces amendements parce qu'il y a d'autres dispositions du projet très forte et d'autres amendements qui nous permettront de défendre pleinement nos territoires ruraux puisque c'est l'objet même de cette loi en tous cas d'une grande partie de ces dispositions. Mais je voudrais dire au ministre. Qui ne doit pas pendant tout ce débat nous opposer le vote du Sénat à la loi climat et résilience, car le vote d'une loi, c'est un tout, ça n'exclut pas que nous ayons eu des désaccords profonds avec un certain nombre de ces dispositions et l'objet même de notre travail de cet après-midi c'est de corriger ces dispositions avec lesquels nous sommes en désaccord et dont le gouvernement a d'ailleurs fait un usage abusif, notamment en renforçant les pouvoirs de la région. Nous ne considérons pas que la région est une collectivité pertinentes pour régir la planification urbaine c'est une compétence que la loi de décentralisation de 1982 à donner aux communes et aux maires et nous voulons en rester au respect des libertés locales. Messieurs Joyandet. Merci madame la présidente, monsieur le ministre. Alors vous n'allez surtout pas me convaincre en me demandant de faire confiance à la région pour organiser le le le territoire de mon secteur rural, je parle de la région que je connais bien, je ne veux surtout pas parler de toutes les régions à la fois. de de de vous dire ce que je vais faire sur le ministre. Un petit département comme la Haute-Saône pas un kilomètre d'autoroute de 130.000 habitants. Plusieurs dizaines d'entreprises ultra-performante qui exportent. Notre participation à la balance commerciale est positive de 425 millions d'euros par an. C'est pas si mal pour un petit département rural qui a pas d'autoroutes. Si vous nous donnez même pas la possibilité donnée 200 m2 aux 300 m2 à ces entreprises pour se développer. Quel avenir pour un petit département comme le nôtre. Impossible.

Je vous laisse dire la suite, donc c'est pas possible, il faut vraiment mettre un coup d'arrêt à ces contraintes qui sont mises à nos territoires. Sans doute les plus dynamiques. Alors quand vous nous dites qu'il faut évidemment contraindre les grandes sur les les grands secteurs urbains. Je comprends mais la contrainte. Moi je veux de la contrainte pour personne, je ne veux opposer ni le secteur rural au secteur urbain. On a besoin de tout le monde donc sortez-nous quelque chose d'équitable dans lequel on puisse croire et qui soit applicable. Donc Monsieur le Ministre, attention par rapport à ce qu'on va faire les décrets regardez-les bien avant de les signer, parce qu'on ne trouve pas ce que nous ce que nous votons ici alors on est un certain nombre à vouloir carrément simplifier supprimé mais je veux respecter le travail qui a été fait par la commission spéciale bravo madame la présidente, et par notre rapporteur je veux respecter ce travail je veux croire une fois de plus ce qu'on va faire quelque chose qui sera équitable pour nos territoires et pour l'avenir en général de de notre pays qui a besoin d'une osmose entre la ruralité et les territoires urbains, donc je vais retirer cet amendement. D'accord merci. Monsieur saumon. Madame la présidente. Monsieur le Ministre juste pour préciser un peu ce et compléter ce qu'a dit Philippe Bas, effectivement il y a quand même une mise en concurrence dont craignent un certain nombre de communes d'intercommunalité au département. Quand vous regardez par exemple la région des Hauts-de-France. Vous savez qu'aujourd'hui sur les 400.000 hectares qui sont consommés, 100.000 hectares sont consommées pour des le foncier économique et quand on regarde quelle est la proportion à la fois de la représentation par rapport à la population et à la fois ce qui pourra être définir le sera dettes qu'il y a quoi d'avoir des inquiétudes. Pour autant, je sais que le président de la région est attentif à l'équilibre territorial mais il y a quand même de quoi se s'inquiéter et je vous rappelle pour compléter ce qu'a dit Philippe Bas, c'est que les départements, à mon sens, et selon la loi notre été en responsabilité de la solidarité sociale et de la solidarité territoriale pour pouvoir. Contrôler effectivement que chacun des territoires puissent avoir de l'attractivité avoir du développement. Je ne suis pas certain qu'avec cette délégation au conseil régional via laissera dettes garantissent au département et à toutes les intercommunalités, d'avoir le développement qu'elle souhaite. Merci. Il n'y a plus d'explications de vote. Je vais donc mettre aux voix. D'abord l'amendement 6 rectifié de Madame Goulet qui est pour deux double avis défavorable, pardon, qui est pour. Qui compte. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Et ensuite, nous avons un 39 de Madame Goulet inquiet pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Nous passons maintenant à l'article premier avec des demandes de parole.

cet amendement revient sur un, un manque évident. De la loi climat et résilience, qui est que on a un objectif à moins 50% très clair pour la prochaine décennie avec tous les débats sur sa mise en oeuvre mais. Nous aurons. Du temps pour y revenir mais après. Que se passe-t-il après. C'est-à-dire on parle d'une trajectoire qui nous amène à 0 en 2050, on est à moins 50 en 2031. Mais après il n'y a plus. Aucun chiffre donc la la proposition qui est faite là, ce qui est effectivement une trajectoire. Moins 50 en. 2031 par rapport à la période de référence, moins 75 pour 110 ans après, toujours par rapport à la période de référence, ce qui veut dire d'ailleurs que si des territoires parce que effectivement il faut de la souplesse dans la loi ne font pas, ne consomment pas les 50%. Dans les premières décennies ils pourront consommer un peu plus dans la 2ème décennie mais on ne dépensant pas les 75% à la fin de la décennie et moi à 87%, j'ai pas mis 87 et demi d'un point de vue mathématique. En 2041, je crois que c'est très important quand même que l'État nous précise comment il voit les 20 ans qui vont suivre la première décennie qui est vraiment un, un angle mort de de la loi. Autre conséquence de cet amendement. Essayé vraiment de simplifier puisque le terme est beaucoup utilisé je moi je regrette profondément qu'on ne soit pas restée sur les 30 ans uniquement sur les Hénaff. On a eu l'occasion d'en parler en commission spéciale, c'est-à-dire la tache urbaine d'un côté les espèces naturelles agricoles, forestiers, de l'autre ça aurait profondément simplifier la loi et la aurait rendu certainement plus lisible, donc cet amendement effectivement son présupposé, c'est qu'on resterait sur l'ensemble de la période sur les avec une trajectoire de baisse régulière, ça me semble un amendement quelque part de bon sens et il faudra qu'on comprenne un jour pourquoi l'État n'est pas allé sur les jusqu'en 2050. Madame la présidente, en fait. Je souhaite dire à notre collègue que cette proposition de loi recherche plutôt de la souplesse. Comprends parfaitement le le le l'urgence climatique et celle que vous ressentez à Doha cranté des trajectoires ambitieuses. il y a aucun problème là-dessus mais on vise plutôt à lever des contraintes ici que de, que d'en rajouter. À ce stade qu'on. C'est dans cette recherche de souplesse. Que nous voulons nous inscrire et puis nous voulons dire aussi que les élus sont déjà dans la sobriété foncière depuis longtemps et qu'on peut leur faire confiance pour eux mêmes s'inscrire dans dans dans la trajectoire donc en l'état, ce sera un avis de retrait ou défavorables. Monsieur le Ministre. Je vais également demandé le retrait au sénateur Dantec parce que le gouvernement aborde la période 2031 2050 avec humilité. On on est déjà pas en 2031. Je ne vois pas comment on fera l'objet à un moment ou un autre d'une clause de revoyure quand on approchera de ce moment pour regarder comment le texte que nous aurons voté aura été appliqué, donc avant de déterminer la période qui suit. Il conviendra de tirer les leçons. De là où nous en serons et. De ce que seront les besoins pour être totalement transparent. Si nous étions vote initial d'un texte que là-dessus, on pourrait faire des trajectoires mais on est en train de réviser des choses sur lesquelles on a parfois été un peu vite. Donc je me garderai d'aller rajouter des périodes de 31 2050 alors que il faut d'abord qu'on regarde comment on aboutit. Très bien monsieur Dantec. Oui j'en j'en j'entends évidemment ce qui est ce qui a été dit. Mais il y a 2 questions de posées, il y a cette question sur la trajectoire. C'est bien entendu la réponse du rapporteur du ministre et il y a l'autre question qui est. Mais pourquoi donc est-on sorti des Hénaff. Pour les 20 ans qui suivent cette question là. Qui va revenir sur l'article 9 notamment est quand même une question extrêmement importante, c'était aussi le le sens de cet amendement d'appel que je peux retirer parce que c'est vraiment pour ouvrir le le débat, donc je vais le le retirer mais il faut qu'on revienne sur cette question des sur la période 2032 1050. Merci madame la présidente. Je salue tout d'abord les les auteurs de cette proposition de loi qui apporte des réponses à des questions majeures de droit à construire de de développement économique et d'aménagement du territoire. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'objectif than mais le temps m'est compté. Alors j'aborderai rapidement de points. En 1er lieu une problématique spécifique aux milieux ruraux avec la sédentarité des populations qui caractérise nos territoires. La restriction de permis de construire est synonyme, vous le savez de fin de construction de nouveaux pavillons donc de fin d'arriver dans les villages de jeunes couples avec enfants donc de flétrissement d'effectifs scolaires dans ces communes et donc à terme de fermetures de classes et d'écoles. C'est un sujet basic. Que j'ai d'ailleurs abordé avec le recteur de l'académie d'Amiens car il me semble que cette évolution than aura un impact évident sur la démographie scolaire qui n'a pas été suffisamment étudiées. Il faut l'avoir en tête et autant que faire se peut l'anticiper le 2ème point que je souhaite aborder dans mon intervention porte sur le sujet des grands projets nationaux et même internationaux comme le canal Seine Nord. Ce projet de 116 kilomètres qui va connecter la liaison fluviale Stanesco 20.000 kilomètres de voies européenne va générer, vous le savez, des milliers d'emplois lors des travaux et des milliers d'autres à terme par le développement des plateforme multimodale. Les 1036 hectares de consommation nette de cette infrastructure ne doivent évidemment pas être inclus dans le calcul than surtout au niveau régional. L'article 4 que nous abordons dans un instant de cette proposition de loi et donc un moindre mal puisqu'il prévoit de comptabiliser séparément au sein d'une enveloppe nationale ces grands projets, il lutte était selon moi plus judicieux de les exclure complètement du calcul Lausanne nationale mais faute de grives, on mange des merles. Je compte donc sur vous, mes chers collègues. Pour que la version finale du texte ne pénalise pas les régions qui accueillent de grands projets vertueux sur le plan environnemental, comme le canal Seine Nord grande infrastructure attendue au sein du continent européen. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues de tout d'abord permettez-moi de saluer le le travail des auteurs de cette PPL. Je voudrais aussi dire qu'il était important donc de revoir ce dispositif qui est mal adapté à nos territoires ruraux, même si bien évidemment nous partageons l'objectif de réduire la consommation de l'espace dans notre pays. Nul ne. Ne conteste cet objectif mais il est nécessaire de faire une application différenciée plus territorialisée et mieux adapté aux territoires ruraux les règles. Doivent répondent donc à la diversité des territoires et des besoins afin d'assurer la revitalisation de nos territoires ruraux, on ait fait une application uniforme. De de l'objectif de réduction notamment de moins 50% à horizon 2031. À toutes les communes signifierait que près de la moitié d'entre elles disposeraient d'une enveloppe d'artifice.

celles qui ont fortement artificialiser disposerait quant à elle d'enveloppe toujours importante. Donc c'est très important effectivement ça été rappelé d'ailleurs tout à l'heure par notre collègue. Bruno Sido. les grands les les grands travaux, les grands chantiers d'intérêts nationaux dans notre département, Haute-Marne et Meuse. Le projet Cigéo de stockage de déchets nucléaires. Qui est en projet si nous comptabilisons donc à l'échelle du département, bien évidemment ça freine complètement les possibilités de, de construction et de développement et donc. L'intégration qui est fait et la mutualisation qui est faite dans ce texte de loi. Va dans le bon sens. Je voudrais enfin. Rappeler que la crise sanitaire a fait émerger de nouveaux besoins dans nos territoires ruraux, une nouvelle vision de la ruralité qu'il nous faut conforter, il faut donc donner aux territoires ruraux les capacités de répondre aux attentes de leurs habitants et nous devons hein s'inverser la spirale. Merci. Monsieur Paco. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, permettez-moi, à mon tour de saluer la qualité du travail de notre rapporteure de la présidente, mais dans la lignée de ce qu'on dit certains de mes collègues auparavant. Je voudrais vous dire que si l'enfer est pavé de bonnes intentions avec Lausanne. On a un cas d'école. D'autant plus que. Les politiques publiques. Sont pétris de la porcelaine de leurs contradictions. Ainsi, alors que l'ANRU c'est un mot qu'on n'a pas prononcé mais l'rue nous a fait déverser des milliards pour mettre des tours Rabat pour aérer des quartiers le than parle de densification et de verticalité. Alors que. On parlait jadis d'aménagement du territoire, le mot lui-même il a disparu du vocable gouvernementale et même de l'architecture ministérielle, il y a une ministre de la cohésion des territoires d'aménagement point alors veut-on faire de la ruralité. Ça a été dit, une réserve de Peaux-Rouges. Veut-on transformer nos campagnes. En conservatoire de la vie rurale en éco-musées. La version née des. Décrets gouvernementaux la version Dusan et des décrets gouvernementaux. C'est un espèce de monument technocratique. Bâtie avec des parpaings de de de malthusianisme de décroissance mais sans aucun bon sens. Alors il est grand temps effectivement de réécrire Suzanne à l'encre. De de la lucidité et de la proximité et c'est ce qui va être fait, je l'espère, on l'espère. On est tous pour la sobriété foncière mais pas pour le zéro zéro artificialisation nette ça claque comme un dictate comme une condamnation. À l'asphyxie comme une condamnation à la mort lente de nos campagnes et alors sans reprendre. Apollinaire qui voulait qu'on rallume les étoiles, moi ce que je souhaite c'est que les 30.000 petites lucioles qui illuminent. La France, hé bien elle ne s'éteignent par parce que le brasier le grand brasier des métropoles ne suffira pas pour éclairer réchauffer. Tout le pays. Madame Préville merci. Si madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Réduire l'artificialisation est une nécessité. Ces dernières années qui ont vu l'équivalent d'un département artificialiser en 10 ans n'ont pas été vertueuse pour le moins pour lutter contre le dérèglement climatique et préserver la biodiversité. Car c'est bien de cela dont il s'agit ou pas. Nous devons ralentir le rythme d'artificialisation hé bien mieux cadrer notre développement pourtant nécessaires lui aussi ne serait-ce que parce que la population française augmente. Cela étant, les décrets pris l'été dernier en application Dusan voté dans la loi climat et résilience ont non seulement été vécue comme particulièrement sévères voire brutaux mais ont eu des conséquences dans un territoire rural comme le mien, assez draconiennes pour certaines communes d'une certaine manière, la confusion règne le seul maître mot ayant été cette fameuse division par 2 d'ici 2030 sans tenir compte des spécificités des caractères particuliers. En un mot, ce qu'on appelle différenciation, même pour des situations qui pouvait paraître évidente, comme par exemple une commune ayant une école, une autre particulièrement attractive ayant un grand nombre de construction récente et donc en fort développement ou une autre ayant une entreprise avec un bel avenir, hé bien ces communes que je viens de ne ont vu leurs droits à construire drastiquement diminué cette année rien comprendre. Les élus s'il ne désespère pas se questionne sur leur rôle. Cette proposition de loi apporte des solutions concrètes que vous devez entendre Monsieur le Ministre, néanmoins il faudra reconnaître la particularité de chaque territoire sous peine de passer à côté des aspirations légitimes des élus qui sont très conscients des enjeux et qui adhère unanimement à cet objectif, on peut et doit leur faire confiance pour les rencontrer régulièrement comme nous tous ici, je peux le dire, tout le monde s'accorde à dire qu'on ne peut pas continuer ainsi, nous devons le faire avec Intelligence et avec les élus qui sont responsables. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, nous avons le souci que ce fameux Anne ne soit pas une machine à broyer la ruralité et surtout empêcher son développement. Pour ce faire, il faut se baser sur des données fiables. Lorsqu'on nous dit que un petit département est harpiste, artificialiser tous les 10 ans. Ils conviennent de se baser sur des données non contestable. Lorsque l'on regarde les chiffres de la Dreal par commune, on s'aperçoit que c'est le parcellaire cadastrales qui est retenue comme critère et non l'artificialisation réel aussi se doter d'un véritable outil de mesure pour évaluer l'artificialisation. Est il est important et même primordial pour nos territoires mais aussi et surtout pour la ruralité aujourd'hui cet outil n'existe pas. Des outils alors que nous avons des outils satellitaires pour mesurer les parcelles au niveau de la PAC au niveau agricole nous ne l'avons pas pour mesurer réellement l'artificialisation c'est quand même étrange. Je souhaite que nous nous basons sur des outils de mesure fiable et incontestable pour Lausanne. Quand nous avons pu constater après vérification Trifine nous sur le parc naturel régional des Grands Causses que souvent les évaluations faites par l'État sont très supérieurs à la réalité. Partant ainsi d'un postulat qui est complètement erronée. Madame la présidente de la commission spéciale. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Bien entendu, Monsieur le Ministre, nous partageons tous, l'objectif de sobriété. Qui était fixé dans cette loi climat et résilience, je fais partie de ceux qui ne l'ont pas voté. Parce que je subodore et un certain nombre de choses que finalement nous voyons maintenant poindre au travers de ses décrets d'application qui ont heurté, nombre d'élus. Vous savez, Monsieur le Ministre, tout ceci est très injuste pour un certain nombre de territoires. Je vous citerai 2 exemples dans mon département du ta. Après moultes et moultes tergiversations de l'État en fait, nous allons avoir la 69 l'autoroute entre Castres et Toulouse qui va voir le jour et de les travaux débutent ces jours-ci. comment expliquer aux élus de ces territoires que maintenant qu'il va y avoir cette artère qui va permettre d'irriguer ce territoire et qu'ils seront totalement bloqués par rapport à la nécessité d'accompagnement donc des perspectives de développement de ce territoire.

ils n'auront pas cette opportunité, cette possibilité de pouvoir répondre aux besoins des des populations parce qu'ils ont été particulièrement vertueux jusqu'à présent, qui n'ont pas ou peu d'artificialiser et donc dans ce cadre là cette cette loi climat et résilience est parti comme injuste parce que si vous me permettez l'expression pénalise de plus particulièrement les bons élèves parce que, comme cela a été dit par certains collègues. La moitié de 0, ça fait 0 avec tout ce que cela comporte. Donc il est important de tenir compte de ce message et de ses éléments, et je terminerai par un poème, Monsieur le Ministre, dans une petite commune. Quelques jours après ce magnifique résultat que nous avons eu à Londres une municipalité qui voudrait construire un terrain de rugby ne pourra pas le faire parce que ce sont deux l'artificialisation et donc par rapport à cela, Monsieur le Ministre, j'espère que le gouvernement ne saura écouter la voix des élus et des territoires ruraux. Et les orateurs écouter un peu la présidente aussi. Monsieur Éric Kerrouche. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, madame la présidente, monsieur le le rapporteur. La question du Dusan. Traverse l'ensemble de nos, de nos communes et d'une certaine façon. L'urbanisme est un peu devenu l'arc. Définissait Gide l'urbanisme né de contraintes vis de lutte et meurent de liberté. En l'espèce sur le sujet Dusan. Il est évident que. Cette proposition de loi amène de nombreuses, tout n'est pas résolu la question de la période de référence qui fait que certains ne vont pas être placé dans la même condition que d'autres ou celle de la différenciation des territoires qui n'ont pas les mêmes trajectoires reste toujours importante mais des améliorations, il y en a singulièrement sur cet article 1

Philippe Bas disait que la région n'avait pas de compétences particulières en matière d'urbanisme. Mais il n'en demeure pas moins que depuis la création de l'établissement public régional en 1972, elle en a une essentielle qui est celle de la planification cette planification ici un rôle important mais il fallait qu'il y a un temps suffisant qui soit consacrée au dialogue territorial. Pour élaborer un document qui est plus que complexe comme vous le savez pluriannuel et qui structure toutes les décennies à venir. C'est d'autant MU plus complexe que les règles de de comptabilisation de l'artificialisation des dans les décrets sont floues et que la publication de ces décrets a été tardive. C'est un temps nécessaire, parce que dans l'enquête que nous avons réalisé avec le groupe en novembre 2022. Moins de la moitié des élus locaux s'estimer suffisamment informés et surtout plus la strate de communes étaient basse plus cette information était considéré comme limité, nous sommes donc satisfaits de cet article, tout en restant attaché au respect des délais de consultation du public en matière de démocratie environnementale. Je vous remercie, merci. Si Monsieur Bonnecarrere. Oui madame la présidente. Monsieur le Ministre, en soutien des différentes expressions de de mes collègues et de la PPL, je voudrais avoir de niveaux d'observation au niveau local un niveau national sur le niveau local vous dire Monsieur le Ministre, que le classique aujourd'hui, c'est d'entendre nos collègues nous demander s'ils doivent renoncer à des projets là où depuis longtemps dans des problèmes de sécurité sur une départementale, le président de l'Interco nous dit mais comment je peux accepter qu'on fasse un créneau de dépassement demandé depuis toujours alors que cela va me consommer. Mon et la capacité d'artificialisation là, une aire de covoiturage ou le maire vous dit mais non, regardez ce que cela me donne. Ailleurs dans le département du Tarn. Un vélo route que l'on ne veut plus faire, ne parlons pas d'équipements de type usine, une usine pour produire de l'hydrogène Vert 15 hectares. Monsieur le Ministre, la commune ne peut pas donner, donner suite. Tout ceci à un moment. Où vous avez entendu la voix de la ruralité à travers mes collègues. Profondément dans un département comme le temps mais je crois que c'est généralisable, les collègues ont eu le sentiment qu'après des décennies de métropolisation c'était enfin le moment où il y avait un retour d'un mode de vie vers la ruralité et c'est à ce moment-là que l'on bloque les possibilités d'aménager. Outre les conséquences sur le foncier je terminerai sur le niveau national en faisant simplement 2 observations une nous vous avons entendu souvent dire mais la loi climat et résilience a été votée je nuance Monsieur le Ministre, c'était en garde l'engagement de la convention nationale à une époque où l'Assemblée nationale était dans sa splendeur en termes majoritaire et où elle disait c'est comme ça il n'y a rien à équilibrer. C'est une forme d'échec du bicamérisme et vous dire enfin que dans un pays qui a l'endettement que chacun de nous connaît le déficit que chacun de nous connaît 40 à 60 milliards d'investissements financiers sur la transition énergétique, il faut préserver les éléments de la croissance et je crois que Lausanne ne le permet pas aujourd'hui une ce. Merci madame Jacques. Madame Jacques. Bien. Monsieur Boyer. Madame Jacques, vous étiez pas inscrite. Oh bah, excusez-nous. Mais Monsieur Boyer, vous êtes bien inscrit. Vous avez demandé la parole et vous l'avez d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup, madame la présidente. je voudrais revenir. Sur le l'observation de mon collègue à la marque tout à l'heure sur la notion de l'artificialisation. Parce que faut bien qu'on parle tous de la même chose. Lorsque l'on dit qu'il y a 243.000 hectares. Artificialisés un département de perdu tous les 10 ans on se base sur quoi pour annoncer ces chiffres-là alors je vois Observatoire national d'artificialisation. Lorsque l'on considère un lotissement dans une petite commune rurale, avec une dizaine de lots de 600 m2, est-ce qu'on considère qu'il y a 6000 m2 qui ont été artificialisés. Tu. Une question. Et lorsqu'il y a un immeuble qui est construit dans une zone urbaine au urbaine sur une superficie de environ mettons 200 m2 sur cinq ou six niveaux où on va effectivement faire. On a, c'est certain. Il est certain qu'on artificialiser beaucoup moins. Alors est-ce que sur une maison construite sur un terrain de 600 m2. On considère, c'est la maison qui en surfaces artificialisées ou est-ce qu'on considère que les les espaces verts, le jardin. Le parc. Ne sont ne font pas partie de la surfaces artificialisées. Je veux dire que c'est une notion qui est importante parce qu'on a vite multiplié les surfaces artificialisées en zone rurale, par rapport aux surfaces artificialisées en zone urbaine. Alors si on les considère effectivement la surface totale d'un lotissement surfaces artificialisées. Il est certain qu'on va réduire très sérieusement les surfaces qui vont rester à urbaniser dans les 10 ans dans les 10 ans qui viennent et et plus tard jusqu'en 2050. Mais ça veut dire surtout que on va vers la disparition de la maison individuelle dans nos territoires. Or aujourd'hui c'est le mode de vie auquel aspirent nos concitoyens. Alors est-ce que demain on veut construire des petits immeubles dans nos petits dans nos petites communes, un petit immeuble dans une commune de 300 habitants avec un habitat ancien qui a bien été préservé, mais si on veut développer l'habitat et ben effectivement il faudra faire un petit immeuble sur 4 5 niveaux mais je ne crois pas que ce soit très positif. merci merci madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues, je voulais prendre la parole quelques instants au début de, de cet article 1er. Nous aurons l'occasion de de de rentrer dans le détail du texte et sur un certain nombre de mesures techniques, peut être pour revenir sur sur deux ou trois grandes grandes orientations. Il est clair que ce sujet-là suscite beaucoup d'attentes. Parce que c'est le 1er sujet d'inquiétude de nos élus, Monsieur le Ministre d'avoir pris conscience de cela. Depuis son arrivée au ministère d'avoir intégré un certain nombre d'attentes et et et je me réjouis que notre commission et que le Sénat et puis porter. Donc cette PPL avec la procédure accélérée, que vous nous proposez aujourd'hui. Et je voulais attirer votre attention sur 2 sujets en fait un sujet qui est. Celui de l'espérance. Il faut laisser à nos territoires de l'espérance. Il faut que chacun pense qu'il a encore le droit de se développer. Qu'il a la possibilité de se développer. Et il faut lui conférer des droits même si demain ils ne les utilisent pas tous. D'où l'importance de la gouvernance que nous mettrons en place pour justement organiser mutualisés ensuite les possibilités que chacun aura de développer son territoire et le 2ème, c'est du bon sens ça a déjà été évoquée dans le début de ce débat et ça ne manquera pas de revenir tout au long de ce débat, j'imagine. Entre les définitions les nomenclatures les références. Ce que j'appelle aussi moi les double peine pour des territoires comme les nôtres, les territoires ruraux qui ont déjà effectivement peu construit et qui demain seront encore davantage. Privé de construction. et où un certain nombre de, de, de sujet viennent viennent ici ce ce ce ce percuter quand on parle par exemple des projets nationaux, moi j'entends et je trouve parfaitement légitime que ceux qui ont la chance d'avoir des projets d'intérêts nationaux ne soient pas complètement impec impacté mais comment accepter qui ruisselle re-sur les autres qui n'ont pas la chance d'avoir ces projets nationaux. Voilà donc je voulais juste attirer votre attention sur ces 2 points qui me semblent présidé devoir présider à nos débats garder à chacun de l'espérance et agir avec bon sens. Merci. Merci madame madame Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à mon tour de saluer le travail mené par nos collègues Valérie Létard et Jean Mathis. Pour que cette proposition de loi transpartisane puisse voir le jour. On le voit bien dans nos débats, ce texte est nécessaire car il est indispensable d'entendre ce que les maires et les élus locaux nous disent face Ozanne, il est indispensable d'entendre les inquiétudes et les légitimes interrogations et les incompréhensions également que peut soulever l'application du zen, alors bien évidemment face au réchauffement climatique. Nous devons agir, préserver la biodiversité ne pas artificialiser à outrance et cette réalité est déjà. D'ailleurs celle de très nombreux maires qui n'ont pas attendu la loi climat pour faire des efforts de sobriété foncière et qui ont placé l'environnement au coeur de la de la réaction. Et il ne faudrait pas demain que Lausanne devienne l'acronyme qui mettent à mal le développement de nos communes et les enjeux si importants de la ruralité ou encore le besoin de réindustrialisation dans notre pays et des questions très concrètes se posent et on le voit bien dans les différents échanges peut avoir avec les maires. Comment les maires pourront demain répondre à la volonté des jeunes générations de rester et de s'installer dans les communes. Comment répondre-t-il au besoin de construction des services de proximité, on le voit bien avec la question du périscolaire mais également comment pourront-ils répondre au souhait d'installation des entreprises, alors je crois que ce ce texte. Vise justement à chercher ce point d'équilibre qui est oh combien. N'est-ce nécessaire, on le voit bien de souplesse de pragmatisme mais également de bon sens et je salue les outils très concrets qui le met en place. D'une part le sursis à statuer encore le droit préemptions et ça a été dit la garantie rural avec le un hectare qui est finalement un outil simple clair pour permettre aux petites communes de continuer à se développer. Attention hein. Un point et on l'a vu hein lors des auditions de la commission spéciale, celle de l'interprétation également des différentes dispositions et des recours qui risquent de se multiplier et d'empêcher, finalement, des projets importants pour les communes de se réaliser. Merci la parole est maintenant monsieur Joly. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il était en effet j'avais dit avant moi important de revoir les modalités d'application de l'objectif légitime du zéro artificiel sinon L'adaptation apparaissait cependant nécessaires pour les espaces ruraux dans lesquels les élus sont inquiets sur les possibilités de construire un avenir pour les territoires dont ils ont la charge. le comté le le contexte dans lequel nous étudions ce c'est cette proposition de loi et cette perspective du zéro artificialisation nette. Rappeler ce contexte qui est celui qui s'inscrit dans une des décennies du tout métropolitain et sur sûrement du trop métropolitain. Un contexte qui est celui de l'élaboration des Sraddet des Scott D. P. lui autant de documents normatif ou les petites communes des territoires ruraux peinent à se retrouver. Contexte également qui est celui de l'application au cours de ces dernières années une application stricte du règlement national d'urbanisme rendant juridiquement impossible toute construction sollicité. Après également le rétrécissement de la place de l'État et des services publics. Tout ceci donnant un sentiment qu'il n'y a pas ou qu'il ne peut y avoir d'avenir pour les territoires ruraux. Or, et ça a été dit, des besoins de construction existent pour accueillir les populations nouvelles qui ont décidé de choisir la campagne pour vivre la vie qu'il souhaite. Et d'ailleurs on sait qu'il y a là aussi une attente de territoires ruraux et d'envie de territoires ruraux mais également pour construire pour les autochtones qui aujourd'hui bah sont soumis également à l'assèchement du marché immobilier les les urbains venus les rejoindre. Il était donc important d'ajuster les modalités d'application de cet objectif. Je redis légitime du zéro artificialisation nette à la diversité, l'adapter à la diversité territoires. C'est le sens de la PPL que nous examinons qui pourra être enrichie par les amendements qui ont été déposés. Je vous remercie. Et surtout d'avoir été capable de placer le curseur. Qui ne posent pas mais qui entraîne le curseur qui respecte dans les territoires parce que le défi, il est grand. Il est grand dans ce sens. Où aujourd'hui on n'a voté beaucoup de textes. Mais Monsieur le Ministre. Il faut trouver de la cohérence dans tout cela, on a voté des textes sur l'obligation pour des propriétaires d'avoir des logements. Qui soient en conformité en termes d'isolation. S'ils veulent les louer. Mais est-ce que les familles auront les capacités de pouvoir faire cette rénovation. Donc. Autant de sujets. Dans la vie il y a naissance et il y a disparition. Et dans un territoire, quel qu'ils soient petits comme grands, il faut effectivement permettre la naissance donc des constructions neuves. Mais il faut aussi gérer les disparitions. Et ça veut dire Monsieur le Ministre, ça nous entraîne obligatoirement vers des réformes fiscales. Sujet qui n'a pas encore trop été abordée mais qui va être la conséquence. Comment allons-nous traiter les friches des friches industrielles, les friches agricoles les friches urbaines. Mais surtout, Monsieur le Ministre on a un vaste plan industriel en France de reconquête dans nos territoires de réindustrialisation de repositionner dans nos territoires, l'activité économique là aussi ça nous oblige. Parce que vous ne trouverez pas des entreprises locales ou extérieur venir s'implanter dans un territoire qui n'offrent plus de perspectives. Je voudrais terminer mon propos en disant sous simplement. Le travail qui a été fait. N'est pas un travail qui. Comme on aurait pu. Imaginer qui exclut mais au contraire qui peut nous rassembler et qui doit nous permettre de nous retrouver et qui doit donner l'espoir à l'ensemble des territoires. Merci à eux.

Sur la nécessité, aux termes du texte que nous examinons la nécessité d'une cohérence entre les objectifs qui sont fixés finalement par le gouvernement sur un ensemble de domaine il y a un objectif de sobriété foncière que nous partageons. Il y a aussi un objectif je voudrais précisément attirer l'attention sur 2 sujets particuliers, il y a un objectif d'adaptation et de transformation de notre modèle agricole. Pour l'adapter au réchauffement climatique. Pour les mises aux normes des bâtiments agricoles pour le bien-être animal, objectif fixé par le gouvernement pour la souveraineté alimentaire pour développer des circuits courts, pour transformer nos produits mais quand on transforme une production laitière, par exemple, pour développer des circuits courts et de la vente directe. Il faut construire une laiterie parfois une cave d'affinage, donc tous ces objectifs qui sont fixés à notre modèle agricole pour les années à venir qui sont importants pour la souveraineté alimentaire pour l'indépendance de la France dans le domaine alimentaire nécessite un moment des extensions ou des créations de bâtiments agricoles et donc évidemment il faut tenir compte de cet objectif-là que nous partageons tous, je le sais dans le cadre de, du projet de sobriété foncière 2ème objectif. Je sais que le gouvernement. Vos ministères et d'autres ministères travaillent ardemment sur. Le renforcement de l'attractivité des territoires ruraux sur qui pourrait donner lieu, peut-être un, un, un projet de loi. Mais pour renforcer l'attractivité des territoires ruraux, il y a des territoires ruraux qui ont besoin d'accueillir des entreprises d'accueillir de nouveaux habitants. Et et donc l'idée du un hectare par commune. Je sais que vous allez me dire mais que vous êtes d'accord avec cet objectif. Sauf qu'à un moment il faut que ça se concrétise sur le terrain et l'idée de un hectare par commune. Ce n'est pas quelque chose d'aberrant. Nous avons affaire à des petites communes rurales est souvent. Dispose de milliers d'hectares naturel travaille pour. Pour préserver la biodiversité pour capter le caveau carbone à travers des forêts à travers des espaces Natura 2000, vous le savez, puisqu'on a travaillé ensemble sur ces sujets. Dire que ces communes-là les sécuriser en leur disant que si elles ont une opportunité pour accueillir un artisan ou pour accueillir un couple de jeunes qui peut s'installer. Une sécurité avec un hectare. C'est tout à fait essentiel. Voilà donc je voulais changer vraiment qu'on veille à la cohérence des objectifs fixés par le gouvernement. monsieur Rambo. Merci madame la présidente, effectivement de mots aussi pour aborder un sujet qui n'est pas présent dans cette. Proposition de loi qui est le volet financier, même si notre collègue Daniel Gremillet vient de vient de l'esquisser mais je crois qu'il faudra qu'on soit une fois la séquence terminée qu'on soit capable d'adapter effectivement une fiscalité cohérente avec l'objectif alors le collègue, membre de la commission des finances. Jean-Baptiste Leblanc. Il y a il y a quelques temps, a fait un rapport à sujet il va falloir que maintenant qu'on qu'on se mette autour de la table hein il va, il va falloir qu'on peut, on soit capable d'aligner nos régimes de fiscalité locale avec l'objectif de sobriété foncier. Ça veut dire qu'il faudrait être capable ben de supprimer les règles fiscales manifestement contraire à l'objectif. Ça veut dire qu'il faudrait être capable aussi d'adopter une une fiscalité incitative à la préservation, voire à la reconquête des espaces agricoles naturels et forestiers et ça veut dire aussi qu'il faudra qu'on soit capable d'adopter une fiscalité qui encourage le renouvelle urbain et et la densité. C'est à mon avis quand même. Le prochain chantier que l'on a, si on veut arriver à cet objectif du merci. Merci la parole est maintenant Monsieur Dantec.

la droite sénatoriale des fonds c'est. Ils sont avec justesse la production agricole. La l'Ouazzane elle défend la production agricole c'est-à-dire les Terres qu'on consomme aujourd'hui avec l'étalement urbain, c'est les meilleures Terres maraîchères de Loire-Atlantique c'est les Terres du du Bassin parisien la l'Oisans, c'est ce qui va permettre justement de maintenir la production agricole en France et pas que de la production extensive. Les bâtiments agricoles dans les 10 prochaines années ne sont jamais considéré en artificialisation ça reste de L'Hénaff, par exemple, et ça je crois que c'est c'est quelque chose qui est assez mal compris. Un des premiers objectifs de la loi, c'est de maintenir la capacité de production agricole de la France. Ça je crois que sur les bancs de la droite, c'est quelque chose qui vous parle le 2ème point. Quand on dit laissons laissons de la liberté aux territoires aux communes. Eh ben si on laisse cette liberté sans encadré. Je peux vous dire où est-ce qu'on va développer des projets urbains, on va avoir une grande conurbation Nandrin parce qu'là le dynamisme. Il est à fond, ça va pas aider l'Est de la France. Pas du tout, ça va si on laisse toute seule liberté aux territoires. On va continuer à aggraver en fait la, la différence de développement entre l'Ouest et l'Est qui aujourd'hui est parfaitement. Documentée au contraire et c'est probablement un des points qui manquent dans le débat et qui a manqué, probablement dans la manière dont, dont l'État a présenté ses lois hein c'est que ça doit être une loi d'aménagement du territoire qu'il doit y avoir une prime peut être encore plus forte que ce qu'on a écrit parce que ça c'est un point d'accord avec le rapporteur, et la présidente peut-être être encore plus précis sur le fait que les territoires qui ont peu urbanisée ont encore plus de droits. Parce que ça rééquilibrera le territoire, il faut parler d'aménagement du terrain. Merci la parole est maintenant monsieur Oui. Ben présidente pour faire écho à ce que dit notre collègue. Dantec. Si on veut que ce soit une politique d'aménagement du territoire. Faut-il encore que cette politique associent fortement les élus et singulièrement les élus de notre territoire et je pense tout particulièrement aux mères. Tout à l'heure notre collègue Sautarel a parlé du bon sens. Je crois qu'il a éminemment raison si on veut. Que les aménagements je veux à mon tour saluer parce que finalement c'est le point plus positif du travail qui a été réalisé à la fois le rapporteur et la présidente c'est qu'ils ont. Fait en sorte qu'il y a une collégialité dans leurs travaux mais qu'ils ont surtout éclairer leurs travaux avec cette notion de bon sens, je crois, mes chers collègues, que le temps est venu de faire en sorte que la politique que nos débats puisse être compris à l'échelle des territoires et la vertu de ce texte. On a évoqué la question de la garantie. C'est justement de pouvoir être compris et de relever d'une certaine justice à l'échelle des territoires, je crois qu'il faudra être vigilant. Monsieur le Ministre, à ne pas perdre au fil de nos débats et dans les échanges et les négociations dans ce qui pourra Net finalement de ces travaux. Cette notion de de bon sens parce qu'elle est attendue par les maires et les élus de nos territoires. Le second point. Et là je mets la solennité dans dans mon propos. C'est que. Pour avoir été, avec Françoise Gatel, rapporteur de la loi 3DS et avoir vu la parution des décrets. Je crois que si on continue à fonctionner comme ça. Alors ça ne marchera pas. Je crois que si nos travaux ne sont pas fidèlement repris dans les décrets qui paraîtront alors je le dis, nous allons pouvoir nous économiser beaucoup de temps de travail. Je le dis avant même que le les débats avec nos échanges aient eu lieu parce que sinon on réduit à néant le travail parlementaire et la nécessaire compréhension qu'appellent de leurs voeux les les les élus des territoires et qui doit se retrouver dans la nature des travaux que nous menons. Donc je crois qu'il faudrait être vraiment vigilant à cet aspect-là de nos travaux pour que ceux qui demain. Jair Merah. Soit le plus fidèle à ce que nous aurons évoqué ici. Oui madame la présidente. Monsieur le rapporteur. Mais chez mes chers collègues. Je voulais juste faire une remarque préalable aussi à ce stade. Monsieur le Ministre. Pour revenir sur la notion de consentement que vous avez évoqué tout à l'heure et je reprendrais un peu les, les propos de mon collègue Fabien Genêt et Philippe Bas tout à l'heure. Nous avons débattu ici de la loi climat et résilience nous avons contribué j'ai participé longuement à ces débats. Dans un objectif d'améliorer un texte qui n'était pas le nôtre. un certain nombre de mes collègues ont voté ce texte parce qu'il considérait que la version modifiée par le Sénat était meilleur avait été améliorée par rapport à celle qui nous avait été présentée initialement c'est là l'objectif

Quel est l'objectif de de cette de cette PPL encore une fois, améliorer ce texte, améliorer les dispositifs de de la loi than parce que nous sommes arrivés à une situation dans le texte actuel qui ne permettait pas la moindre le le le le la réalisation des objectifs parce qu'il était devenu trop technocratique et pas assez appuyée sur la différenciation des territoires, nous allons travailler sur ce texte et je salue la le travail qui a été fait par la Commission et par notre rapporteur et sa présidente dans cet esprit-là, cela ne vaut pas consentement à ses objectifs. Je voudrais être clair là-dessus je je ne partage pas la philosophie même déclinistes de ce texte, il y a d'autres moins bien sûr que nous avons des défis devant nous un défi économique, la balance commerciale française et et dans une situation catastrophique, nous avons un défi démocratique. Les habitants ne ne se reconnaissent plus dans dans le pouvoir de cap de la capacité d'agir de nos élus et nous le renforcerons pas et nous avons un un enjeu écologique et cette loi ne réglera pas ces enjeux cet enjeu écologique de cette manière-là. Nous avons aussi un enjeu d'aménagement du territoire. Nous allons-y travailler nous améliorerons ce texte au ministère je l'espère je viens ça ne vaut pas consentement. Fabien Genêt. C'est à vous. Merci madame la présidente, puisque mon collègue Cédric Vial n'a pas pu terminer sa phrase sur l'aménagement du territoire je vais la compléter. Puisque nous travaillons ensemble sur ces sujets, je crois que nous nous sommes très nombreux à parler d'aménagement du territoire, mais aujourd'hui Monsieur le Ministre, peut-être qu'il faudrait passer des mots à l'action et pour nous, la politique d'aménagement du territoire ça ne consiste pas simplement à accompagner les grands mouvements les grandes tendances de ces dernières décennies. Ces tendances de métropolisation de déménagement du territoire rural et effectivement aujourd'hui en en Saone-et-Loire on en a parlé dans cet hémicycle il y a malheureusement quelques jours l'exemple donné par la fermeture de la maternité d'hein malheureusement nous montre combien sur un certain nombre de territoires en déclin. Eh bien. Le déménagement suit le déménagement et provoque celui-ci et, et je crois puisque monsieur le ministre, il faut aussi que vous repartiez de cette assemblée en en ayant le sentiment que nous sommes capables de vous proposer des solutions. Une des solutions, justement c'est de pouvoir réinvestir c'était à victoire en déclin puisque dans une commune comme autant par exemple qui est passé de 20.000 à 13.000 habitants en quelques décennies, hé bien vous avez un certain nombre de logements vacants qui peuvent être reconquis et pour cela, effectivement il faut une vraie volonté. C'est pourquoi d'ailleurs j'avais proposé un amendement qui souhaitait mettre dans le sera d'être un certain nombre de choses sur la politique de réindustrialisation malheureusement le couperet de l'article 45 de et sa lecture faite par la commission spéciale. Nous prive de ce débat et cela m'inquiète un peu parce que parler, parler de cette lutte contre. les problèmes d'artificialisation sans parler de ce que l'on peut mettre dans le train d'être ça me semble un peu équivoque. Mais je crois qu'effectivement sur ces politiques de réindustrialisation, cette volonté de remettre du développement économique dans ces territoires en déclin, ce sera un bon moyen. Hé bien d'utiliser toutes les aménité qui les composent et d'utiliser ce qui a déjà été finalement artificialiser par le passé pour ne pas le faire à nouveau dans le futur. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre. Chers collègues, quelques remarques là. La première c'est que nous sortons d'une période où n'existe pas. et qui pourtant a vu la dévitalisation rural et l'hyper métropolisation qui n'a pas empêché l'étalement urbain donc Lausanne n'est pas la cause de ces difficultés. Comme il n'est pas la cause non plus. De la naissance de ses tâches commerciales au péri. écoutons-nous, chers collègues, on est au Sénat. Donc comme il n'est pas. Comme la confiance au maire n'a pas empêché qu'il y a d'immenses tâches commerciales qui. Se qui naissent ici ou là et qui participe. Non pas au développement économique de notre pays, mais plutôt à sa défiguration. Donc je voulais d'abord signalé ça ma 2ème remarque c'est pour dire effectivement je pense qu'il manque un propos. Descriptif sur la volonté d'aménagement du territoire et notamment sur le rééquilibrage entre mairie entre métropoles et territoires ruraux et ce manque coûte ensuite lorsqu'on rentre dans les débats sur Lausanne et j'entends les demandes de, de respect d'espoir qui sont donnés et je pense qu'il faut d'ailleurs trouver des réponses. À à cette demande. 3ème remarque il manque le volet financier. Je me permets de le dire parce que, élu de la métropole du Grand Paris. Je me rappelle avoir fait le tour de toutes les villes lorsque nous étions dans les débats préparant la création de la métropole et tous les maires nous présentait parfois une usine un une un petit siège social de telle ou telle entreprise comme son principal atout, y compris des villes qui avaient sur leur territoire des bois des forêts ou des Terres agricoles qui pourtant étaient des atouts bien plus important que une usine de 50 salariés. Pour l'équilibre de cette métropole mais personne ne rémunère ni les Terres agricoles, ni les espaces forestiers qui pourtant sont essentiels à notre survie c'est de survie, y compris de l'humanité qu'on parle avec ça donc il faudra un jour regarder ce volet financier. Hé bien c'est vrai que ça a été dit et ça a été dit de manière quasi unanime. Lausanne z'ero articulation nette à 2050 c'est partagé par tous, tout le monde le souhaite. Tout le monde le veut, parce que c'est une nécessité absolue pour la question agricole pour les enjeux de souveraineté alimentaire et et on le voit bien pour les questions de biodiversité. Mais en tout cas sur la question agricole, on sait que c'est t'une évidence et qu'il faut y aller. Donc moi je voudrais déjà salué cet objectif effectivement de la Convention citoyenne parce que je crois que c'est le seul objectif qui a été retenu de cette manière-là et qu'on retrouve dans un, Et puis pour une fois. D'avoir une politique sur le temps long. Parce que c'est vrai que c'est assez rare qu'on ait des objectifs 2050, des orientations. Alors oui c'est pas évident. Oui c'est pas facile. Mais ça veut dire qu'il faut se donner les moyens de comment on va tenir ses objectifs. À moyen. À court terme, à moyen terme et puis jusqu'à 2050. Donc oui c'est pas évident mais en tout cas moi je voudrais déjà quand même saluer que pour une fois on a cette orientation et on a ce temps long ensuite. Abordé la question de l'urbanisme, du projet de territoire parce que oui ça va être compliqué, ça va être difficile à mettre en place et que si on travaille pas sur l'urbanisme, sur la question de l'aménagement du du territoire mais au plus près justement du territoire. On n'y arrivera pas, on ne fera pas que par bon sens parce que là, le problème du bon sens et que il est dans les, dans tous les sens et et que ça ne, ne règle en général jamais rien et puis ensuite à un constat, ça a été rappelé par mon collègue. La question de la désertification. On n'a pas attendu l'âne pour avoir ses problèmes de désertification dans les territoires ruraux et ça diffère question elle est liée. Au problème de de service public, au manque d'anticipation aux problèmes de transport. Problème à à l'ensemble de, de ces problèmes-là, donc c'est évidemment de ce côté-là qu'il faut qu'il faut travailler et sur les plus petites communes, moi j'ai un exemple sur une intercommunalité de de 10.000 habitants, les communes qui ont mis en place un PLU très exigeant. Ce sont les communes qui ont gagné le plus d'habitants dans les 10 dernières années Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. J'entends depuis un moment, invoquer en permanence le bon sens. C'est quoi ce bon sens. Est-ce que c'est le bon sens. Voilà près de chez nous, le bon sens qui regarde toujours devant sa porte mais qui oublie la globalité le bon sens. Est-ce que c'est celui qui nous a amenés où nous sommes aujourd'hui devant ce mur du réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité. Je pense que voilà il y a pas de bon sens, sans vision globale et on ne peut pas inventer invoquer comme ça le bon sens, sans savoir ce qu'il y a derrière. J'entends parler aussi de les bons élèves. C'est qui ces bons élèves. Est-ce que ce sont dans des communes rurales. Des maires qui n'ont pas artificialiser parce qu'il ne voulait pas artificialiser ou simplement des maires qui n'ont pas artificialiser parce qu'il n'en avait pas les moyens ou parce qu'il y avait pas de besoin. Il y a la notion de bonne élève aussi à à réinterroger et puis. Toujours cette opposition je pense complètement stérile entre la ruralité d'urbanité. Je pense qu'il y a de la ville que par qu'il y a de la campagne de la campagne que parce qu'il y a de la ville. Rappelons-nous que chaque Français à peu près 3000 m2, 3000 3000 m2 de surface agricole utile. Donc si on devait refaire du pavillonnaire partout, je peux vous dire qu'il resterait plus du tout de monde agricole, donc il faut regarder tout ça Vision idéale idéalisée de la campagne La Petite Maison dans La Prairie mais regardons nos bourgs anciens les bourgs anciens avait une très forte densité. C'était pas du collectif mais c'était des maisons de la vraie maison de ville même dans des bourgs anciens et donc à un moment dans les années 70, et bien on a pensé qu'il en fallait pour être heureux, il fallait grignoter, il fallait avoir une maison avec 3000 m2 je pense qu'on en est plus là, il faut regarder où on est et si on suit cette trajectoire tendancielle, hé bien on sait que l'on va dans le mur donc Lausanne effectivement il va falloir y travailler et on est là pour essayer de l'améliorer. Merci. Merci la parole est maintenant à Cécile Cukierman. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, si vous me permettez une toute petite pointe d'ironie. Je n'avais pas compris que l'objectif cet après-midi était de battre le record, les records de prise de parole sur articles qui ont eu lieu la semaine dernière mais c'est pas grave. Je vois qu'en tout cas Lausanne passionne tout autant que d'autres textes tant mieux peut-être d'ailleurs parce que nous avons un objectif partagé qui est donc. De limiter le plus possible les fractures qu'elles soient sociales ou territoriales. Je crois en tout cas que le nombre d'interventions sur ces prochains article 1er, Monsieur le Ministre. Est évocateur, s'il en était besoin. D'abord. De l'inquiétude que suscite la mise en place parce que mal pensées parce que mal mise en oeuvre parce que des décrets. Qui ont été bien plus loin que ce qu'ont voulu les législateurs. Existe. Et puis parce que, à travers les interventions. On voit finalement quoi telle que Lausanne a été pensé au départ il ne permet pas de réfléchir globalement la l'aménagement du territoire, mais ils nous opposent. Moi je suis désolé, mes chers collègues. Mais j'ai tout, on vit dans un département donné, de préserver l'agriculture et l'industrie et de permettre d'avoir des logements de qualité. Et je pense que pour bien vivre pour bien vivre individuellement pour bien vivre collectivement c'est pas l'un ou l'autre c'est pas l'un mieux que l'autre c'est un nom semble et donc je crois que c'est en tout cas ça qui doit nous guider. C'est pour ça que nous voterons l'article 1er avec les assouplissements telle que prévue par la commission spéciale et puis ensuite pour terminer j'entends tout ce qu'on se dit, la France est un pays merveilleux, en 2050, on est sur des projections de 10 milliards d'habitants sur la planète. Donc je crois qu'effectivement Monsieur le Ministre, vous l'avez dit, oui, on aura des clauses de revoyure parce que son nom ta sera les gens et les guerres et les famines dans certaines parties du monde, soit on aura des choses à revoir globalement à l'échelle mondiale. Merci la parole est maintenant hein. Jean-Marie Mizzon. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais revenir un instant. Non pas sur la sobriété verbale. Mais sur la sobriété foncière. Après tout, c'est quand même le sujet du jour. Et quand on s'intéresse à cette question en mesure que. Les chiffres qui paraissent dans différents ouvrages diffère beaucoup. Et celui que j'ai vu le plus souvent, mais est-il le bon. C'est que la France serait d'urbaniser. À 8%. Et sur ces 8%. J'arrondis. La moitié serait des surfaces à perméabilité des infrastructures des maisons des industries, des parkings et Et l'autre moitié des potagers, des jardins, des terrains de foot, des terrains de golf. Mais c'est 8%. Et donc les 92 autres %. Ce sont pour moitié aussi je schématise, des. Espaces forestiers. Et des espaces. Naturels et espace pour l'autre moitié agricole. D'ailleurs ce chiffre sont corroborés par la densité de la France. La France est un pays qui a 104 habitants au kilomètre carré. L'Allemagne c'est plus du double l'Angleterre également. Les pays les la Belgique c'est quatre fois plus. Les Pays-Bas, c'est 5 fois plus. Il y a presque une urgence là-bas. Mais ici à 8%. pardon sur la sobriété foncière comme si ça 2 devenait une religion. Ce fait sévère. Allons-y. Moi je suis aussi pour la sobriété foncière mais je suis aussi pour la clairvoyance. Et voyez-vous, Monsieur le Ministre mais c'est pas de vous ça. C'est votre président de la République qui. Dans la culture du en même temps qu'il anime à chaque instant de chaque jour, comme dirait. Dalida.

La parole est à Serge mais Riou. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre. D'abord je je remercie. Les rapporteurs pour la qualité du travail sur un sujet qui est pas simple mais qui est extrêmement important pour notre territoire à titre personnel, j'ai pas voté la loi climat et résilience, mais je partage l'absolu des cécité d'avoir une vision globale sur la consommation de nos espaces fonciers, on pourra pas continuer à consommer 30.000 hectares par Parce que sinon niveau de l'agriculture, de l'alimentation de la biodiversité, on ira très vite dans le mur. Mais ça se fait quand même à un rythme très inégale dans les territoires et à ce sujet, la mutualisation des grands projets qui paraît quelque chose d'évident n'est pas aussi simple. Les grands projets se font essentiellement dans les zones urbaines et ce sont des territoires ruraux qui vont en prendre une part à leur compte. C'est donc pas sur l'objectif de la loi que je voulais. Je vous dont je voulais parler c'est c'est sur l'opacité dans la mise en oeuvre. La difficulté dans la mise en oeuvre. J'ai, j'ai rarement vu une loi qui pouvait être aussi technocratique. On a l'impression si vous voulez que les lieux décisions sont très éloignées d'estrade. Scott. C'est une loi qui dépossède des élus locaux, les maires de leur pouvoir de décision souvent au profit des bureaux d'études qui devrait éclairer les décisions et non pas se substituer aux décisions de des maires c'est donc. Une loi qui est vécue comme une application au niveau des décrets extrêmement opaque difficile et mal acceptée dans les territoires ruraux pour lesquels c'est plus la fermeture des espaces qui nous guette, c'est plus la déprise agricole et la friche que la bête que la bétonisation. Merci la parole est maintenant à Jean-Baptiste Lemoyne. Merci beaucoup madame la présidente. Donc nous sommes sur cet article 1 qui vise à décaler d'un an, la production des documents. Et régionaux et des Scott et des lui et je pense que ça ne pose aucun problème. D'une part parce que d'ailleurs ça a été dit dans dans le rapport 50%. Des Scott prévoit d'ores et déjà une réduction significative d'ailleurs supérieure à 50% à échéance 2040 et donc je pense qu'il y a pas de crainte à avoir. Quant à l'adoption de cet article et et de ses effets par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé et puis. Les propos du collègue Cédric Vial. Me faisait rappeler un petit peu ce qui s'était passé aussi il y a quelques années dans cet hémicycle sur la loi notre. Finalement le Sénat l'a voté. De crainte. Que la copie soit pire s'ils ne la votaient pas. Et la loi notre quelques années après, on en voit le résultat. Ce sont des régions XXL. Ce sont des EPCI XXL et moi je vous le dis, si c'était à refaire, hé ben je le referais pas. Et je pense qu'on est nombreux. Dans le Sénat ici au Sénat. À avoir aujourd'hui cette position et donc tout ça pour dire que sur l'objectif qui nous réunit aujourd'hui, aujourd'hui, hé bien il faut entendre la voix du Sénat parce que c'est la voix je crois de la sagesse de l'équilibre et d'ailleurs le travail transpartisan en attestent. L'épisode des décrets a laissé quelques traces et le ministre a a dit son souhait de les réécrire, il pourra peut-être nous dire justement où il en est dans ce travail. Et puis il faut le dire aussi parfois la façon de faire de certaines régions n'a pas facilité les choses, moi je le vois. La commune d'Auxerre. Je peux vous dire, à se retrouve pas du tout dans les documents qui ont été élaborés à Dijon à Besançon et nous n'avons pas besoin de jacobinisme régional la décentralisation c'est pas ça c'est la vitalité de tous les territoires d'autant plus que on on hérite d'un passif. Qui est significatif. Ça a été évoqué par certains parfois des grandes zones commerciales aux entrées de nos communes qui ne leur font pas honneur des zones pavillonnaires aussi parfois qui ont été construites hélas un peu sans respecter le caractère du pays et on voit ce que ça donnait. Christophe dit lui s'est penchée dessus. Voilà pourquoi, madame la présidente. Sur l'article, il faut que nous ayons le débat et que nous le votions. À terme, je vous remercie. Merci la parole d'amitié avec Merci madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues. Notre collègue Cécile qui Hermann l'a dit tout à l'heure effectivement le nombre de prises de parole révèle les inquiétudes que suscite. Ce texte de loi votée il y a 2 ans, elles sont réelles et nous faisons remonter de des territoires. L'ensemble des préoccupations et c'est tout à fait légitime pour ma part. J'ai tendance à ne pas parler de 0 artificiel sur net parce que je considère que cet objectif est quasi inatteignable. Autant il faut que l'on fasse des efforts sur la sobriété foncière pour éviter que l'on en consomme trop autant peut être cet objectif de viser au 0 ratification date peut paraître prétentieux parce que il faudra constamment qu'on puisse s'adapter aux évolutions de notre temps. Il faudra constamment que l'on puisse trouver des espaces pour le développement économique qu'ils soient industriels mais qu'il soit également agricole pour répondre aux besoins de logement de nos concitoyens. On est loin d'y avoir répondu à l'heure actuelle, c'est dire que les défis sont nombreux et moi, je veux dire que l'examen de ce texte est particulièrement. Salvateur dans le sens où j'espère que le gouvernement va entendre les différentes préoccupations qui remonte des territoires et les s'intégrer dans la manière d'interpréter. La loi qui a été votée parce que c'est bien cela le problème, c'est que l'interprétation qu'on a fait les services de l'État a été bien souvent. Soumise à contestation. Et il importe donc que l'on puisse bien de prendre en compte la réalité de ce qu'a fait remonter la représentation nationale. Merci la parole est maintenant à Jean-Michel Arnaud. Oui madame la présidente. La longueur des interventions cet article 1er montre le malaise qu'il y a dans les territoires. Je voulais porter témoignage de mon vécu dans la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur la première région de France qui a mis en place, on sera dette. Hein, serait d'être conçu. À Marseille, à Nice et à Toulon, de manière excellente. Je n'en doute pas, mais dans tous les cas avec une compréhension du au pays des territoires les plus ruraux qui reste à démontrer. Et nous avons ensuite. Une sorte.

Et au bout du compte des élus. Une population qui ne comprend plus ce que l'on fait dans nos territoires qui ne comprend plus, où on les amène. On se demande où sont les Philippe Lamour où sont les Olivier Guichard de l'aménagement du territoire qui ont mis en place des politiques importantes en matière de structuration et aujourd'hui nous sommes dans une situation où il y a une cassure avec nos concitoyens qui attendent. Des solutions en matière d'habitat des propriétaires qui s'interroge sur la manière donc ils vont pouvoir demain louer leur logement et effectivement un équilibre entre développement économique préservation des Terres agricoles et capacité à bien vivre dans nos territoires. Je crois qu'il est important que à travers ce texte et je salue le travail fait par Jean Baptiste. Et également par Valérie qui apporte des solutions pragmatiques à un texte qui était inaudible dans nos territoires et je reviens également sur ce qu'a dit Monsieur le Ministre tout à l'heure, ce n'est pas parce que le Sénat, le Parlement a voté ce texte qu'il a voté le détail de chacun de ces éléments et c'est bien évidemment lorsque les décrets ont été publiés que ont été révélés dans les territoires, la réalité de la portée de ce qui avait été voté et c'est bien là la difficulté que nous avons entre un texte voté par les parlementaires et la réalité transmise interprété par l'administration, dans les territoires qui est en contradiction avec les objectifs qui étaient des objectifs de sobriété et d'équilibre et d'aménagement du territoire. Merci. Jean-Marie Vanlerenberghe derrière. Auteur en principe. Merci madame la présidente, moi j'essaierai effectivement. D'être sobre et donc de parler d'être bref. Je voudrais quand même saluer le travail qui a été effectué par Valérie Létard et puis Jean-Baptiste Leblanc qui est essentiel pour répondre effectivement à l'inquiétude. Que l'on sent monter de tous nos territoires 2 ou 3 remarque rapide. Une première. Concernant. La gouvernance régionale. Jean-Baptiste Lemoyne la rappeler attention jacobinisme régional je l'ai vécu, je le vis encore et je pense qu'il est important de rapprocher le plus possible la gouvernance. Du territoire. Donc, c'est une gouvernance de proximité dont on a besoin dans ce domaine. 2ème remarque concerne les grands projets. Ça a été dit par un certain nombre de vos collègues des grands projets régionaux, ils doivent être comptés à part. On a, je suis de la région de France, un grand projet d'envergure d'ampleur européenne nationale régionale c'est le canal Seine Nord. Beaucoup de communes vont être impactés par ce canal. si on ne fait peser sur ces communes. Je dirais évidemment l'artificialisation. Passer la double peine. Donc je crois qu'il faut absolument qu'il y ait une mesure très claires qui soient prises dans ce domaine. Et puis dernière remarque, ça concerne Lescott l'épée, j'en ai présidé hein. Je peux vous dire que on a appliqué la loi notre sur ces Scott c'est pas lui. On a été, je dirais vertueux dans ce domaine. Si effectivement aujourd'hui on applique à nouveau. La règle des 50%. Ça devient effectivement très difficile à gérer. Est ce qui ne serait pas possible de lycée de la période 2011 jusqu'à 2031. Les efforts d'artificialisation qui auraient été effectués. Dans ces Scott et dans CP à lui. Et dernier point sur les décrets je crois Monsieur le Ministre, que souvent malheureusement dans les décrets, on ne respecte pas l'esprit du texte fait très attention à ce qu'ils seront pris ensuite. Monsieur le ministre vous souhaitez aussi intervenir. Pas sur l'article hein mais mais quelques mots quand même sur tout ce qui a été dit, parce qu'il y a des choses si je les laisse passer, là, on risque de partir dans des directions qui ne sont pas les bonnes. D'abord. Sur les décrets. Ils ont été pris le 29 avril. Je suis arrivé le 4 juillet, je les ai suspendu le 6 août et le 29 août. J'avais la première réunion de travail avec la présidente Prima et de manière transpartisane avec une partie des sénateurs donc je propose que sur ce point je ne vous renvoie pas au vote de la loi climat et résilience et vous ne me redit pas qu'il faut écouter les parlementaires parce que sinon on serait pas là. Dans cette configuration sur un texte sénatorial 2ème point. La moitié de la consommation d'espace. Sur les 10 dernières années. C'est avec une densité moyenne inférieure à 8 logements à l'hectare. Dit autrement, la moitié de la consommation s'est faite avec un pavillon et 1100 m2 d'espaces agricoles autour. C'est dire les marges que nous avons et c'est dire à quel point il serait faux de dire ce serait la fin de la maison individuelle si on passait de 25.000 à 12.500. Ça voudrait dire qu'on aurait plus des terrains de 1000 m2, mais les marges ne sont absolument pas d'aller imaginer qu'on met des tours en milieu rural, c'est faux. Troisièmement, pour que les chiffre soit juste 9% c'est la surface artificialisées de la France à la minute où nous nous parlons. Ce 9% il est à comparer aux 5. De de 1982. C'est ça le sujet, c'est les 70% d'artificialisation en plus en l'espace de 40 ans qui ont été marquées par 10% de la réduction de la surface agricole dans notre pays et nous ne sommes pas sur un zéro parce que je rejoins la formule de Monsieur Paco le problème du zéro artificialisation nette c'est que ça claque comme formule marketing mais on parle d'après 2050. On ne parle pas de maintenant et il y a des gens qui entendent le zéro comme si s'impliquer demain matin alors qu'on discute de comment on répartit 125.000 hectares pour les 10 ans qui viennent plus 170.000 hectares de friches plus des logements vacants. Donc on a un sujet sur lequel il y a les voix et les marches pour être capable d'avancer enfin je termine là-dessus. Faisons attention à ne pas parler que de densité. Oui on a une densité par habitant plus faible que les autres mais le paradoxe. C'est qu'on a une surface d'artificialisation par habitant plus élevé. Je vais le dire autrement. Pour 100.000 habitants, nous avons 47 km2 d'artificialisation et ça, c'est le chiffre le plus élevé d'Europe. Parce qu'on a décorrélés. Une artificialisation qui reposait sur le fait d'accueillir des habitants et des activités. Par une artificialisation aujourd'hui on a fait effectivement des zones commerciales de périphérie qui ont fait exploser une partie du foncier. Et par le fait qu'on est parti sur des lotissements qui sont pour le coup, elle en compte du bon sens de nos anciens. Il y avait pas Greta Thunberg. Il y avait pas le Grenelle de l'environnement, il y avait pas, il n'y avait pas les acronymes et la Convention citoyenne mais c'est pas, c'est quoi. Il y a 200 ou 300 ans dans toutes les communes de ce pays le modèle c'était pas, je pose une maison avec un jardin autour c'était je réserve les jardins pour avoir des espaces qui permettent de se nourrir et je fais en sorte de coller les maisons y compris pour limiter les matériaux que nous faisons et nous centre-bourg dans toutes nos communes rurales. Ils répondent à ce modèle. Et ça a pas été une injonction de la Dreal ou de qui que ce soit. C'était le bon sens de nos anciens pour limiter les matériaux et limiter les espaces agricoles. Je dis pas qu'il faut retenir, là-dessus on a d'autres modes de vie mais je dis que pour partie. On ne peut pas ne pas regarder un minimum ce qui s'est fait par le passé et se dire qu'entre le modèle qui consiste à avoir 8 pavillons à l'hectare. Et le modèle qui consiste à ne pas avoir un mètre carré pour que la terre respire on a largement les voies et moyens avec 125.000 hectares et tout ce que je viens d'indiquer, de trouver des trajectoires qui soit respectueuse à la fois des besoins de l'humanité. Ils sont réels. Et d'une planète qui nous fournit la plupart des systèmes dont nous avons besoin, y compris pour continuer à vivre en bonne santé, dans de bonnes conditions. Alors nous allons prendre l'amendement 186 de Monsieur Dantec. Oui merci madame la présidente. Cet amendement est une tentative, probablement un peu prétentieuse. D'arriver à un compromis sur sur les dates. La, la commission spéciale considère qu'il faut laisser aux régions. Plus de temps pour le Qu'effectivement avec cette nouvelle contrainte hein Dusan il faut rebalayer les documents même si quand même beaucoup de régions ont déjà anticipé. Donc on laisse plus de temps aux régions, mais le calendrier proposé repousse l'ensemble du calendrier aussi pour les les Scott et les et et les plus et si vous regardez bien par rapport aux municipales. Ça veut dire que les nouvelles équipes municipales vont arriver en phase d'élaboration du Scott. Vont attendre que le Scott soit adoptée et devront encore après. Hein le le plus et ce qui veut dire qu'on sera déjà très très proche de 2031 et donc. On aura finalement très peu d'années pour que les nouveaux plus. À l'échelle des communes ou des lui finalement. Utilise. Face, vive la règle du moins 50% qui n'est pas. Comme l'a dit le ministre. Encore un zéro artificialisation. Donc nous ce que l'on propose, c'est que les nouvelles équipes municipales arrive juste au moment où le Scott est adopté et un an derrière jusqu'à la fin 2027 pour un, un, faire leurs propres plus c'est un calendrier plus cohérent et simplement pour faire ce calendrier on baisse de 4 mois le temps donné en plus aux régions et on baisse juste en fait ensuite de 2 mois pour les Scott et pour les plus en réduisant le temps. Pour le le préfet et et l'autorité administrative de valider le nouveau document, ce que nous faisons déjà dans la proposition de la Commission pour l'Australie. Donc c'est une proposition à mon avis assez de bon sens qui qui respecte à la fois le calendrier électoral et l'arrivée des nouvelles équipes et qui répond aussi à beaucoup d'inquiétude sur le fait. Une mère on est trop court. Monsieur Dantec. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement. Madame la présidente. Ce sera un avis défavorable, parce qu'en fait si je reviens à la à la jeunesse de l'histoire, on a voté ici, quelles que soient les bancs souvent. La territorialisation de l'objectif, c'est-à-dire un droit de propositions que pouvait exercer Scott et en réalité, ce droit de propositions août qui n'a pas été très accompagné ça a été dit ça et là dans les interventions, je vais pas m'étendre hein le manque d'ingénierie notamment ça ça que je fais allusion, ce droit de propositions a atterri, quand il a atterri sur la table des régions le 22 octobre, qui avait jusqu'au 22 février pour discuter c'est pas sérieux comme délai de discussions pour une concertation réelle donc non c'est ça c'est pour permettre une vraie concertation. Alors il est évident qu'il faut sécuriser juridiquement. Tout cela

Si vous me permettez je vais éclairer tout ce qui va se passer sur l'article 1 en disant que le gouvernement fait confiance à la sagesse du Sénat. Et ce qu'il faut être sur un an sur huit mois et cetera de toute façon nous considérons qu'il faut assouplir les délais. Je ne connais pas la date à laquelle la discussion avec l'Assemblée aura lieu. La position initiale et elle est plutôt là bas de 6 mois mais qu'on ait une position qui amène une CMP avec une version un peu plus haute. À huit mois ou à 12 mois, ne me choque pas et donc ce sera sagesse je reprendrai pas la parole sur ces différents éléments de calendrier parce que c'est la concrétisation de l'assouplissement et du fait de se donner un peu de temps. Merci je vais donc me donner la parole à Monsieur Dantec pour une explication de vote. Oui effectivement on, on cherche à anticiper une CMP donc l'Assemblée d'ici moi nous on on dit 12 mois. Moins. L'amendement que je propose dit huit mois, mais surtout il faut bien comprendre quand même que pour les communes. Qui vont devoir mettre en oeuvre. Le moins 50%, les nouvelles équipes municipales la Saint-temps extrêmement court extrêmement court et comme l'a dit le rapporteur. Pour le préfet, c'est possible. Donc en fait on ne perd rien sur la mise en oeuvre pour les communes et pour. Hein, hein à l'échelle du Scott en grattant ses quatre mois là donc. Et pour avoir beaucoup échangé avec un certain nombre d'acteurs communaux, y compris avec des maires. De Loire-Atlantique. Avec lesquels on on les interroger pour dire à ce que vous voulez beaucoup beaucoup de temps. En plus, ils ne veulent pas obligatoirement donc je je pense que ce qu'on propose la éteint est vraiment un bon compromis et qui correspond à la dynamique politique de l'élection municipale. qui me semble assez cohérent qui sera peut-être sur la table du compromis en CMP avec l'Assemblée nationale. Je vais donc mettre aux voix il a reçu un avis défavorable de la commission et un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 231 monsieur pieds-noirs. L'article 1er prévoit globalement une accélération de la procédure de modification d'Estrada, tout le monde l'a l'a bien compris et notamment. En proposant le de réduire de 3 mois à un mois le délai laissé aux préfets pour approuver le sera d'être alors je vous propose, à travers cet amendement tout en poursuivant l'objectif d'accélération mais sans prévoir de délais trop contraint de un amendement qui propose donc de passer ce délai d'approbation par le préfet. À deux mois à mi-chemin. Donc ce qui correspond au premièrement à un délai classique en matière de droits d'urbanisme que l'on peut observer à d'autres sur d'autres exemples et Kate comme mon collègue, une forme de d'anticipation sur une une éventuelle CMP sur ce texte puisque on est à mi-chemin entre les deux délai proposé jour. Quel est l'avis de la commission. Madame la présidente. C'est un avis défavorable, parce que le préfet est associée en amont de toute révision de. En amont de l'élaboration de du projet de sera dette pardon a donc bien connaissance en avant sa transmission pour approbation ce délai d'un mois nous paraît insuffisante, donc c'est bien. Merci monsieur sagesse. Monsieur Piednoir. Il est retiré. 2 amendements faisant l'objet une mission commune, commune, on commence par le 187 de Monsieur Dantec. L'enquête publique a lieu en même temps que le, le travail de de l'autorité environnementale. Alors qu'on a quand même 2 ans. Entre. L'adoption du sera dette et l'adoption du du ça n'est absolument pas nécessaire, c'est-à-dire que si on avait l'enquête publique après l'avis de l'Autorité environnementale qui est clair, évidemment. L'enquête publique, on aurait exactement les mêmes délais. Donc moi je propose qu'on en revienne hein hein. Ce qui est la règle habituelle qui est que, on a d'abord la vie des personnes. Associées et de l'autorité environnementale puis l'enquête publique, et ça ne change rien, ça n'a pas le lien avec l'amendement précédent. Ça ne change rien au télé qui sont aujourd'hui proposées notamment les deux ans quand même entre l'Austra dette et le Scott.

En fait, pour rappel en commission monsieur Dantec. Nous avons étendu cette possibilité de mener des consultations simultanées aux modifications des squats et des PLU il pour répondre à l'inquiétude exprimée par les élus des collectivités locales sur le calendrier donc sur un avis défavorable. donc je vais. Monsieur le Ministre toujours sagesse sur les deux amendements. Je vais donc mettre aux voix 187 qui a reçu un avis défavorable de la commission. Un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté le 261 qui a reçu un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté le 157 monsieur saumon. Oui madame la présidente, monsieur le ministre. Aujourd'hui, nombre de communes rurales se voit opposer des refus d'autorisations d'urbanisme voir des excès d'interprétation de règlement ou référence à une jurisprudence. Toujours plus. Restrictive la trajectoire than et déjà anticiper avant même que les documents qui en fixeront les disponibilités territoriale ou communal ne soit adoptée, je pourrais citer les exemples dans mon département de Doulan ou Amiens. Alors les élus locaux sont déférés au tribunal administratif si d'aventure il juge le devoir de les accepter.

et donne aux élus locaux responsables pourtant détenteurs de la compétence urbanisme vidé de sa consistance de subir l'empêchement voir le ralentissement de leurs projets. Cet amendement propose d'étendre le spectre d'intervention de la commission départementale de conseillers et de conciliation sur saisine des élus locaux pour défendent les droits à construire lors de litiges la délivrance et l'élaboration des documents d'urbanisme soumis à la loi than afin de garantir le droit de chaque commune et le respect du juste équilibre territorial des droits à construire, à quoi servirait, y a-t-il servi de voter une loi 3DS si quelques mois après dans une autre loi on éloigne la décentralisation ont dévitaliser la déconcentration et on gomme la différenciation. Madame la présidente. Je comprends l'intention évidemment monsieur saumon le. Néanmoins, il les, il paraît que cet cet amendement transforme la logique de de la commission de conciliation que que nous avons mis dans cette PPL donc en opposant les collectivités les unes aux autres, alors que nous cherchons de la conciliation de la coopération entre entre les niveaux.

Pourrait continuer à s'appliquer même une fois qu'on aura modifié l'âne en faisant en sorte d'en corriger les défauts puisque la commission de conciliation aura à connaître de tout ce qui concerne Lausanne c'est-à-dire les trajectoires donc tous les documents d'urbanisme et on transformerait à partir Didier temporaire. Un dispositif dont on peut comprendre l'intérêt à court terme on un dispositif qui viendrait superfétatoire ou dangereux à moyen ou long terme. Il est maintenu. Je le mets donc on voit cet amendement 157 double avis défavorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté je l'article 1er qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté après un article 1er un amendement 46 monsieur. Oui merci madame la présidente. J'allais dire comme un âne, tauromachie. Nous allons faire un Mano Ahmad avec madame ex Estrosi Sassone puisque nous avons présenté le même amendement demain donc moi je me permettrai de présenter juste le cadre juridique je laisserai ma collègue et amie présenter les motivations. Donc nous souhaitons donc insérer un article additionnel ainsi rédigé au 1er alinéa de l'article 191 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ces effets, les mots d'atteindre sont remplacés par les mots de tendre vers. Merci madame la présidente. Donc pour faire suite à l'intervention de mon collègue de Goa dans nos amendements. Ce que nous avons voulu faire ses visées à redéfinir une rédaction qui soit plus incitative et programmatique plutôt que contraignantes de l'objectif de zéro artificialisation nette telle qu'il est prévu dans l'article 191 de la loi climat et résilience, pourquoi parce qu'aujourd'hui, le texte prévoit bien une définition de la notion d'artificialisation nette des sols mais il renvoie à la publication d'un décret pour la définition des notions de sols artificialisés ou non n'artificialiser or ce décret, nous le savons tous maintenant il fait l'objet aujourd'hui d'une action contentieuse pendante devant le Conseil d'État et vous-même Monsieur le Ministre, vous avez annoncé sa réécriture aussi en l'absence de définition précise tant sur la notion d'artificialisation de renaturation de sols artificialisés ou de non artificialiser. Il nous semble, à travers cet amendement que l'objectif de la loi doit rester incitatif et programmatique. D'autant plus que l'échéance et particulièrement lointaine puisqu'elle vise 2050 de plus. Je rappellerai également que l'inscription d'un objectif contraignant peut entraîner des conséquences juridiques particulièrement grave et importante. Comme nous l'avons vu récemment avec l'affaire du siècle, ces organisations citoyen avec les citoyens qui assigne l'État en justice pour inaction face au changement climatique. Monsieur avait. Défendu. Je vais donc demander l'avis de la commission sur ces trois amendements identiques hein enfin sur cet amendement,

Pour autant, je me rappelle aussi le cadre de cette commission spéciale qui vise à donner des outils aux élus et à préciser des définitions. Donc. C'est en cela que proposent de cheminer. Avec ce ce texte de sagesse. Monsieur le ministre, on est plus sur l'article hein donc défavorable pour les mêmes raisons. À partir du moment où on explique qu'on croit à la démarche qui consiste à lutter. Contre l'étalement urbain cette borne de 2050 et là évidemment une valeur symbolique extrêmement forte et là aussi je ne doute pas qu'entre maintenant et 2050, on aura d'autres occasions d'évoquer, c'est un ou qui n'est pas personnel mais qui est institutionnel. Une partie du chemin qu'il nous restera attendre mais c'est une borne européenne dans le même temps monsieur Beuchere pas. Explications de vote. oui madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La semaine dernière en audition sur la mission d'information, créée par à l'initiative du groupe RDSE. Nous Odyssey oignons Monsieur Alain Lambert. Président de la commission nationale d'évaluation des normes. Et notamment des normes pour les collectivités locales. Monsieur le Ministre. Que nous a-t-il dit. Arrêtez de vous remettre à des décrets. La loi et travesti au fur et à mesure dans les décrets. Et donc je vais soutenir ces amendements. Parce que je le crains. Monsieur le Ministre, l'administration. Ici, pas forcément la volonté politique parce que le diable est dans les détails et on sait combien vous avez à voir et à faire. Il n'y a rien de personnel. Mais l'administration. À Paris. Comme l'administration locale. Interprète sur interprète prend de l'avance. C'est ce que nous ne cessons de dénoncer et donc déjà presque en avance sur les conclusions de la mission d'information et sur l'invitation d'Alain Lambert bien connu dans cet hémicycle. Je vais donc voter l'amendement proposé par collègues. Monsieur ai. Merci madame la présidente. Je ne comprends pas bien votre position. Monsieur le Ministre, parce que à plusieurs reprises depuis le début de nos débats. Lorsque vous avez été interrogée sur cet objectif de 2050. Vous avez dit vous-même et vous venez de le répéter qu'effectivement c'était assez loin, qu'on pouvait revenir éventuellement dessus pour évaluer cette cette politique et donc, si effectivement c'est si loin que cela, et cela demande une évaluation dans quelques années, je pense que de notre, de nos deux collègues et tout à fait le bienvenu puisqu'il garde la direction. Il garde la volonté mais je crois qu'il permet également de prendre en considération tout ce que vous avez entendu sur nos bancs. Depuis le début de l'examen de ce texte et je pense que cette prise en compte. Cette prise en compte des inquiétudes que nous vous avons rappelé. Serait tout à fait bienvenue. Ce sera un geste tout à fait important d'autant plus que je rajouterai par rapport à ce qu'a dit mon excellent collègue Bachar que bien sûr il y a la façon dont l'administration va appliquer ces textes mais moi ce qui me marque beaucoup pour participer. À l'élaboration d'un lui dans ma communauté de communes du Grand charolais c'est que désormais. Au-delà de la loi. Il y a le message porté par tout cela et je vois que beaucoup de mes collègues intègre déjà. Tout ça de façon un peu jusqu'au-boutiste et comme ça déjà été dit sur. D'autres bancs et bien effectivement se disent qu'il faut plus aucun développement et je pense que dans les années qui viennent on va avoir beaucoup de difficultés à accueillir des entreprises logistique entreprises industrielles parce qu'effectivement tout le monde n'a qu'un mot à la bouche, Lausanne et c'est parfois effectivement compris de façon très très accessible. Je rajouterai également les bureaux d'études qui effectivement nous accompagne dans l'élaboration de ces documents et qui sont pour le coup, toujours très velléitaire et donc je pense que dans l'expression de la volonté parlementaire le fait de pouvoir clarifier les choses et adopter cet amendement serait tout à fait bienvenue et conforme à tout ce que l'on veut faire avec ce texte. Madame la présidente de la Commission spéciale. Merci madame la présidente, chers collègues, tout en comprenant et en partageant l'intention qui est la vôtre. Je crains vraiment. Et. Ça a été l'objet de toutes nos réflexions et du travail que nous avons fait sur l'article de que nous, nous sommes sur un article qui est programmatique que le vrai sujet qui nous inquiète aujourd'hui et je vais aller au bout de mon explication. Le vrai sujet qui nous inquiète, aujourd'hui, c'est le caractère prescriptif ou non prescriptif du sera le vrai débat sur lequel nous sommes tous inquiets c'est cet aspect qui est dans l'article de si l'on veut vraiment être efficace concret et agir au bénéfice des territoires et de faire en sorte que tout en ayant des ambitions fortes pour atteinte des objectifs que nous avons tous répété. Considérer comme étant essentiels. On sait que nous devons aller vers la sobriété foncière mais je pense que si on veut effectivement ne pas être dans une espèce de Scott régional où tout va être vertical Izé. Extrêmement descendant agissons sur l'article 2, celui-là ne changera rien, simplement moi je pense vraiment que si dans ce texte, nous revenons sur les objectifs alors que nous avons dit du début à la fin de la commission spéciale que les objectifs, nous les partagions y compris suite 2050. À ce moment-là, nous saurons ce qui avons détricoter la loi climat. Nous ne voulons pas remettre en question les objectifs ce nous ce que nous ne comprend pas tout ce que nous ne comprenons pas pardon. C'est pourquoi il n'y a pas une coproduction entre une vision stratégique de l'État et des territoires qui peuvent être acteur aussi de leur propre développement. Il faut que nous agissions sur l'article 2. Soyons présents mais si nous votons ces amendements. Alors je pense que on nous le reprochera et nous n'atteindrons pas la la cible que nous souhaitons tous. Je vais donc mettre aux voix, ces trois amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable de la commission est défavorable du gouvernement qui est pour

est contre.

Oui madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans nos outre-mer la trajectoire Dusan et de la réduction du rythme de l'artificialisation est fixé, vous le savez par l'article 194 de la loi climat et résilience qui le confie Auxerre schéma. D'aménagement régionaux. La loi climat et résilience n'obligeant pas les ça à réduire de moitié leur consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers par rapport à celle des 10 années précédentes, l'obligation qui s'impose en cas d'absence d'évolution des schémas régionaux à Paris disproportionnée cette règle devient une double peine pour les collectivités d'outre-mer pour lesquelles le schéma régional ne serait pas mis à jour aussi notre amendement prévoit d'écarter l'obligation automatique d'un objectif de moins de 50% au niveau infra-régionale en cas de retard de l'échelon régional. Merci. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement Le rythme d'artificialisation 2000 d'ici 2031. Donc je comprends fort bien la logique de votre amendement il serait baroque en effet que les collectivités se voient mécaniquement imposer une réduction. De 50% si les Sarr n'était pas modifié dans dans les temps. Mais si nous supprimons cette disposition quelles incitations aurait les régions d'outre-mer à modifier leur dans le délai imparti. Il est certain qu'une modification des soeurs d'ici 2024 n'est pas tenable. C'est pour cette raison que la PPL prévoit que comme pour les Sraddet. Un délai d'une année supplémentaire pour les modifier. Précisément et donner du, du temps sera donc un avis défavorable. Monsieur le Ministre, quel est votre avis. Sagesse parce que j'entends en même temps la problématique de caractère automatique. Pour partie en décalant les délais, on augmente le délai enfin on augmente la possibilité que les régions puissent modifier mais si à la fin, ça n'est pas fait et que c'était automatique comme c'est l'objectif que nous ne souhaitons pas. Que c'est pas ce qui est prévu pour la partie métropolitaine. Ce sera un avis de sagesse. Bien je vais donner la parole monsieur Mohamed Soihili pour une explication de vote. Oui un délai supplémentaire d'un an en cas de non respect, c'est bien l'aveu. Que. Ce n'est pas ce n'est pas satisfaisant. Vraiment il faut me connaître les territoires d'outre-mer pour penser que. Une une compensation d'un délai supplémentaire. Peut suffire à atténuer les effets automatiques engendrerait la loi si on on ne la changeait pas. C'est pour ça que vraiment j'insiste sur cet amendement les collectivités d'outre-mer sont. Déjà suffisamment assujettis à des à des contraintes pour ne pas en rajouter. Et je. Vraiment je vous exhorte chers collègues à voter cet amendement. S'il n'y a pas d'autres explications de vote, je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la commission et un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 17 un article additionnel de Madame Espagnac. Oui madame la présidente merci ça. Cette disposition organise le report de l'échéance de la loi climat pour les communes situées en zone montagne au sens de la loi montagne. À cet effet, elle exclut ces communes de l'application de la première période décennale de réduction de 50% de la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers par coordination afin de ne pas faire peser un effort plus plus conséquents sur les communes non montagneuses, des régions qui comprennent des communes de montagne elle modifie le sera d'être de ces régions. Le décompte de la consommation des Hénaff observés sur les 10 dernières années. Base de calcul de la réduction de l'artificialisation. Afin d'en exclure la consommation observée dans les communes de montagne. Quel est l'avis de la commission. Supplémentaires pour rester dans le cadre telle qu'on s'est fixé et là sans sans en une. Toute évidence et puis les spécificités des territoires sont déjà prises en compte par par les régions. C'est d'abord laissera dettes et plusieurs dispositions de la PPL ne cesse de, de conforter ses spécificités de de de la loi montagne outre est source de complexité que cela pourrait engendrer dans l'élaboration des squats et des lui qui couvre à la fois des communes de montagne et d'autres communes. Je réitère retrait ou défavorables. Monsieur le ministre. Au mot près, la même position que le rapporteur. Madame Espagnac, je veux dire. À l'article de Monsieur le Ministre aux États vous pour l'amendement 159. Nous sommes. Sur un noeud. Gordien. Et l'amendement du gouvernement, ça n'a rien de très original, ce sera. De préciser que nous souhaitons maintenir la portée juridique du Sraddet tu et Dussart. Si nous ne le faisons pas. On peut gagner du temps sur le reste de nos échanges, parce que si la trajectoire n'est qu'indicative. Rien ne nous garantira qu'on sera en situation de diminuer. Cette consommation foncière. Donc cet article, c'est un rendez-vous de vérité sur l'effectivité du dispositif et il fait clairement partie des lignes rouges pour nous. La commission sur cet amendement du gouvernement. Alors Madame la Présidente effectivement c'est le noeud gordien. Le point dur là la ligne rouge écarlate la la fameuse là voilà. Alors ça été exprimées ça et là sur sur tous les sur tous les bancs. Nous ne voulons pas ici au Sénat, je dis nous c'est peut-être Un peu exagéré mais enfin on ne sont très nombreux à penser que il y a une forme de jacobinisme régional dans ce sera dette qui devient de plus en plus contraignant normatif inclusif intégrateur alors que quand on reprend l'histoire de ce sera d'être finalement. Que nous dit que nous dit-elle. L'histoire de sa dette nous dit que c'est un document de. d'ensemble de d'orientation de stratégie et non pas de planification, sauf pour les dernières dispositions qui concernent la biodiversité. Quand on regarde en réalité en détail. Alors en même temps il y a un sens de l'histoire ne sont pas naïfs sur le sujet. mais en l'état, nous pensons vraiment que ce ce sera être ne va pas devenir normatif tout tes es dans le détail et le diable en particulier donc les mots de prise en compte. Nous y sommes tous collectivement très attaché. et non par les mots de mise en compatibilité la prise en compte laisse plus de marge manoeuvre un petit peu plus de liberté. Alors, je vous assure qu'il faut faire confiance aux élus pour s'inscrire dans la tragédie. ce sera d'être d'autant plus que l'État est partout. À côté des régions pour contrôler la légalité des trajectoires. Il y a des clauses de rendez-vous très régulière qui font que. Nous ne pouvons que collectivement cheminer dans dans le bon sens mais encore une fois, vraiment ça serait un signal important donné au Sénat que d'accepter la prise en compte le Sénat accepte le fascicule réglementaire mais il veut changer la nature du rapport juridique à ce fascicule. Réglementaire.

Le caractère. Non obligatoire. Des fascicules du sera dettes est une ligne rouge pour le Sénat. Si vous partez du principe. Que vous ne voulait pas en discuter, nous serons en opposition frontale. Le centralisme. Régional. N'a rien à envier au centralisme d'État surtout quand vous en fait le bras armé par la loi. La région n'a pas de compétence en matière d'urbanisme. C'est une véritable inversion de perspective par rapport aux grandes lois de décentralisation. De 1982 et des années qui ont suivi et qui ont confié aux maires et aux représentants des communes dans le cadre des plans locaux d'urbanisme intercommunal le soin de mettre en oeuvre la planification urbaine et je crois que là nous sommes effectivement, et vous le dites avec franchise sur un point qui est un point absolument essentiel pour lequel nous nous séparons absolument.

pour rappeler l'attachement qui est le nôtre au Sénat aux libertés locales en général et donc sur l'urbanisme en particulier, la place des communes, la place centrale des communes ne peut pas être remise en cause L'histoire de la décentralisation de de de notre pays qui serait totalement renversé c'est un déblocage d'ailleurs que l'on rencontre aujourd'hui ou d'incompréhension avec l'application Dusan c'est c'est ce sentiment qui est plus qu'un sentiment de voir la maîtrise de son développement, la maîtrise de de de de de l'avenir de son territoire de sa commune échapper aux maires, aux élus locaux et l'incompréhension que ça suscite auprès de la population. Donc je crois qu'effectivement on est sur un noeud gordien et et et et qui sera Alexandre est-ce que ça sera le Sénat où le gouvernement mais mais vous comprenez bien que c'est une ligne qui pour nous est indépassable. Et j'ajoute que la territorialisation Dusan qui nécessite que l'Austra dettes soit un outil stratégique et non pas prescriptifs est absolument essentiel dans la vision qui est la nôtre. Voilà donc je voulais juste ajouter ses, ses arguments à ceux qui avaient déjà été développé merci. Oui merci. Monsieur le Ministre. Je pense que l'on a déjà évoqué cette question que le ça très de sera dette deviendrait un super-Scott et ce n'est pas absolument pas d'abord l'objet de la loi c'est pas l'esprit de ce que nous avons voté, c'est même complètement contradictoire. Et ça créerait de fait une tutelle de la région sur tous les autres territoires à toutes les collectivités en dessous avec. Une espèce de de déclinaisons automatique qui empêche complètement la respiration, la liberté et l'Intelligence collective dans dans les territoires. C'est pas parce que. On on laisse la discussion, le travail se faire la réflexion commune. L'aménagement du territoire en commun. Se mettre en place, que ça va être la chienlit ou l'impuissance. Je suis désolé d'avoir ces termes un petit peu un petit peu triviaux mais c'est quand même un peu ça qui est qui est sous-entendu et moi je crois beaucoup que donner un cap et une vision c'est laisser les autres s'emparer des outils trouver les voies les mots et les les voies et les moyens les plus adaptées pour que sur le terrain ça colle et la différenciation c'est tout simplement ça. Madame Challes Archer. Oui, Monsieur le Ministre, nous avons mis en place, vous le savez sans doute, une mission d'information sur l'avenir du maire et de la commune. Les auditions se multiplient au sein desquels nous entendons les voix des maires très simplement s'exprimer en faux contre les effets pervers de la loi notre. Je parle aussi des lui qui sont pour eux un véritable problème et qui bien entendu ne comprennent pas les excès qui ont amené cette zéro artificialisation nette. Ce sont des territoires notamment les territoires ruraux qui vont devenir des territoires dortoir dans lesquels les enfants du pays ne pourront plus avoir une maison à accéder à la propriété dans lesquels des entreprises familiales sur plusieurs générations ne pourront pas construire de siège social attractif pour des cadres et et pour des employés qu'mérite d'avoir. Autrement dit, ce seront des territoires qui vont mourir. Or ces territoires-là n'ont pas envie de devenir des réserves d'Indiens ou les urbains pourront venir. Eh bien. Voilà s'amuser dans les champs, dans les prairies, ils ont tout simplement envie de vivre de leurs propres moyens et également se développer faire en sorte que systématiquement une puissance puisse déterminer l'avenir de ces territoires est une erreur majeure, c'est non seulement une erreur mais c'est aussi un mépris pour l'exercice du maire pour le travail qu'il représente pour le dévouement qui est le sien pour ces équipes qui mieux que personne connaît, ce qui est bon pour l'avenir de leur territoire et le défendent en général de façon totalement bénévole. Donc vraiment je vous demande d'entendre notre discours ici au Sénat, comme vous le savez puisque vous l'avez été vous-même, sénateur et maire le Sénat défend les collectivités et des nous à les défendre.

moi je vous entends. Mais vous croyez vraiment qu'un maire de petite commune seul face finalement aux préconisations de l'État. Il va, il va s'en sortir mieux c'est pas vrai. On a besoin de région forte qui rééquilibre le territoire régional sinon vous allez avoir des métropoles, elles existent et des petites communes sans moyens qui vont faire au mieux mais qu'ils n'y arriveront pas et qui ne régleront aucun problème d'accès au logement, aucun problème. De développement économique. Ça n'est pas vrai. Nous non nous ne sommes plus en 1982, le monde n'est plus celui 19.182. La loi notre a dit que face à un monde complexe, il fallait de la planification régionale. Ce que nous rajoutons. Dans, dans le travail de la commission spéciale où il y a des avancées, c'est en amont du strat une conférence beaucoup plus puissante et ouverte. Compris à des maires de petites communes à à des élus départementaux et après nous avons besoin d'un schéma prescripteurs sinon nous ne répondrons à aucun strictement aucun des défis. Sur lesquels vous insistez. Seul il ne répondra à aucun de ces défis, vous aurez simplement un développement totalement, totalement lié à la puissance des grandes villes et des métropoles. Au contraire, c'est la région qui peut rééquilibrer après le rapport de compatibilité n'est pas un rapport de conformité. La Convention citoyenne proposer la conformité ici la compatibilité. Bah oui, donc vous voyez on a évité on a évité le désastre. Donc le rapport de compatibilité laisse beaucoup et tous les jurisprudences vont dans ce sens là beaucoup de marge de manoeuvre au bloc communal. C'est le bon équilibre et il faut renforcer par contre à la concertation en amont. Oui merci madame la présidente, chers collègues, en complément de tout ce que mes collègues ont dit rappeler évidemment. À la base que le texte sorti de CMP de la loi climat et résilience. Avait explicitement refusé ce rapport obligatoire de de compatibilité. C'était dans le texte sorti de CMP c'est un décret qui mais la compatibilité. Nous sommes dans la prise en compte dans le texte sorti de CMT c'est pourquoi Monsieur le Ministre, je l'ai rappelé en complément de ce que monsieur le rapporteur, a dit ça fait évidemment partie des lignes rouges de la CMP, vous l'avez bien entendu nos collègues l'ont rappelé. C'est important de le préciser pour redire peut être très rapidement ben les scotches fixe déjà des trajectoires de baisse de leur consommation foncière depuis bien longtemps. Ils n'ont pas attendu de de ce soir. Contraindre par un un Scott régional bien longtemps disant que les trajectoires de consommation foncière diminue parce que toutes les collectivités ont pris conscience s'applique des Scott Grenelle et ça remonte à quand. À des années de cela des facteurs, 4 des facteurs de beaucoup de territoires sont déjà dans trajectoire de diminution donc voilà on doit trouver la capacité à adopter effectivement une stratégie exigeante et de faire confiance aux territoires pour l'adapter à leurs spécificités. Merci beaucoup madame la présidente. Bon dans sac dans une logique de de subsidiarité. La logique veut que le mouvement soit ascendant. Et que chacune des collectivités puissent exercer son propre pouvoir de façon autonome et sans être lié par par l'échelon supérieur. On a besoin d'une société subsidiaire. Au moment où parfois les choses sont. Trop vertical. À tous égards. Après je pense que le ministre hein quand il dit. C'est le noeud gordien et. Et je ne suis pas favorable. À cet article 2 je pense que c'est pas pour être désagréable et je pense qu'il partage un certain nombre de préoccupations qu'on a tous sur ces bancs. Je pense que son sujet à lui c'est comment s'assurer que mis Boutabout tous les documents fait. Au niveau communal, intercommunal Scott et caetera. Face en sorte quand même qu'on arrive à tenir les objectifs et donc ça veut dire que. Il faut qu'on se prépare aussi dans la suite des travaux parlementaires en vue de la CMP et cetera. Peut être à imaginer un dispositif qui permette de concilier. Cette autonomie des collectivités à décider de leur destin et de leur maîtrise. Du foncier et on l'a vu avec des trajectoires qui sont quand même bien orienté. Et un mécanisme qui permette, si à un moment, on voit que il y a un dérapage, parce que mis Boutabout l'ensemble des documents font que, on est loin des objectifs à ce moment-là, il puisse y avoir des mécanismes de discussion d'arbitrage et cetera mais si c'est peut-être ça qui. Qu'il faudra imaginer travailler à la suite de cet article de. Voilà, c'est le point que je voulais évoquer à cet instant des débats, le président. Monsieur misons. Merci. Dans le président. Monsieur le Ministre. Quelle est la dernière grande compétence stratégique qui reste encore de la main de certaines communes. L'urbanisme. Que c'est dur. Bientôt. Étape par étape. Et avec cet amendement, Monsieur le Ministre. Vous mettez un coup de canif. À la relation de confiance qui prévaut toujours entre la région. Et les communes. Aucune région ne demandent à bénéficier de cette faculté. Aucun élu. Ni. Locaux ni nationaux. Ça a été rappelé par. La la présidente l'état tout à l'heure ne veut de cela et vous. Vous essayez de nous l'imposer. Rappelez-vous Monsieur le Ministre, peut-être êtes vous trop jeune. Du temps des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Quelle est la règle qui s'appliquer et qui n'a jamais posé aucun problème. C'est de la compatibilité. On se parle, on s'écoute, on se respecte. C'est cela que vous êtes en train de mettre à mal et je dois vous demande solennellement de bien y réfléchir. Merci madame la présidente. La semaine dernière. Pendant, dans tous nos longs débats on entendait. Projet de société contre-projet de société. Moi j'ai l'impression, Monsieur le Ministre, qui à 2 visions très différentes de l'organisation d'entrée publique lorsque j'entends les écologistes. Je vois je ressens profondément. Qu'il y a pas de confiance. Envers les élus et qu'il faut donc aspirer remonter. Mais quand on est dans l'aspiration que le remonter. Ainsi, on sait très bien qu'on a un effet technostructure et que nous disent les maires, que nous disent les élus, ils n'en peuvent plus de cette technostructure qui donne, qui leur donne l'impression que la place des élus et sans cesse en retrait et que nous disent nos concitoyens, ils nous disent proximité et que s'est-il passé depuis la loi nôtre la création de ces grandes régions où voyez-vous la proximité dans cette organisation dans ces 13 grandes régions, donc il faut redescendre au plus près des territoires. J'ai j'ai un amendement dans ce sens. Tout à l'heure car je pense que nous ne pouvons pas avoir une organisation d'autres républiques qui Aspire constamment par l'eau donc il me semble que ce qui vous est dit ici avec force, Monsieur le Ministre, c'est que oui, malheureusement. Même en Gironde. Il peut y avoir un jacobinisme régional et voire même un jacobinisme Girondins parce que ce n'est pas l'effet des élus qui siègent à la Réunion. C'est l'effet nems de la technostructure. Que représente, aujourd'hui, par leur taille, les régions issues de la loi d'autres et puis comme l'a très bien dit la présidente de la Commission spéciale il y a là des faits. Ce qui nous. Pose problème puisque nous avions voté un texte qui ne prévoyait pas cette dimension prescriptives. Et on se retrouve si nous n'avions pas vous dire si c'est pas si nous sommes attachés avant tout à la libre administration des collectivités et que vous êtes ici. Retrait de scripts, créer un schéma prescripteurs qui limite la libre administration laisser les territoires s'organiser on parlé de République différencier, il y a peu, nous sommes là dans le contraire de l'indifférenciation que nous souhaitons.

huit, hé bien nous allons suspendre. La séance est suspendue. Elle sera reprise à 21h 30 pour la poursuite de l'examen de ce texte.